La séance est repris j'informe le Sénat que trois candidatures. Pour siéger au sien au sein de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion. Du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 2027 ont été publiés ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie de la santé. Du travail des transports et de l'agriculture. La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.-- La parole je crois est à monsieur le Ministre, qui l'a demandé.-- Merci, merci Monsieur le Président, en application de l'article 44 alinéa 6 du règlement du Sénat, le gouvernement sollicite l'examen par priorité des articles 20 23 et 24 au début de la discussion des articles.-- il y a-t-il un orateur contre. Cette demande de priorité.-- Quel est l'avis de la commission.-- La commission est favorable. La commission est favorable. Donc, je consulte le Sénat sur la demande de priorités présentée par le gouvernement. Qui est donc est favorable.-- Qui est favorable à la demande de priorité.-- Qui est contre.-- Qui s'abstient. Bon donc. Elle est donc. Décidée. Dans la discussion générale. La parole est à. Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Monsieur le président, madame la rapporteure messieurs les rapporteurs pour avis mesdames et messieurs les sénateurs se réunissent cet après-midi afin d'examiner le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie de la santé, du travail des transports et de l'agriculture issus de vos travaux en commission le droit français s'enrichit régulièrement de dispositions décidé conjointement avec les autres États membres. La création d'un cadre européen unifié sur de nombreux sujets permet de mieux protéger et de mieux accompagner nos industries, nos opérateurs et nos concitoyens partout en Europe. Ce projet de loi a pour objet de transposer et mettre en oeuvre un certain nombre de directives et règlements que l'Union européenne a adopté ces 3 dernières années. Il procède également à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union rendue nécessaire. Vous savez que le texte à bord d'un nombre très variée de sujets sur lesquels je ne me prononcerai pas de manière exhaustive à la tribune et laisserait évidemment le débat dans l'hémicycle, nourrir les échanges sur la plupart des nombreux points qui ont suscité votre mobilisation par voie d'amendement. Je veux néanmoins évoquée dès la discussion générale plusieurs points qui revêtent une importance particulière. Au-delà du renforcement de la trique Timité de l'épargne retraite et. Et de la désignation des autorités compétentes pour la supervision et le contrôle du peuple produit européen d'épargne retraite à article Un amendement du gouvernement après l'article de vous proposera définir les règles de fonctionnement et le régime fiscal et social du sous-comptes français de ce produit pour le rendre pleinement effectif conformément au règlement 1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 et au règlement, délégué de la commission du 18 décembre 2020. Et ainsi de préserver les acquis de la loi pacte. Ministre délégué en charge de la transition numérique. Je suis défendra également devant vous. L'article 5, traitant du régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués. C'est-à-dire la blockchain. Figurant parmi les mesures proposées par la Commission européenne en septembre 2020 sur la finance numérique pour stimuler l'innovation. Le règlement européen sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués qu'on appelle aussi DLT entrera en application en mars 2023. Visant à tirer parti des possibilités offertes par l'émergence des cryptoactifs qualifiables d'instruments financiers. Le régime pilote sera mise en place pour une durée de 3 ans pouvant être prolongé de 3 années supplémentaires. La création de ce régime est innovante puisque pour la première fois un texte européen d'application directe autorise certains acteurs de marché à déroger à certaines exigences de la réglementation de droit commun sous certaines conditions. La France s'est battue pour obtenir un régime pilote ambitieux qui permette de conduire des expérimentations à taille industrielle sur les usages de la blockchain. Aussi le règle le gouvernement se réjouit de pouvoir disposer d'un régime créant une zone d'expérimentation pour l'utilisation de la technologie Blockchain dans les domaines des instruments financiers déterminant pour rester dans la course des innovations financières à l'échelle mondiale, avec l'entrée en application de ce régime. La place de Paris va disposer d'une opportunité unique de répondre aux nombreuses questions qui se posent quant au potentiel de la blockchain, ces applications et les synergies que cette technologie pourrait générer. C'est donc une étape La place de Paris pourrait aujourd'hui devenir la place de la mise en oeuvre du régime pilote et en tirer un Avantage comparatif substantiel. Le gouvernement vous proposera cet article 2 amendements qui poursuivent pour le premier, l'objectif de mettre au titre nominatif, en plus des titres au porteur d'entrer dans le périmètre d'application du règlement 858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022. Cette évolution permettra de répondre à une demande que nous jugeons pertinente des acteurs de la place. Le second amendement à cet article 5 vous proposera de modifier le règlement, la réglementation applicable en vue d'organiser la répartition des compétences entre autorités nationales et afin de permettre aux différents types d'acteurs concernés de candidater aux exemptions ouverte par ce régime pilote.-- Je souhaite également évoquer l'article 8 de ce texte dont je sais qu'il a fait débat. Pour des raisons qui honore le Parlement. Mais dont je veux redire ici que les orientations politiques européennes qui en sont à l'origine, ont aujourd'hui été fixé, il n'est donc pas question pour le gouvernement de revenir sur ses arbitrages politiques. En revanche, l'opérationnalisation de ses objectifs requiert un très important et laborieux fastidieux travail technique afin de modifier plusieurs dizaines de pages de code ce travail technique visera le plus haut niveau d'ambition en matière de durabilité, tout en assurant la lisibilité des futurs reporting tant pour les entreprises que pour les investisseurs ou associations souhaitant avoir une vision consolidée des pratiques d'une entreprise. Une habilitation et donc une étape nécessaire pour la bonne mise en oeuvre des mesures de publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises. Le gouvernement espère que les auditions que vous avez pu mener sur ce sujet vous auront convaincus de la pertinence du véhicule retenue afin d'aboutir à sa complète mise en oeuvre. Nous nous engageons à mener ce travail technique en pleine association avec les parlementaires qui le souhaiteront. Je veux également m'arrêter un moment sur l'article 12 de ce projet de loi cet article vise à habiliter le gouvernement à transposer la directive 882, du 17 avril 2019 relatives aux exigences en matière d'accessibilité applicable aux produits et La France comme de nombreux autres pays européens a été mise en demeure de transposer cette directive qui fixe de manière détaillée les obligations que devront respecter les fabricants importateurs et distributeurs de certains produits ou prestataires de service à compter du 20 du 28 juin 2025. La directive de 2019 vise à harmoniser les législations des États pour rendre accessible certains produits et services comme les sites Internet les billetteries les systèmes et équipements informatiques grand public les services bancaires, les livres numériques et commerce électronique. Sur ce sujet important pour nos concitoyens en situation de handicap et pour toute la société. À vrai dire nous accusons un retard que l'équipe qui n'est plus acceptable. Le travail technique, exigeant que cette transposition implique demande la poursuite du travail interministériel d'ores et déjà engagés. Dans cet article une habilitation de quatre mois et demandé je veux cependant précisé qu'un groupe de travail interministériel finalise les écritures législatives de cette transposition afin qu'elle puisse être intégrée par amendement au projet de loi au cours de la navette parlementaire. Le texte contient par ailleurs de nombreuses dispositions relatives aux prérogatives des ministères sociaux. Je pense notamment à l'article 14 qui portent des mesures concernant le congé parental d'éducation. Le congé de paternité. Le congé de solidarité familiale et de proche aidant. Je sais que vous êtes investi sur cet article en commission Madame la rapporteure. L'article 23, quant à lui permet de ratifier des ordonnances désignant l'autorité administrative chargée de prononcer des sanctions financières dans le cadre de la surveillance du marché des dispositifs médicaux des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de leurs accessoires et de leur produit de l'annexe 16 du règlement de l'Union européenne. 2017 745. Là aussi, je sais que la commission des affaires sociales à travailler à l'amélioration des outils de lutte contre le risque de rupture de dispositifs médicaux et à la possibilité de publier les éventuelles sanctions financières prononcées par l'autorité administrative en la matière. Enfin le projet de loi comporte un certain nombre de dispositions relatives au secteur des transports dont je note qu'elles ont suscité une mobilisation particulière de la chambre haute, ainsi que de nécessaires mesures d'adaptation du code rural et de la pêche maritime à la mise en oeuvre de la programmation 2023 2027, de la politique agricole commune dont vous savez qu'elle est un outil vital pour pour nos agriculteurs je vois. Merci, monsieur le Ministre, dans la suite de la discussion la parole et tu as la présidente Pascale Gruny, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur

Monsieur le président. Mesdames et messieurs les ministres, messieurs les rapporteurs pour avis, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mes chers collègues. Au sein de ce texte aux dispositions très diverses qui n'ont pour point commun que d'assurer la mise en conformité du droit national au droit européen. La commission des Affaires sociales s'est penché sur les articles qui concernent le handicap le travail et la santé publique concernant le handicap. L'article 12 propose d'autoriser le gouvernement à prendre par ordonnances, les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2019 882 du 17 avril 2019 relatives aux exigences en matière d'accessibilité applicable aux produits et services. Les premiers jalons de cette exigence d'accessibilité ont été posées par la loi du 11 février 2005. Par rapport à la réglementation existante, la directive procède à un double élargissement en rendant obligatoire ces exigences d'accessibilité, un plus grand nombre de produits et un plus grand nombre d'acteurs économiques et ce à compter du 28 juin 2025. L'article 2 de la directive en énumère la liste. Au regard de la technicité des mesures et de la nécessité d'harmoniser les réglementations qui concerne aussi bien le secteur bancaire, que les transports ou la culture, le recours à l'habilitation me semble justifiables compte tenu des retards rencontrés dans l'application des mesures d'accessibilité physique, nous devrons être attentifs au calendrier de mise en oeuvre de ces nouvelles obligations par les opérateurs économiques. Concernant les dispositions relatives au travail. La commission a approuvé l'article 14 qui sécurise les droits des salariés prenant des congés familiaux en ajustant notre droit aux exigences qui découlent de la directive du 20 juin 2019 sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. À l'issue d'un congé de paternité d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale le salarié conservera le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. Les salariés du particulier employeur les assistants maternels et les assistants familiaux employée par des personnes privées pourront bénéficier des congés de proche aidant et de solidarité familiale en outre l'ancienneté d'un an requises pour le bénéfice d'un congé parental d'éducation ne sera plus comptabilisée à la date de naissance de l'enfant de son arrivée dans le foyer. Mais à compter de la demande du congé par le salarié. Dans le prolongement de ces mesures la commission ajouté les périodes de congés de paternité aux périodes de congés assimilée à une présence dans l'entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation entre salariés. La commission a également adopté les articles 15 et 16 qui adapte le droit du travail à la directive du 20 juin 2019 relatives à des conditions du travail transparente c'est prévisible dans l'Union européenne. Cette directive impose aux employeurs d'informer les salariés sur les éléments principaux de la relation de travail en leur transmettant 15 types d'informations dans un délai de 7 à 30 jours la précision de la directive européenne ne laisse presque aucune marge de manoeuvre au législateur pour transposer ses exigences dans le droit national. Nous avons donc approuvé l'article 15, hein, qui prévoit que l'employeur remettent aux salariés un ou plusieurs documents établis par écrit, précisant les informations principales relatives à la relation de travail. J'attire toutefois l'attention du gouvernement sur la nécessité que ces démarches supplémentaires imposés aux employeurs soit applicable et surtout simple il conviendra d'accompagner les entreprises notamment les TPE-PME dans la mise en oeuvre de cette obligation par l'élaboration du document type à remettre aux salariés. Nous avons approuvé la suppression de la possibilité pour des accords de branche, conclu avant 2008 de fixer des durées de période d'essai plus longue que la durée légale. Nous avons également entériné le renforcement de la formation des salariés en CDD ou en contrat d'intérim sur les postes en CDI à pourvoir au sein de l'entreprise. L'exclusion des dispositions de la directive au salarié employé par chèque emploi service pour de courtes durées ou par l'intermédiaire du guichet unique du spectacle occasionnels nous a semblé justifiée. Ces ajustements sont nécessaires et suffisants pour que notre droit du travail soit conforme au droit européen. Concernant les dispositifs relatives à la santé. La commission a globalement pris acte des adaptations mise en conformité de notre droit. L'article 19 tire les conséquences pour les installations de chirurgie esthétique de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt Van bord. Concernant la publicité dans le Champ de santé est aujourd'hui hein si postuler un régime d'autorisation de principe cependant encadré pour des motifs de santé publique et de dignité de la profession. Sur ce sujet, j'estime que l'enjeu est aujourd'hui celui de l'effectivité des contrôles, notamment sur les réseaux sociaux. L'article 20 concerne les denrées alimentaires destinées à des fins médicales des ADF MS. Il s'agit de transcrire de transcrire pardon droit français la dénomination au niveau européen. Ah ces produits très encadré sur leur composition et l'information qui leur est jointe cependant cet article va au-delà du seul changement de terme une distinction est en fait selon les risques présentés par les denrées. La commission a souhaité sur ce point, prévoir un encadrement plus strict des modes de délivrance et renforcer les exigences de contrôle médical. Le gouvernement, profitant de cette adaptation a en outre prévu un changement de la distribution d'une partie de ces aliments. Les produits distribués aujourd'hui principalement par la forme à la pharmacie centrale de l'AP-HP pourrait désormais être délivrés en officine. Cette modification qui me semble recevable a cependant fait naître de vives inquiétudes auprès de patients atteints de pathologies du métabolisme. Je souhaite que le gouvernement puisse au cours de la discussion du texte. Apporté des garanties quant aux capacités de distribution de l'ensemble des spécialités mais aussi rassurer sur les conditions de prise en charge qui n'ont pas vocation à être modifié l'article 21. Adapte le dispositif national de déclaration de la composition des mélanges dangereux par les industriels au système européen de déclaration unique créée en application des dernières modifications du règlement dit CLP de 2008. Ce portail a l'Avantage de dispenser les industriels de remplir autant de déclarations qu'il existe deux pays où se déploient leur activité. Mais il a vocation à remplacer notre portail national qui alimente depuis 12 ans la base des centres antipoison qui peuvent avoir à connaître de ces produits à des fins préventives ou curatives. L'article 21 réécrit en conséquence les dispositions adéquates du code de la santé publique et du code du travail. L'article 22 adapte le droit français au paquet médicaments vétérinaires adopté en janvier 2019. Il s'agit d'une part de ratifier l'ordonnance du 23 mars 2022, qui a récemment adapter notre droit à ces nouvelles règles européennes et d'autre part de tirer les conséquences d'une nouvelle répartition des compétences entre l'cessent et les directions départementales de la protection des populations. Lesquelles récupère la gestion des établissements de fabrication d'aliments médicamenteux. L'article 23 vise à adapter le droit national au règlement européen relatif aux dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, entrée en vigueur, récemment il ratifie pour cela 2 ordonnances prises par le gouvernement en 2022 pour apporter au code de la santé publique. Les modifications nécessaires et porte directement des dispositions relatives notamment le pouvoir de sanction de l'administration des douanes qui n'avait pu être incluse dans les ordonnances ces règlements permis d'harmoniser les normes applicables dispositifs médicaux d'améliorer leur sécurité et de renforcer la transparence du marché. C'est pourquoi la commission a adopté l'article 23 en y ajoutant toutefois des dispositions qui visent à nous permettent de lutter plus efficacement contre les pénuries des de dispositifs médicaux et de mieux anticiper les ruptures. Enfin, l'article 24 soumet les pharmacies d'officine à une pénalité financière en cas de manquement à leur obligation de sérialisation des médicaments. Cette opération qui garantit l'usage unique des boîtes de médicaments est une obligation européenne depuis février 2019 mais le taux de pharmacie connecté au système qui permet de la réaliser vient tout juste de dépasser 50%, alors qu'il est plus proche de 80% en moyenne. Ailleurs en Europe. En conséquence, la Commission européenne fait peser sur l'état français. La menace d'une sanction pour manquement de l'ordre de 300 à 400 millions d'euros. L'Arctique reprend le dispositif que nous avions voté dans le Plfss pour 2022 mais qui avait été censuré par le Conseil constitutionnel optionnel. À ceci près qu'il rend la pénalité forfaitaire. C'est sans doute une bonne solution pour rendre la menace claire et facile à prononcer, par les équipes de l'assurance maladie et donc de nature à mettre davantage d'officines en conformité avec la réglementation au nom de la commission, je vous invite donc à adopter ce projet de loi dans la rédaction qui résultent des travaux de nos différentes commissions. Je vous remercie. Merci madame la présidente. Et je donne maintenant la parole à. Monsieur Laurent Duplomb, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. C'est le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La commission des affaires économiques s'est vu délégué par la commission des affaires sociales. 2 articles agricole de ce projet de loi du. Ils sont plus technique que politique. Le 30, l'article 30 corrige notamment une incohérence du code rural à propos des aides à l'installation des jeunes agriculteurs. Le 31 ratifie huit ordonnance qui en des domaines très variés adapte le code rural au droit de l'Union européenne. Je suis chargé en tant que rapporteur de vous donner la position de la commission sur ces 2 articles. Concernant l'article 30. Cet article rend sans équivoque la possibilité de décentralisation des aides à l'installation. au terme d'une ordonnance de janvier 2022, les mesures n'en surface du Feader seront transférées aux régions qui les demandent, pour la programmation 2023 2027, de la politique agricole commune. Je pense que le Sénat tout entier. Salut. Le principe de cette réforme.-- Pour l'accompagner. La commission a adopté mon amendement demandant un bilan annuel. Par région, consolidé par l'État à l'échelle nationale. De la politique de transmission et d'installation ce bilan permettra de se réunir, de se prémunir contre 3 dérives potentielles. La première, un manque de lisibilité des aides pour les agriculteurs. La deuxième l'accroissement des disparités entre régions chacune ayant des priorités politiques différentes et enfin la 3ème. Un manque d'efficacité, elle se prémunir à contre un manque d'efficacité si des comparaisons n'encourage pas une saine émulation. L'installation est de première importance pour notre agriculture, et il n'est pas envisageable que l'État ne garde pas un oeil dessus. La commission a en outre entendu. de dans la loi la condition d'une capacité professionnelle préalables pour bénéficier des aides à l'installation, préférant les installations viable au projet mal ficelé. Comment en effet prétendre réussir une installation sans un bagage technique minimal en agro en agronomie en biologie ou en gestion d'entreprise. On ne peut pas demander aux agriculteurs de respecter un nombre sans cesse croissant de règles et d'injonction et en même temps laisser passer des installations, sans formation nous ne confondre ont pas vitesse et précipitation. Chasse, s'agissant de l'article 31. Je m'attarderai surtout sur la méthode. En effet, sur le fond je vois 5 bonnes raisons de ratifier les huit ordonnance. Premièrement, elle relève du droit en vigueur, puisqu'elles produisent dès leur publication des effets assimilable à la loi, les modifier serait source d'insécurité juridique. Deuxièmement elles adaptent le droit à des règles européennes d'application directe. Notre marge de manoeuvre est plus limitée que dans le cas d'une transposition de directives se fait de ce fait ses ordonnances relève du toilettage technique. La France a été à l'initiative de plusieurs dispositions européennes justifiant les ordonnances et Amber à un bénéfice par exemple par la reconnaissance de la mention produit de montagne. Les sols sur-transposition qui maintiennent des standards plus élevés en matière de catégorisation des maladies végétales et animales et de sélection végétale et animale. Apparaissent justifiée par un motif d'intérêt général suffisant. La performance sanitaire et économique de notre agriculture en dépend. La ratification n'empêche pas de faire preuve de vigilance dans le contrôle de leur application. Le président de l'Ordre des vétérinaires m'a par exemple indiqué que la libre prestation des services. Donner lieu à certaines pratiques d'optimisme d'optimisation fiscale réglementaire voire sanitaire. Mais sur la forme, les conditions dans lequel ces ratification sont proposées au Parlement ne sont pas satisfaisantes, à plusieurs titres. D'abord nous avons disposé d'un temps très limité pour examiner Dadu. Ensuite les articles propose la ratification de huit ordonnance alors qu'un texte de ratification en contient en moyenne pas plus de trois.-- Et le caractère disparate du texte nui à l'exercice à l'exigence de clarté et de sincérité du débat. Enfin, et pas des moindres, la ratification de ce texte en propose.-- Plus de 5 ans et trois mois en moyenne après leur publication. sur le précédent quinquennat ce délai était en moyenne de un an, un mois et sept jours soit 5 fois moins pour être plus précis pour cinq ordonnance datant de 2015, la ratification interviendra carrément de. Après leur publication un découplage d'une telle ampleur et quasiment inédit.-- D'autant que les textes européens j'ayant justifié ces ordonnances remonte encore plus loin. Car pour la, pour le plus ancien, il est de 2005. L'examen au Sénat intervient donc à contretemps.-- Près de 17 ans après. Le véritable débat et ont eu lieu au sein du Conseil de l'UE de l'UA et au Parlement européen il y a plus de 10 ans pour certains textes.-- Donc il est vrai que ce délai à mon sens est beaucoup trop important. Voilà en ces quelques mots ce que la commission des affaires économiques voulait vous dire sur ce texte, Monsieur le Ministre, merci. Merci monsieur le rapporteur. Et je passe maintenant la parole à Cyril va rapporteur pour. Avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis un avis favorable à l'adoption du projet de loi, sous réserve des amendements adoptés à son initiative sur les quatre Arctique relatif au transport qui relevait de ses compétences. Avant toute chose elle a unanimement regretté les délais d'examen ça été rappelé imposé pour l'examen de ce texte qui malgré son caractère extrêmement technique emporte des conséquences très concrètes pour nos concitoyens. D'une part et pour les professionnels du c'est du secteur des transports. D'autre part. Sur le fond, la commission a veillé à enrichir à compléter la transposition de la directive Eurovignette relative à la taxation des véhicules lourds empruntant certaines infrastructures routières. Elle a adopté plusieurs amendements visant à relever l'ambition du texte en faveur de la transition écologique et à accompagner les transporteurs dans leur verdissement de leur flotte.-- 99% de la flotte de poids lourds fonctionne au diésel. Le défi de la décarbonation pour ce secteur est donc considérable. La commission a par ailleurs regretté le caractère incomplet du projet de loi initial qui se cantonnaient à transposer la directive Eurovignette au seul des futures concessions autoroutières et ne prévoyait pas de mise en conformité de l'ordonnance relative à l'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises par la collectivité européenne d'Alsace. Avec le droit européen revisité.-- Dans la continuité de ses travaux précédents et notamment de l'examen du projet de loi de ratification de cette ordonnance. Elle a donc adopté l'article 26 Bis qui vise à remédier à cet oubli fâcheux. Nous ne saurions accepter Monsieur le Ministre qu'une telle modification passe par la voie de l'ordonnance. Alors que c'est l'objet même de ce projet de loi que de transposer la nouvelle version de cette directive et que la navette parlementaire sera l'occasion d'ajuster le dispositif si cela s'avérait nécessaire. S'agissant de l'article 28 relatifs aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires, la commission a souhaité d'une part mieux garantir les droits des personnes handicapées ou à mobilité réduite. D'autre part elle a cherché en conformité avec le règlement européen en la matière a reporté la date d'application de certaines de ses obligations. Afin de ne pas entraver le bon déroulement d'ouverture à la concurrence et de ne pas créer d'inégalités entre les voyageurs, selon qu'ils choisissent ou non l'opérateur historique.-- La commission de l'aménagement du territoire et de développement durable a enfin souhaité ratifier une ordonnance de transposition de la directive relative aux installations de réception portuaire pour le dépôt des déchets des navires dans le prolongement des recommandations du groupe de travail sur la modernisation des méthodes de travail du Sénat. Moi, si monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les principaux éléments que je souhaitais porter à haute attention au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Je vous remercie. Merci monsieur le rapporteur. Et je passe maintenant la parole. Au président Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission des finances. Monsieur le président, Monsieur le Ministre. Mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le gouvernement nous présente aujourd'hui un nouveau projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne. Un an après le précédent. Il nous a saisis dans des délais particulièrement contraint puisqu'il a déposé son projet de loi le 23 novembre, alors que nous examinions le la loi de finances. La commission des finances dispose d'une délégation au fond sur neuf articles les articles hein à huit et l'article 13 qui porte sur des sujets très différents. 5 articles sont des demandes d'habilitation. Le Sénat, appréciant peu les ordonnances. Monsieur le Ministre, je me suis donc attachée à vérifier qu'elles étaient suffisamment circonscrite qu'il n'était pas possible de les transposer en dur et que les délais proposés nous permettait de respecter nos obligations européennes. J'ai dit que, dans plusieurs cas, c'est le retard pris par le gouvernement pour transposer des directives ou pour adapter notre droit à celui de l'Union européenne qui conduit ce même gouvernement a demandé des habilitations et exigé du Sénat en première lecture des des. Nous obliger à une première lecture dans des délais très contraints, comme je l'ai dit. Pour ce qui concerne la présentation des articles j'insisterai uniquement sur ce qu'ils doivent retenir notre attention dépasserait plus rapidement sur les autres par manque de temps. Les articles 1 2 4 5 6 et 13 interviennent dans les domaines assurantiel bancaires ou des marchés financiers les relève avant tout de dispositions techniques. Après un examen approfondi, elles n'ont pas soulevé de difficultés particulières et ont fait l'objet de deux amendements rédactionnels en commission. L'article 3 corrige une erreur de sur-adaptation du droit interne qui a conduit à appliquer à l'ensemble des entreprises d'assurances mutuelles institutions de prévoyance. L'obligation de publier des informations en matière de durabilité. Vous m'autoriserez, monsieur le ministre a rappelé à cette occasion que dans le cadre de l'examen de la loi énergie-climat, le Sénat avait supprimé l'article transposant le règlement européen en ayant déjà relevé qu'il excédait les exigences européennes et c'est le gouvernement qui l'avaient réintroduit dans le texte. Le gouvernement se rend compte aujourd'hui que comme souvent le Sénat avait raison. Les articles 7 et 8 qui concerne les entreprises sont ce qui soulève les enjeux les plus importants. L'article sept porte une demande d'habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer la directive du 24 novembre 2021 relatives à la communication par certaines entreprises et succursales d'informations relatives à l'impôt sur le revenu des sociétés. Sur ce sujet. Je regrette que le gouvernement n'ait pas choisi comme il aurait pu le faire la transposition en dur. Il disposait en effet d'un an pour s'y préparer. De surcroît, nous n'avons pas pu obtenir. Monsieur le Ministre des informations que nous demandions sur 2 questions importantes concernant les obligations déclaratives des entreprises et la définition de la clause de sauvegarde. En conséquence, nous ne pouvons pas accepter l'habilitation et je proposerai un amendement de suppression. L'article lui huit porte lui aussi une demande d'habilitation du gouvernement cette fois-ci pour transposer la directive dite c'est SRD relative à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises. J'attire votre attention sur le fait que la directive n'a été définitivement adopté par le Conseil que la semaine dernière et n'a pas encore été publié au Journal officiel. Ce qui est assez inhabituel. Par ailleurs, la demande d'habilitation était particulièrement large. Dans le texte déposé avant la modification de l'article 8 par notre commission. Le gouvernement nous demander de lui permettent de prendre toutes les mesures qu'il jugeait utile sur les obligations sociales et environnementales des entreprises. Il s'agit là d'un périmètre tout à fait démesurées qui excède très largement celui de la directive, nous avons donc restreint en commission l'habilitation au seuls domaines dans lesquels la législation française ferait doublon avec les nouvelles s'obligations de la directive c'est Pour terminer, j'évoquerai rapidement le sujet de l'encadrement des prestataires de services sur actifs numériques Les P S A N.. La faillite de la société FTX et ses conséquences, tant sur les investissements particuliers que sur les acteurs financiers doivent nous inviter à la plus grande vigilance. Nous proposerons donc un amendement pour prévoir l'obtention d'un agrément et non plus simplement d'un enregistrement beaucoup moins exigeant mais nous en reparlerons tout à l'heure à l'occasion de les examens de l'amendement que je vous présenterai. Je vous remercie de votre attention. Merci. Bien sur, le rapporteur et je passe maintenant la parole à Didier Marie, rapporteur pour avis de la commission des lois. C'est le président, Monsieur le Ministre. Chers collègues, pour commencer je souhaiterais à mon tour souligner que les délais laissés au Sénat pour l'examen de ce projet de loi ont été particulièrement contraint et que cette façon de procéder n'est pas acceptable dans une démocratie respectueuse des droits du Parlement, a fortiori pour un texte technique impliquant le temps de l'expertise nécessaire à l'appréciation des directives à transposer. La commission des lois a été saisie de 6 articles du présent projet elle lui a apporté des modifications de nature à mieux ajustée aux spécificités de notre droit interne les objectifs fixés par les directives à transposer. L'article 9 du projet de loi vise à limiter le gouvernement a transposé par Ordonnance la directive du 27 novembre 2019 sur les fusions scissions et opérations transfrontalières cet article appelle trois observations. En premier lieu et il pose une question de méthode les habilitations à légiférer par ordonnances doivent demeurer une exception, compte tenu de l'existence d'un avant-projet d'ordonnance en cours de finalisation et de l'échéance proche pour transposer la directive au 31 janvier 2023. La commission a décidé de réduire le délai de l'habilitation du gouvernement à trois mois au lieu de 6. En 2ème lieu, la directive permet de faire un choix de transposition concernant la participation des salariés au sein des organes de direction de la société. Lorsque les représentants de salariés représentent plus de 30%. Des membres de l'organe de direction l'État-membre peut choisir de limiter cette proportion à 30% maximum. La commission des lois a estimé qu'une telle option était défavorable aux salariés et a donc supprimé la possibilité offerte aux gouvernements de lever cette option. En 3ème lieu, la directive qui instaure un contrôle de légalité. Anti-abus et anti-fraude permet aux États membres de choisir l'autorité en charge de ce contrôle. La commission a confié la mission de contrôle préalable d'une opération transfrontalière au greffier du tribunal de commerce, en raison notamment de leur expérience en matière de fusions transfrontalières de la volonté exprimée par ces professionnels d'exercer ce contrôle et enfin de leur statut d'officier ministériel. L'article 10 du projet de loi vise à modifier les dispositions du code du commerce qui prévoit une possibilité de dissolution judiciaire d'une société par actions dans le cas où ses capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié de son capital social. Cette sanction correspond à une surtransposition de la directive du 14 juin 2017 relative au droit des sociétés. Le projet de loi propose de remplacer la dissolution par l'obligation d'apurer les pertes au moyen d'une réduction du capital social jusqu'à un minimum qui serait fixé par décret en Conseil d'État. Cette modification maintient ainsi une double sanction mais dans un délai plus long. Elle est apparue à la commission des lois justifié à l'aune des conséquences économiques des crises récentes ainsi que des nouvelles modalités de financement des sociétés qui s'appuie de nos jours, principalement sur l'endettement. J'viens désormais à l'article 11 relatifs aux droits de la commande publique. Cet article étant aux infractions pénales les plus graves, la possibilité pour les opérateurs économiques sanctionné en ce sens de démontrer leur fiabilité en prenant des mesures concrètes afin de pouvoir soumissionner malgré une En ce sens ce mécanisme de régularisation affaiblit considérablement l'effet dissuasif de ces peines qui peuvent pourtant être prononcées pour des infractions allant jusqu'à la traite des être s'humains. Si les directives européennes de 2014 nous impose la transposition de ce mécanisme de régularisation en droit interne. La commission a néanmoins compléter le dispositif initial en inscrivant dans notre législation le principe selon lequel les mesures concrètes prises par l'opérateur économique font l'objet d'une évaluation tenant tenant compte de la gravité de l'infraction commise. Cette précision reprend les termes des directives et contribuerait non seulement à préserver le caractère dissuasif des peines d'exclusion des procédures de passation des marchés publics, mais également d'améliorer la lisibilité du droit de la commande publique cette évaluation ayant été présenté par les services du gouvernement comme implicite, ce qui ne peut satisfaire les législateurs que nous sommes. Enfin la commission des Lois s'est penché sur la transposition de la directive du 20 juin 2019 relatives à des conditions de travail transparente et prévisible dans l'Union européenne s'agissant des agents publics, les trois versants de la fonction publique. L'article 17 du projet de loi vise à transposer dans le droit de la fonction publique, l'obligation pour les employeurs d'informer les travailleurs des éléments essentiels de la relation de travail pour cela un droit pour tout agent public à recevoir de son employeur communication les informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions seraient consacrés dans le code général de la fonction publique. La liste des éléments précis qui seraient communiqués aux agents publics ainsi que les modalités de cette communication serait déterminée par un décret en Conseil d'État qui renverrait lui-même à un arrêté établissant les modèles des documents que les employeurs remettrait aux agents. Je rappelle que les États membres avaient jusqu'au premier août 2022 pour transposer la directive. Si bien que la France est déjà en retard de plus de 4 mois. Il est cependant permis de s'interroger sur la valeur ajoutée du nouveau droit à l'information ainsi créé. Au-delà de la simplification opéré pour les agents. Une fois que les mesures d'application auront été prises. Il conviendra également d'évaluer la charge de travail supplémentaire. Induite pour les employeurs. Je vous proposerai d'adopter ces six Arctique, telle que modifiée par la commission des lois. Je vous remercie de votre attention. Merci monsieur le rapporteur. Et je passe maintenant la parole à au président Jean-François Rapin, au nom de la commission des affaires européennes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Depuis 4 ans. La commission des Affaires européennes, assure une mission de veille pour prévenir les sur-transpositions de textes européens dans le cadre de l'examen des projets et propositions de loi comportant des mesures de transposition en droit interne 2 directives ou des mesures d'application de règlement européen. Elle formule des observations en tant que de besoin, c'est-à-dire. Lorsqu'elle constate qu'il est proposé d'aller au-delà de ce qu'impose le droit européen sans justification documenté ou recevable. L'enjeu est ici de préserver la compétitivité de nos entreprises. Cette mission d'abord mise en oeuvre à titre expérimental a été consacré en 2019 à l'article 73 sex IS du règlement du Sénat. C'est dans ce cadre que j'ai saisi la conférence des présidents qui a décidé de consulter la commission des Affaires européennes sur le projet de loi que nous examinons aujourd'hui. Quelques remarques. Tout d'abord pour relever que le gouvernement propose une démarche de transposition sectoriel par un véhicule dédié ce qui permet en principe de mieux identifier les risques de sur-transposition pour autant la brièveté des délais d'examen et ça a été soulevée largement ici et la très grande diversité des sujets abordés n'a pas facilité le travail d'analyse et la coordination entre les commissions, y compris celle que je préside. Deuxième observation les modifications qu'il ait proposé d'apporter au droit interne sont d'importance inégale. Parmi les plus significatives, la commission des Affaires européennes a notamment relevé la suppression d'une surtransposition qui résulte du choix d'une option plus exigeante ouverte par une directive de 2017. En cas de perte grave du capital social souscrit.-- La commission des lois sur le rapport de notre collègue Didier Marie s'est prononcé favorablement sur l'opportunité de cette démarche. 3ème observation plusieurs transpositions sont tardives et le seront plus encore dans le cas où le gouvernement demande à procéder par voie d'ordonnance avec des délais d'habilitation allant au-delà du calendrier prévu par le texte européen. 4ème observation, il est proposé de recourir à des ordonnances dans 7 cas, le gouvernement motivant ce choix dès lors qu'il s'agit de transposer des textes techniques qui n'ouvre pas de marge de manoeuvre et dont la transposition en droit national exige des mesures d'adaptation et de coordination ainsi que la définition de modalités de modalités d'application outre-mer. Telle n'est pourtant pas le cas de l'habilitation sollicité à l'article 8 pour la transposition de la directive concernant la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises dites. Dès, qui a tout particulièrement retenu l'attention de la commission des Affaires européennes. Je rappelle qu'en 2017, l'ordonnance de transposition de la directive N. F RD qui a précédé la nouvelle directive avait introduit des dispositions plus exigeantes que celles prévues par le texte européen au motif de l'expérience de la France en matière d'obligation de publication d'informations extra-financière qui résultait de la loi de 2001, dite NRE sur les nouvelles régulations économiques et de la loi Grenelle 2 de 2010. l'habilitation solliciter aujourd'hui pour la transposition de la directive c'est SRD est particulièrement large. Elle permet en effet au delà de la directive de procéder à des modifications des obligations des entreprises en matière d'enjeux, sociaux, environnementaux et gouverne et de gouvernance, comme ça a été rappelé par les différents rapporteurs. Il pourrait en résulter des obligations de transparence renforcée pour les opérateurs français susceptibles d'avoir des effets concurrentiels négatif au regard des autres opérateurs européens. Si la commission des Affaires européennes n'est pas compétente pour se prononcer sur l'opportunité d'obligations additionnelles ou d'une extension du Champ d'application de la directive, il lui revient en revanche d'attirer l'attention sur le risque de sur-transposition que recèle en l'état, l'habilitation sollicité par le gouvernement qui se donne 9 mois à compter de la promulgation de la loi pour publier une ordonnance dont les conséquences pour les entreprises sont loin d'être négligeable. La commission des finances et plusieurs de nos collègues ont identifié cette problématique qui sera discuté lors de l'examen de l'article 8, je vous remercie de votre attention. Merci. Donc nous en avons fini avec les présentations des rapporteurs pour avis et je vais maintenant ouvrir la discussion avec les les groupes et la parole est à madame Cathy ah pour polie pour cinq minutes pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'examen de ce projet de loi d'adaptation droit de l'Union européenne nous rappelle que la souveraineté de notre pays a été confisqué par les traités européens au profit d'une Europe ultralibérale ultralibérale qui applique la concurrence libre et non faussée au sein du marché intérieur, d'une BCE indépendante de tout contrôle démocratique. Cette Europe libérale, qui a dépecé notre industrie et démanteler nos services publics, se rappelle à nous en moyenne une fois par an, avec l'examen de ces fameux d'adultes. Se Dadu a été présenté le 23 novembre dernier en conseil des ministres, et bien en première lecture au Sénat. Comme le note justement la commission des Lois du Sénat la nécessité, voire l'urgence à légiférer pour adapter le droit interne au droit de l'Union européenne ne saurait justifier les délais particulièrement courts laissés par le gouvernement au Parlement et en 1er lieu au Sénat pour mener à bien l'examen du projet de loi pour lequel la procédure accélérée été engagée. J'invite le gouvernement à lire l'excellent rapport de notre collègue député André Chassaigne et de Jean Louis Bourlanges du MoDem sur les méthodes de transposition des directives européennes qui proposait que les lois portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne soit réservé aux cas d'urgence de transposition en lien avec un retard important, voire un précontentieux ou un contentieux ou au cas de transposition de directives techniques identifiés comme ne posant pas de difficultés politiques particulières. Avant de conclure, je suis toujours il faut également veiller à conserver une cohérence thématique au sein de ces lois, fin de citation. En effet, comment pouvez-vous défendent des institutions européennes, dont les décisions sont imposées aux parlements nationaux ou avec des prérogatives tellement limité que notre droit constitutionnel d'amendement n'est tu entraver ce projet de loi renvoie très largement au pouvoir réglementaire du gouvernement puisque sur 31 articles comporte cette habilitation à prendre des ordonnances en lieu et place du Parlement et 10 ordonnances à ratifier à cela, vous ajoutez un peu de renvoie un arrêté une mise en conformité du droit français aux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne et vous avez un texte fourre-tout et indigeste qui ne laisse aucun espace aux parlementaires pour amender ou modifier le contenu de ce texte. Pourtant les ingrédients sont importants. Si nous pouvons nous réjouir des mesures en faveur de l'accessibilité des personnes en situation de handicap et de l'élargissement des congé de proche aidant et de solidarité familiale aux salariés du particulier employeur les progrès sociaux sont bien maigres. L'Europe sociale dont on nous vante les mérites depuis 40 ans hé bien loin. Ce n'est malheureusement pas le calcul de l'indemnité de licenciement des salariés travaillant à temps partiel sur un temps plein et non sur celle résultant du congé parental qui permettra de contrebalancer l'ensemble des mesures de régression sociale de l'Union européenne alors que le gouvernement s'est engagé auprès de la Commission européenne à réduire les droits de l'assurance chômage et à casser notre système de retraite. Ce projet prévoit en son article de comme par hasard de, je cite, d'améliorer l'attractivité de l'épargne retraite individuelle européenne d'un côté le gouvernement annonce le report à 65 ans de l'âge légal à la retraite et de l'autre, ce texte va favoriser le développement d'un produit de retraite complémentaire individuelle réglementé au sein de l'Union européenne. Selon l'alinéa 7 du règlement européen ce marché européen plus vaste des produits d'épargne retraite individuelle améliora l'approvisionnement en font des investisseurs institutionnels et favorisera les investissements dans l'économie réelle. Depuis le départ, le gouvernement mène en bateau nos concitoyens au sujet du déficit du système de retraite plutôt que d'assumer qu'il l'a vendu notre système solidaire auprès de l'Europe en échange des aides du plan de relance durant la pandémie de Covid ce texte caresse les multinationales dans le sens des profits en supprimant l'obligation de publier leurs comptes et en autorisant les entreprises condamnées pénalement à candidater à nouveau pour des marchés publics. Si elles font la démonstration de leur fiabilité. Autrement dit une entreprise condamné pénalement pour fraude fiscale ou pour acte de terrorisme pourra candidater pour des marchés publics si elle s'engage à ne plus commettre de nouvelles infractions. Nous voterons donc contre ce texte de loi. Je vous remercie. merci, et la parole est maintenant. À notre collègue Jean-Marie vont Laerenbergh. Pour l'Union centriste. Monsieur le président. C'est le ministre. Merci cher collègue. Madame la présidente. Madame et messieurs les rapporteurs, chers collègues. Je voudrais tout d'abord saluer la qualité des travaux de nos aussi rapporteur et je limiterai ici mon propos aux Affaires sociales. Nous retiendrons d'abord à l'article 12. Que ce projet de loi vient étendre les obligations issues de la loi de 2005 sur l'accessibilité. À compter de 2025, l'accessibilité s'appliquera également. Aux terminaux numériques. Citons par exemple les distributeurs automatiques de billets des liseuses aussi numérique. Nous avons tous en mémoire. Monsieur le Ministre qu'il nous a fallu voter un report à l'obligation d'accessibilité, prévue initialement en 2015. Dès lors, nous invitons le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour accompagner le nouveau changement afin qu'ils s'opère dans les délais. Ensuite, soulignons les dispositions de l'article 14. Qui vise à permettre aux salariés de conserver le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de son congé familial. C'est ici une avancée importante. Dans la mesure où le droit en vigueur, assure. Aux salariés de retrouver son poste ou un emploi similaire mais il restait muet concernant les droits acquis le groupe Union centriste particulièrement attentifs. À l'extension du congé de proche aidant et de solidarité familiale aux salariés du particulier employeur assistants maternels et assistants familiaux employée par des personnes privées. Nous soutenons aussi par ailleurs l'amendement visant à ajouter les périodes de congés de paternité parmi ces périodes de congés assimilée à une présence dans l'entreprise pour la répartition de la réserve. Spéciale de participation. L'article 15. Impose à l'employeur de remettre aux salariés un ou plusieurs documents précisant les informations principales de la relation de travail. Lorsqu'on augmente les contraintes des entreprises, il convient d'accompagner les plus petites d'entre elles pour s'assurer que la mesure sera effective et donc, nous invitons le gouvernement à mettre des documents type à la disposition des TPE-PME. À l'occasion de l'examen du dernier PLFSS. Nous avons été sensibilisés par le secteur des dispositifs médicaux concernant les nouvelles règles applicables en matière de certification. Et l'embolie des organismes certificateurs qu'ils pourraient certifier les nouveaux dispositifs et recertifier aussi le stock. Le texte de la commission il répond. Répond à cette crainte, bien qu'une prolongation temporaire certification aurait pu envisager pour le stock. Et toujours sur le Champ des Affaires sociales. L'article 24, méritent une attention particulière. En effet, la lutte contre la falsification des médicaments est une nécessité au regard des enjeux de santé. Publique mais aussi une question d'égalité entre les patients, les pharmaciens au sein de l'lui l'Union européenne. L'application de cet article contribuera à augmenter la qualité de la chaîne du médicament le le corollaire de cette ambition pour ce. qui ne respecteraient pas leur obligation de sérialisation et la mise en place d'une amende forfaitaire. Alors Monsieur le Ministre lorsqu'on met en place une sanction à l'encontre de ceux qui ne déclarent pas, encore faut-il s'assurer que la déclaration soit faisable en l'espèce. Au 28 novembre 2022. Seule près de 62% des pharmacies, arriver à se connecter au répertoire de vérification des médicaments cela laisse songeur. Voilà le groupe UC votera ce projet de loi dans la version amendée par la commission, je vous remercie de votre attention. Merci je vais maintenant passer la parole à Stéphane Artano pour le RDSE. Monsieur le président, Monsieur le Ministre. Mesdames, messieurs les les rapporteurs, monsieur le vice-président de la commission. Mes chers collègues. Le projet de loi que nous examinons ou la technicité des sujets ne saurait occulter l'importance des enjeux soulevés n'est autre qu'une loi fourre-tout. Où plusieurs dispositions sont transposées son lien entre elles sa cohérence ne tient en effet que l'adaptation de notre droit national aux évolutions décidées par le législateur européen. Sur la forme, nous avons dû travailler ça a déjà été rappelé dans l'urgence un texte dense, dont les dispositions sont, je le répète très technique de nombreux sujets y sont abordés, l'économie, la santé, le travail, transports et l'agriculture. La difficulté de l'exercice, c'est que quelles que soient les réserves que nous pourrions avoir sur certaines mesures, nous devons être à jour de nos obligations ne présenter aucun déficit de transposition et disposer d'un droit national conforme aux exigences de l'Union. Européenne, le groupe RDSE attaché au projet européen ont ont parfaitement cet argument néanmoins les délais très contraints, imposés pour l'examen de ce texte ne sont pas sans rappeler ce que nous avons vécu pour l'examen du projet de loi de finances, les délais constitutionnels imposés pour le budget ne saurait justifier l'affaiblissement du rôle de notre Parlement. J'ajouterai que chaque recours au 49.3, à l'Assemblée nationale le vide un peu plus de son essence. Pour revenir au fond mon groupe attentif à l'expression législative de la solidarité, ainsi qu'à la protection de nos six concitoyens français et européens se réjouit. De l'emphase placés par ce projet de loi en matière sociale notamment. En particulier dans un pays où 12 millions de personnes, relève d'une situation de handicap, l'absence d'une société pleinement inclusive est une anomalie, une atteinte au principe d'égalité des droits et des chances. L'article 12 de ce projet de loi visant à transposer la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux exigences en matière d'accessibilité applicable aux produits et services doit être un des catalyseurs de l'effort collectif on vers une inclusivité toujours plus du Bic de notre société. Les exigences d'accessibilité élargies à davantage de produits à un plus grand nombre d'acteurs ne devrait être effective à compter du 28 juin 2025. Je rappellerai que sont concernés entre autres fabriquons hein. Auteur distributeurs de produits ou prestataire de service du secteur bancaire, des transports ou de la culture. Néanmoins je partage les inquiétudes de la commission des affaires sociales, estimant que l'enjeu réside davantage dans le calendrier de mise en oeuvre de ces obligations par les opérateurs économiques dans l'obligation et la promulgation de ces nouvelles règles en droit interne. Au regard des retards constatés dans l'application de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Le gouvernement devra être volontaire. Quant à la nécessité de prévoir un régime d'incitations voire de sanction de nature à accompagner les opérateurs économiques dont le déploiement des évolutions techniques nécessaires. L'accessibilité des produits et servi. Par ailleurs, sur le fond de sortie de crise sanitaire d'inflation galopante de défis énergétiques et face à la nouvelle menace qu'augure le une fashion Ouédec Jeanne d'Arc de Joe Biden à partir de 2023. Le projet de loi s'inscrit dans un contexte économique particulièrement tendu. Néanmoins, on peut l'espérer. Le texte. Ce participe par certaines de ces dispositions à la facilitation des échanges ainsi qu'au soutien des sociétés en difficulté. Le groupe RDSE est satisfait dans l'ensemble. Des réponses systémiques que tente d'apporter l'Union européenne à travers ses différents règlements et directives. L'élimination de la surtransposition visé à l'article 10 du projet de loi rentre dans ce cadre, on a fait notre droit national conduit aujourd'hui les entreprises françaises. À faire face à un risque de dissolution excessif et considérablement accru comparativement aux entreprises d'autres États membres. Dans le cas où les capitaux propres d'une société devienne inférieur à la moitié de son capital social. Il était temps que cette singularité française prenne fin. Je souhaitais souligner aussi l'harmonisation de la procédure française applicable avec celle des fusions transfrontalières de l'Union européenne. L'introduction en droit national de ces procédures de scissions et transformations transfrontalières sont des dispositions intéressantes parce qu'elles garantiront la protection des droits des parties prenantes renforcée également par un dispositif anti-fraude et anti-abus. Ont enfin pour terminer, plusieurs de mes collègues souhaiteraient être rassurés quant aux orientations portées à l'article 30 en matière d'aide d'un à l'installation en agriculture à feu aucun celle-ci continuent de toucher leurs cibles dans un souci de flexibilité et surtout d'équité. Mes chers collègues. Malgré ses remarques. Mon groupe est à ce stade, globalement favorable à ce projet de loi, je vous remercie.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame. La présidente, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Ce projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie de la santé, du travail des transports. Et de l'agriculture, porte bien son nom. Quand il est un un agglomérat de mesures n'ayant d'autre point commun que de provenir de l'Union européenne. Je commencerai par formuler deux observations en ce sens relatives à l'écriture de la loi. Premièrement, il me semble que la cohérence, un tel texte est aussi limitée que son utilité est certaine. Mais ces transpositions expéditive du droit européen qui s'apparente à du fret législatif interroges sur la manière de transposer le droit de l'Union. Deuxièmement, il est à déplorer que le Parlement n'est plus disposé que de quelques jours pour examiner ces articles techniques et pour débattre de modification directe entre droit ou de demandes d'habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnances. Les amendements adoptés par les différentes commissions montre cependant toute l'importance du Sénat dans le processus législatif et la qualité de son travail. Troisièmement, à ce titre, je regrette que l'étude d'impact ne comporte pas d'élément de droit comparé qui permettrait de mieux apprécier les solutions choisies par le gouvernement par rapport à celles retenues par les autres États membres de l'Union européenne. Cela permettrait de mieux éclairer le débat et la délibération parlementaire. Pour le reste je procès devrait maintenant à une discussion par thématique du contenu du projet de loi. Concernant le volet transport. L'article 26 du projet de loi vise à transposer la directive Eurovignette. Dans sa version révisée en 2022, qui prévoit de nouvelles obligations en matière de taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières. Néanmoins l'Arctique 26 se borne à transposer ces nouvelles obligations au seul péage des futures concessions autoroutières ils ne modifie donc que les dispositions relatives au péage figurant dans le code de la voirie routière. Cela est insuffisant. En effet, l'ordonnance du 26 mai 2021 relatives aux modalités l'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises au courant hein. Certaines voix du domaine public routier de la collectivité européenne d'Alsace. Obéit. Elle aussi aux règles fixées par la directive Eurovignette. La transposition prévue par le projet de loi initial et dont incomplète. Cette ordonnance prise sur le fondement d'une habilitation prévue par la loi du 2 août 2019 relatives aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace permet à la CEA. D'instaurer une taxe sur les véhicules lourds de transport routier de marchandises empruntant son domaine public routier. En l'état actuel du droit, cette ordonnance appliquent des obligations fixées par la directive Eurovignette. Dans sa précédente version avant la révision de 2022. Elle prévoit par exemple que les taux kilométrique de cette taxe sont différenciés en fonction de la classe euro du véhicule. Or les nouvelles obligations prévues par la directive dans sa version révisée prévoit notamment de remplacer cette modulation par une modulation en fonction des émissions de CO2 du véhicule. Faute de modifications pour mettre cette ordonnance en conformité avec le droit européen réviser la taxe instaurée par l'ACEA risque donc de ne plus être compatible avec les dispositions de la directive. À compter de 2024. Afin d'éviter cette situation et alors que les Alsaciens attendent de la mise en oeuvre cette taxe depuis des années. La commission de l'aménagement du territoire et du logement durable a adopté un amendement visant à rectifier cet oubli et à mettre en conformité l'ordonnance sur l'instauration de la taxe alsaciennes avec le droit européen. Révisé. À l'occasion de l'examen du projet de loi de ratification de cette ordonnance pour laquelle j'avais été désigné rapporteur. Le Sénat avait souhaité anticiper la révision de la directive, notamment en permettant de différencier les taux en fonction des émissions de CO2 des véhicules. Cet ajout n'avait cependant pas été maintenue dans la suite de la navette. À présent la nouvelle directive étant entré en vigueur dans sa version révisée en 2022, l'article 26 Bis elle serait par la commission. La joie du territoire permettra à la CEA, d'anticiper les nouvelles aux obligations de la directive à l'amont de l'instauration de la taxe.-- Concernant le volet finances. Le constat formulé par le rapporteur Hervé Maurey. Interpelle. Un peu plus d'un an après sa promulgation le parlement examine de nouvelles de, des dispositions visant à adopter le droit financier assurantiel bancaire économique pour lequel la France pourrait ne pas respecter les délais requis. Je rejoins le rapporteur et la commission des finances et qui ont adopté des amendements avec l'objectif d'harmoniser les exigences de la et de renforcer le contrôle des dirigeants de des mutuelle en l'alignant sur celui prévu par les dirigeants de sociétés d'assurance et d'institutions de prévoyance. Enfin l'amendement visant à restreindre le Champ d'appliquer de l'. Demandée par le gouvernement pour transposer la directive relative à la publication d'informations en matière de durabilité pour les entreprises est utile car le projet de loi très largement ce qui est nécessaire à la transposition de la directive visés. Concernant le volet de la loi, l'essentiel de transposer en droit interne 2 directives relatives au droit des sociétés et de mettre en oeuvre un règlement en matière de protection de l'enfance. Pour lesquels les apports du Sénat sont notables. La transposition par ordonnance de la directive portant sur les transformations fusions et scissions transporte air des sociétés oblige le Parlement à légiférer dans des délais particulièrement contraint. La directive concernée doit en effet être transposées avant le 31 janvier 2023. Je salue la position du rapporteur. Qui prévoit de restreindre les délais de transposition de la directive à trois mois au lieu de 6. notre il était nécessaire de supprimer l'option prévue par la directive permettant aux États de réduire la proportion des représentants des salariés au sein de l'organisme de direction de la société issue d'une opération transfrontalière susceptibles d'être favorable aux salariés. Par ailleurs il convenait également de confier le contrôle de légalité des opérations transfrontalières, aux greffiers des tribunaux de commerce qui ont, il faut le souligner acquis les compétences certaines en matière d'enregistrement des projets de fusions transfrontalières. Concernant le volet santé. En matière de santé publique, là encore, les mesures sont très hétérogènes de la composition des produits chimiques aux exigences à respecter pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales en passant par le taux de connexion des officines de pharmacies. J'ai pas le problème de l'encadrement de la publicité des activités de chirurgie esthétique. La France s'est mise en demeure depuis 2019 par la Commission européenne sur ce sujet important de santé publique à cause de l'interdiction totale de publicité pour répondre à la non-conformité du droit. Au droit de l'Union européenne, il est proposé de préciser que le retrait de l'autorisation est effectué en cas de publicité en faveur de ces structures contrevenant à l'enjeu de protection de santé publique. Comme l'a souligné à juste titre la rapporteuse de la commission des affaires sociales. Pascale Gruny l'encadrement de la publicité pour les activités de chirurgie esthétique doit être mieux contrôlée par les autorités compétentes l'encadrement doit être aussi déontologique pour les ordres afin de prévoir de prévenir les dérives constatées, notamment ses réseaux sociaux. Concernant enfin le volet social. Les apports de ce texte sont divers. En matière de handicap les apports d'une directive de le 17 avril 2019, vont permettre d'améliorer l'accessibilité à divers produits et services du quotidien. Dans un délai relativement court pour un de ces mesures, applicables. Il faudra veiller à ce que le dispositif soit réellement opérationnel à cette date et que les difficultés de réalisation n'entraîne pas de désengagement. Je pense notamment à ce que soit assurée. La couverture du territoire par les distributeurs pour les En matière de droit du travail, des difficultés pourraient survenir dans certaines entreprises, en particulier les. TPE-PME et surtout celles qui ne disposent pas d'un service de ressource humaine notamment. Chers collègues, vous l'aurez compris, notre groupe approuve la mise en conformité de notre droit avait le droit de l'Union européenne telle que modifiée et améliorée par le Sénat. Les abords du Sénat sont nombreux et nous serons vigilants sur les habilitations donné au gouvernement, je vous remercie.

Économie-Santé travail transports et l'agriculture comme à Sun habitude le projet de loi relatif aux dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne s'intéresse à des domaines d'une importance et d'une amplitude importante encore une fois les délais d'études ont été très court, le texte et pourtant d'une technicité importante les rapporteurs l'ont soulevé à plusieurs reprises, notamment lors de l'étude en commission. Je tiens à saluer le travail de chacun sur ce texte, que ce soit en commission saisie pour avis ou au sein de la commission des affaires sociales à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir. Le contrôle de subsidiarité qu'effectuent les parlements nationaux est essentiel au bon fonctionnement du système dans lequel nous vivons. Disposer d'un droit de regard sur l'action de l'Union européenne. D'un caractère essentiel d'autant plus que le droit de l'Union a vocation à être incorporé dans nos droits internes. C'est ce que nous faisons à travers ce projet de loi. J'ai entendu parfois des remarques sur ce genre de texte et sa nécessité sa temporalité. J'aimerais juste rappeler que nous avons un temps limité pour transposer les directives. Dans le projet de loi actuelle. Elles sont d'ailleurs nombreuses. De plus les règlements sont d'application directe, la mise en conformité de notre droit interne est une étape assez décisive non pas seulement parce qu'elle nous permet de respecter nos propres règles et d'éviter à notre pays d'être mise en demeure voir sanctionner mais aussi parce que nos règles en sont enrichis. Ce qui est positif pour les Français, J'aimais de conditions à l'effet positif de l'incorporation du droit européen au sein du droit français de conditions que le groupe les indépendants défend depuis toujours. La première, ce sont une transposition et une mise en conformité correct dans ce projet de loi. J'ai l'impression qu'il y a moins de rectification pour erreur de transposition ou mauvaise mise en conformité que dans les précédents. Il est vrai que la technicité est importante dans ces cas-là, mais le résultat d'une telle situation n'en demandent pas n'en demeure pas moins dommageable pour les Français et le pays. La seconde condition hé bien sur la sur bien sûr la non surtransposition. Ce fut un véritable problème et je me réjouis que la France se soit améliorée sur ce sujet. Mais cette problématique n'est jamais loin. Et nous devons rester vigilants. il ne me semble pas, en tout cas que dans le présent texte nous y soyons confrontés. Ce qui me permet de faire un point sur le fond du texte, comme à l'accoutumée, le texte est riche et très variée. Je m'attarderai sur certains sujets relatifs aux questions de la Santé et des affaires sociales. Tout d'abord l'article 14 concernant la directive relative à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et dans et qui s'intéresse entre autres au congé parental d'éducation au congé de présence parentale et aux congés pour événements familiaux. Le texte proposé par le gouvernement est enrichi par la rapporteure. Organise des avancées intéressantes et nécessaires pour les salariés et leurs familles. Je salue particulièrement les aménagements et ouverture concernant le bénéfice des congé de proche aidant. Ce sujet est d'importance, ici au Sénat où de nombreux débats ont eu lieu concernant cette problématique. Nous connaissons les responsabilités des proches aidants et leur dévouement. À l'article 23, je me félicite qu'un amendement adopté en commission vise à éviter les ruptures d'approvisionnement des dispositifs médicaux. Indispensable et ceux concernant les diagnostics in vitro, les ruptures d'approvisionnement, tout comme les pénuries de médicaments sont des sujets qui me préoccupe alors que nous vivons d'importantes tensions depuis la crise du Covid. Enfin de manière générale les adaptations au secteur de la santé seront propices à des évolutions positives. En revanche, les précisions les précisions faites par la Commission. Quant à des questions de mise à 9h sont à prendre en considération. Le groupe les indépendants convaincu de l'importance pour notre pays de transposer les directives européennes dans les temps et de mettre son droit interne en conformité avec le droit de l'Union votera en faveur de ce projet de loi, je vous remercie.-- Merci cher collègue. Et je passe maintenant la parole à Jacques Fernique. Pour le groupe écologiste solidarité et territoires. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Ce projet de loi de transposition du droit communautaire et, comme à son habitude très disparates et d'une grande technicité. Il va tout de même avoir des impacts concrets sur la vie des Françaises et des Français. Ce n'est effectivement pas correct d'avoir eu un délai si serré pour l'examiner. Bien sûr le le groupe écologiste salue ses efforts de transposition, sachant que la France a longtemps été parmi les mauvais élèves de l'Europe avec des déficits de transposition important du retard a été rattrapé en particulier avec la présidence française de l'UE mais on regrette. Que cette adaptation du droit communautaire dans notre législation par ce texte soit quand même assez minimaliste. Ainsi, la priorité donnée à la décarbonation des transports aurait pu être plus. Le texte se contente un peu du service minimum 100 couvrir les évolutions nécessaires. Je vais y revenir. Bien sûr, notre groupe salue des avancées sociales du texte qui élargit les exigences d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap qui permet un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée des des parents et proches aidants qui renforce la coopération entre pays européens en matière de services d'aide sociale à l'enfance. Mais ces transpositions reste. Le texte ne prévoit pas de mesures structurelles pour renforcer l'accompagnement à la parentalité pour renforcer l'accès au numérique. Il ne prévoit pas de de stratégie sur l'accessibilité. C'est la demande du Collectif handicap qui regrette de ne pas avoir été associé aux travaux de transposition mon groupe sont soutiendra donc la proposition qui ayant reçu un avis favorable, je l'espère sera votée si ce texte comprend des avancées intéressantes quant congé de maternité et de parentalité. Il faudrait aller plus loin avec un soutien pour un congé parentalité. À l'image de ce que propose l'Espagne. De, de l'ordre de cette semaine en ce qui les concerne non transférables rémunéré à 100%. Sur le volet transport cette adaptation prend en compte pour l'essentiel la révision de la directive Eurovignette. Directive dont le nom consacré depuis longtemps ne correspond plus à la réalité parce qu'il occulte le fait qu'il ne s'agit plus pour l'essentiel de vignettes, mais de taxe kilométrique. Alors que dans nombre de pays d'Europe existe déjà des taxe poids lourds significative qui explique en partie un fret ferroviaire qui est bien plus développé que le nôtre. Nos gouvernements à nous successifs n'ont pas su actionner ce levier de rééquilibrage de la concurrence entre la route et le rail. Ce texte n'impactera donc pour l'essentiel que les péages autoroutiers. À l'exception, ça a été relevé de la future taxe poids lourds alsacienne à ce titre, il est bon que la commission Aménagement territoire développement durable et rectifier le texte pour que la collectivité européenne d'Alsace puisse saisir les nouvelles options européennes ouvertes par cette actualisation, on se souvient que l'Assemblée nationale ne l'avait pas voulu et donc là, le Sénat avait raison et il a encore raison d'avoir modifié le texte en ce sens, il faudra donc ceci dit être vigilant sur ce point pour le réseau autoroutier. Le gouvernement écarte pour l'instant les options de redevance facultative, notamment celles liées à la congestion ainsi que le sur péage possible de financement pour financement des infrastructures de transport. Mon groupe proposera des amendements sens, l'article 26 inscrit de dispositifs permettant de renforcer le principe pollueur payeur pour les poids lourds, ils sont les bienvenus mais encore une fois il est regrettable que le gouvernement n'aille pas assez loin, puisque la modulation et la majoration ne sont applicables qu'aux seuls péages des contrats de concession à venir en excluant les contrats en cours. Le gouvernement fait le choix de différer l'obligation d'internaliser dans les tarifs des péages les coûts environnementaux liés à la pollution ne pas vouloir bouleverser l'équilibre économique des contrats. C'est l'argument, ce n'est pas un notre sens une justification suffisante. Bien sûr, ce report est conforme à la directive, mais il est regrettable au regard de l'urgence climatique. La plupart des concessions autoroutières ne se termine qu'après 2030, on ne peut pas attendre une décennie. Il est urgent d'activer le report vers le rail et le fluvial de réduire la part du transport routier de marchandises comme il est urgent d'ailleurs de nous concentrer sur l'intermodalité avec les plans vélo train c'est aussi. Question, ils en ont aussi question dans ce texte de rattraper notre retard sur la moyenne européenne qui se situe, je le rappelle, entre 6 et 8 emplacements vélo par train enfin mon groupe s'opposera l'habilitation donnée au gouvernement, nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs pour transposer par ordonnance la directive sur la publication d'informations en matière, en matière de durabilité pour les par les entreprises. La directive c'est S RD. C'est une étape importante du Pacte Vert européen qui devra procéder à des choix déterminants. Il est donc essentiel d'assurer sa transposition par voie législative. Malgré ces réserves, mon groupe voit des avancées dans ce texte les votera donc pour. Merci. Et je passe maintenant la parole à Frédéric Marchand. Pour le groupe RDPI. Monsieur le président, Monsieur le Ministre Mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Certains esprits chagrins con par ces projets de loi des voitures balais législatif souvent inscrit à l'ordre du jour par l'urgence en raison de l'approche d'un délai limite de transposition, voire de son dépassement. Cela justifie alors l'addition de plusieurs directives souvent sans grand rapport thématique entre elles dans le cas d'une procédure accélérée, je m'abstiendrai donc de toute surenchère. Certains regrettent même une incursion de l'Europe dans notre cadre législatif à ceux-là. En revanche, je leur dirais que c'est tant mieux. L'Europe, comme l'a indiqué le président de la République à la Sorbonne, il y a déjà 5 ans, c'est notre histoire, notre identité, notre horizon ce qui nous protège. Ce qui nous donne à l'avenir de textes législatifs actuels sont imprégnés de cette idée européenne structuré par exemple autour d'une économie de marché régulé par une politique volontariste et innovante. Je pense aux investissements massifs de France 2030 dont 40% de ce soutien est issu des aides de l'Union des exigences environnementales ambitieuses. Je pense au projet de loi. Relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables qui vise à participer à réduire les émissions de l'Union européenne d'au moins 55% d'ici à 2030, mais aussi en faveur d'une agriculture résilientes stratégique et innovante. Par l'application de notre plan stratégique national qui traduit la PAC 2023 2027. Je pense aussi aux crédits de la mission Agriculture du projet de loi de finances 2023 curieusement rejeté par les 2 travées opposé de cet hémicycle il y a 15 jours. En d'autres termes, il n'est pas opportun d'opposer nos objectifs issue de notre engagement européen dont les directives en sont les actes concrets et les projets de loi qui découlent de cette philosophie européenne dont nous sommes tous en grande partie les garants. C'est donc avec une certaine fierté que je suis ici devant vous pour vous faire part de quelques remarques sur ce 11ème, projet de loi Dadu examiné depuis 2010 un projet de loi certes assez compliqué a scénarisé dans sa globalité, mais qui comporte cependant de très belles avancées en matière de droit du travail d'égalité des droits et d'ambition écologique. Ce projet de loi renforce tout d'abord le droit du travail pour les jeunes pères, aujourd'hui lorsqu'un salarié s'absente dans le cadre d'un congé de paternité

pour les droits que le salarié tient de son ancienneté, plus de droits aussi en matière de transparence et d'information pour les salariés du secteur public. Les articles 17 et 18 consacre ainsi le droit pour tout agent public ou praticien hospitalier de recevoir de son employeur des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions. Concrètement, il s'agira notamment de la rémunération du temps de travail de son droit à la formation ou des modalités de cessation de fonction aussi en matière d'égalité des droits. Le texte prévoit de renforcer la loi de 2005 concernant les exigences d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Cette loi voulue par le père des lois handicap Jacques Chirac avait permis de nombreuses avancées obligation d'accessibilité des transports collectifs et les établissements recevant du public en disant concrétisation du droit à compensation du handicap, création des maisons départementales des personnes handicapées. La directive 2019 882 transposer ici par ordonnances propose d'aller encore plus loin pour cibler un plus grand nombre de produits, un plus grand nombre. Acteurs, je pense, notamment, une meilleure accessibilité des billets des distributeurs automatiques de billets de titre de transport ou les bornes d'enregistrement automatique. Dans le domaine des transports publics ferroviaires justement l'article 27 visent à renforcer les droits des voyageurs en situation de handicap ou à mobilité réduite. Ainsi, à compter de juin 2023, les services régionaux devront porter assistance aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap à l'embarquement et au débarquement des trains.-- Il reste toutefois encore beaucoup à faire. Les commerçants, les restaurants et les transports représentent encore un retard conséquent le métro reste peu accessibles les arrêts de bus rarement. Et moins d'un tiers des gares ferroviaires nationales sont adaptés.-- En matière d'ambition environnementale. L'article 26 vise à encourager un transport de marchandises plus écologique en conditionnant les taxes de circulation au nombre de kilomètres parcourus et quantité de dioxyde de carbone émise des poids lourds cette modulation se substitue donc à celle prévalant en fonction de la classe euro telle que le prévoyait la précédente version de la directive Eurovignette. Ce dispositif vise donc un approfondissement de l'approche pollueur payeur et passe par le développement de mécanismes de tarification ciblée. Enfin dans le cadre du Pacte Vert pour l'Europe et du programme en matière de finance durable. Le Conseil européen a donné il y a quelques jours, son feu Vert définitif à la directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises. C'est l'objet de l'article 8 de ce projet de loi. Concrètement, les entreprises devront rendre compte de la manière dont leur modèle économique influe sur leur durabilité et dont les facteurs externes de cette durabilité comme le changement climatique ou les questions relatives aux droits de l'homme influence leurs activités.-- Ainsi les investisseurs et les autres parties prenantes seront mieux à même de prendre des décisions en connaissance de cause sur les questions de durabilité. C'est une mesure forte pour construire une économie au service des personnes et à renforcer l'économie sociale de marché de l'Union, nous y sommes donc très attachés. Alors forcément la décision du Conseil, elle date du 28 novembre l'encre n'est pas encore tout à fait sèche et il nous est demandé d'agir rapidement par ordonnances mais devant de si grandes avancées pour les citoyens. Alors que le périmètre a été encadré par le rapporteur en commission doit-on vraiment traîné des pieds et affaiblir le dispositif. Pour conclure, mes chers collègues si par définition ce projet de loi de transposition manque un peu de cohérence il est clairement orienté vers plus d'égalité, plus de droits et plus de cohésion sociale. Traduction d'une Europe solidaire et écologique voulue par beaucoup d'entre nous sur ces bancs aussi notre groupe, il sera donc très favorable, je vous remercie. Merci cher collègue.-- Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je suis très heureux de saluer dans la tribune d'honneur du Sénat. La présence de 2 parlementaires albanais monsieur Edouard Chelsea, président du groupe d'amitié Albanie-France, président de la commission de l'économie et des finances de l'Assemblée albanaise et de Madame Ermonela Felag vice-, présidente de l'Assemblée. Albanaise. Ils sont accompagnés par notre collègue Pierre Ouzoulias Président du groupe d'amitié France-Albanie. Cette visite intervient à la fin d'une année importante dans le processus d'intégration européenne de l'Albanie. Après que le 19 juillet dernier une conférence intergouvernementale a officiellement lancé l'ouverture des négociations d'adhésion entre l'Union européenne et l'Albanie Tirana vient d'accueillir le 6 décembre le 1er sommet Union européenne Balkans occidentaux. Dans la région. Mes chers collègues ont votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter à nos amis parlementaires albanais un fructueux séjour et la plus cordiale bienvenue.--

merci chers collègues nous allons reprendre la discussion avec l'intervention de. Madame Michelle Meunier, pour le groupe socialiste, écologiste, Les républicains. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Une fois n'est pas coutume, notre haute assemblée est appelée à examiner un texte législatif de transposition de directives européennes dans notre droit national. La dernière fois que nous nous penchions sur ce type d'exercice. C'était à l'Automne 2021 pour transposer les directives dans le domaine des transports, de l'environnement et des finances à l'époque notre groupe insistait sur les vulnérabilités qui pesaient sur l'édifice européen à 27. À la sortie de la crise sanitaire. C'était il y a un an et ces circonstances déjà exceptionnelles nous paraissent éloignées tant l'actualité politique de notre continent subit désormais le choc de l'invasion russe en Ukraine, à nos portes et ses conséquences énergétiques palpable au quotidien. Dans ce contexte, décliné en lois nationales, l'incarnation du rêve européen de son cadre communautaire revêt évidemment une importance que nous ne saurions négliger. Ce projet de loi composite comme cela a été dit et répété choisi à cette reprises un vecteur habituel pour la transposition, je veux parler du recours à des ordonnances pour bien des sujets cette carte blanche accordée à l'exécutif peut se justifier les directives transposées sont suffisamment. La matière technique. Ainsi le 1er chapitre consacré aux activités d'assurance et d'épargne retraite n'appelle pas de réserve particulière toutefois certains articles recours aux ordonnances pour transposer des dispositions sur lesquelles notre travail parlementaire aurait permis une écriture législatif direct. Ainsi l'article 8 relatif à la publication d'informations en matière de durabilité des entreprises transpose la directive la directive CS RD relatives aux informations extra-financière qui doivent être fournis par les entreprises. Avec mes collègues du groupe socialiste, écologiste et républicain. Nous proposons de ne pas habilité. Le gouvernement, nous avons déjà pu aborder le reporting RSE dans cet hémicycle, notamment lors de l'examen de la proposition de loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Ce sujet est suffisamment sensible pour mériter de croiser nos regards et d'attendre la publication de la directive. Un autre sujet couverts par ce projet de loi appelle une grande vigilance de notre part, je veux parler de l'article 12, cet article transpose une directive relative à l'accessibilité aux produits et aux services pour les personnes porteuses de handicap. Elle aurait dû être transposée avant juin 2022 la France a été mise en demeure, comment ne pas voir un manque d'intérêt de votre gouvernement, Monsieur le Ministre. Pour le quotidien des personnes concernées. Le secteur associatif du Champ du handicap ne s'y trompe pas. Il nous rappelle que la France accuse un retard énorme en matière d'accessibilité universelle. En dépit des textes adoptés et. Attend beaucoup de la transposition dans ce contexte nous législateurs aimerions donc pouvoir exercer ici pleinement notre mission tenir la plume pour écrire la loi afin de répondre aux questions posées et relayer les équipes les inquiétudes qui s'expriment, à savoir des questions sur le contrôle des mesures prises en faveur de l'accessibilité des questions des inquiétudes quant au régime de sanctions qui s'appliquerait aux entreprises, aux administrations ne rendant pas leurs produits ou leurs services accessibles. Il faut entendre aussi une méfiance quant au délais lointain d'entrée en vigueur et une crainte surtout celle que la parole des personnes concernées ne puisse guider la transposition. Voilà pourquoi Monsieur le Ministre, je vous propose de prendre l'engagement devant nous de maintenir le dialogue avec les représentants associatifs, des personnes en situation de handicap. D'autres dispositions du Champ de l'action sociale sont en revanche les bienvenus. La transposition des directives relatives au congé parental ou congé des aidants vont être harmonisées au bénéfice d'employer actuellement exclus notamment ce les salariés du particulier employeur. C'est un pas en avant qu'il convient de saluer, eu égard à la faible attractivité du métier d'assistants maternels. Ma collègue Angèle Préville interviendra tout à l'heure pour poursuivre cette analyse et détaillera les autres dispositifs en matière de transport et au cours de l'examen. Notre collègue Jean-Claude Tissot développera l'analyse des socialistes sur deux articles relatifs à l'agriculture il détaillera les réserves que nous formulons sur la régionalisation de la dotation des jeunes agriculteurs qui fait peser le risque de voir apparaître de fortes disparités de traitement entre les régions, je vous remercie de votre attention. Merci cher collègue. Et je passe maintenant la parole à Michèle Canet. Mais pour le groupe Union centriste. Merci notre collègue le jeu Jean-Marie. Vanlerenberghe tout à l'heure, le groupe de l'Union centriste votera ce texte relatif à différentes dispositions d'adaptation du droit de l'Union Européenne dans notre pays. Tout simplement parce que vous le savez bien, le groupe de l'Union centriste est un groupe aux convictions européennes affirmé et il nous semble important que cela se traduise notamment par des règles de vie et de fonctionnement au sein de l'espace européen qui soient les plus commune possible et donc. Toutes les dispositions qui permettent justement d'avoir des conditions de vie de concurrence qui soit identique, ce sont bien entendu généralement je soutenue par le groupe de l'Union centriste avec enthousiasme au sein de notre de notre hémicycle bien entendu Monsieur le Ministre. Alors ce texte. Cela a été dit par les précédents orateurs il traite de différentes dispositions assez disparates d'ailleurs ce que l'on peut regretter c'est que certaines n'a mis beaucoup de temps à se traduire en fait. Dans notre droit puisque. Certaines directives ont déjà été adoptées depuis très longtemps, il eut été souhaitable qu'elle puisse être être intégré dans notre droit plus tôt mais bon. Aujourd'hui, cela sera fait, je l'espère avec. Nos collègues qui leur. ce que l'on peut regretter un tout petit peu dans ce texte, c'est d'une part que le gouvernement est beaucoup recours aux ordonnances. Alors cet article dans le texte traite du recours aux ordonnances et franchement nous trouvons. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre que cela est beaucoup trop bas, tout simplement parce que si l'on regarde la situation du quinquennat précédent. Un peu moins de 400 recours aux ordonnances, ce qui est tout à fait considérable, 340 ont été effectivement traduite dans le droit mais. Nous nous disons assez clairement ici au Sénat, que nous ne souhaitons pas qu'il y a ce recours aux ordonnances, tout simplement parce que nous voulons notamment éviter qu'il y a des questions de sur-transpositions nous sommes extrêmement vigilants sur le sujet des questions de surtransposition qui. Arrivent et donc le fait de pouvoir à introduire dans le droit dur par les assemblées parlementaires l'essentiel des textes, je crois qu'on court au fait que nous puissions veiller à ce que. Il n'y ait pas ces sur-transposition qui sont toujours. Négatives en tout cas appréciée négativement. Laurent Duplomb. On pourrait parler de l'agriculture par exemple on a tendance à vouloir toujours être plus vertueux que les autres, alors même que cela entame la compétitivité de beaucoup de nos entreprises dont Veillon. Madame la rapporteure à ce que justement. Nous soyons extrêmement vigilants là-dessus et puis. Sur les aspects financiers de ce texte. Je dois ça salué notamment les propositions formulées par le rapporteur de la commission des finances. Notre collègue Hervé Maurey, notamment pour ce qui a trait aux questions de Quito actif aujourd'hui on voit bien que ce sont des dispositions particulièrement. Émergente qui. Suscite l'intérêt de beaucoup de nos concitoyens en France bien entendu, mais dans le monde également, il ne semble qu'il faut quand même être extrêmement prudent avec l'ensemble de ces dispositifs de façon à ce que ça ne se retourne pas contre. L'ensemble des usagers et je dois dire que les dispositions que la rapporteure pour avis a a proposé à la commission des finances vont dans le bon sens, d'une certaine régulation des dispositions pour l'écriture a été fait, donc. J'espère que l'assemblée suivra les propositions de la commission des finances en ce sens. De façon à ce que nous arrivions à une bonne régulation voilà, chers collègues. Les quelques mots que je souhaitais vous dire en titre du groupe de l'Union centriste. En vous souhaitant une bonne après-midi de travail. Merci Monsieur le Ministre Moderna Ministre de votre écoute. Merci et pour dire terminé la discussion générale, je passe la parole à Madame. Angèle Préville pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues de grande technicité technicité ce texte qui nous est soumis, aura des conséquences très concrètes pour les professionnels de transport routier et pour les voyageurs ferroviaires, la marge de manoeuvre dont nous disposons est réduite puisqu'il s'agit d'adapter notre droit interne au droit de l'Union européenne acté l'inscription de ces mesures exigeante est absolument nécessaire car elles permettront de faire avancer la transition écologique dans le transport routier se sont à vrai dire les têtes de pont de futures mesures plus fortes encore, espérons-le. Je rappelle que nous visons une réduction des gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030. Enjeu colossal de responsabilité devant les graves conséquences déjà effective du dérèglement climatique et le secteur du transport représente l'un des l'une des plus importants source d'émissions de gaz à effet de serre 4 articles ont été examinés par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, deux concernent des corrections d'erreurs au sein du code des transports. Je n'y reviendrai pas. Les 2 autres apportent quelques avancées. L'article 26 tout d'abord vise à transposer la directive Mais en l'état actuel du texte, un nombre considérable de véhicules lourds échappera à la modulation des péages routiers en fonction des émissions de CO2 et à la redevance, des coups pour coups externes liés à la pollution atmosphérique puisque le seuil d'application est établie à 3 5 tonnes. Je pense aux véhicules utilitaires légers. Entre 2,5 et 3,5 tonnes dont le nombre a considérablement augmenté ces dernières et je pense aux petits camions bâchés par exemple aujourd'hui il concurrence les poids lourds y compris sur les longues distances, il peut donc en résulter une forme de contournement de l'esprit du dispositif puisqu'ils échapperont ainsi à une possible taxation car le but est bien d'inciter par le principe pollueur-payeur. Au renouvellement du parc de poids lourds en diminuant le prix payé par les moins. Tout en taxant davantage les plus émissifs. C'est pourquoi nous proposerons un amendement permettant d'inclure ces véhicules utilitaires utilitaires légers dans le Champ de la redevance et de la modulation des péages autoroutiers. Cela dit cette modulation aura un impact limité puisqu'elle ne s'appliquera qu'à 235 kilomètres d'autoroute, sur les 9200 que compte notre pays en effet sauf. Seuls les contrats de concession attribué après le 1er janvier 2010 sont concernés. Un petit manque d'ambition, certainement. Il aurait été intéressant en cas de recettes supplémentaires de favoriser le développement du report modal ferroviaire et fluvial indice ça indispensable pour lutter efficacement contre le changement climatique. Nous avons pourtant un réseau ferroviaire et un réseau fluvial extrêmement. Mais quelque peu délaissés et pour tout dire, nous n'en tirons pas de réelle bénéfique écologistes s'agissant maintenant de l'article 28, transposant un règlement visant à uniformiser les obligations pour les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets. Il permet de donner aux voyageurs des informations plus claires renforcent leurs droits notamment en matière de transport du vélo pour le train et d'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite prévoir d'étendre aux services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs l'obligation d'indemnisation en cas de perte ou d'endommagement d'équipements de mobilité comme les fauteuils roulants de dispositifs d'assistance en cas de perte ou de blessures d'un chien d'assistance paraît juste. On ne peut que s'étonner que de telles dispositions ne soit pas acquis pas applicable à présent effectivement nous avons du retard en la matière. Les mesures relatives au transport nous semble donc aller dans le bon sens nous avons soutenu la plupart des propositions du rapporteur lors du travail en commission. Toutefois, nous pensons que des améliorations peuvent être apportées. Nous les nouveaux les soumettront au cours de cette séance en espérant qu'elle puisse obtenir votre soutien je vous remercie de votre attention. Merci cher collègue. Donc la discussion générale est Close et nous allons passer à la discussion de la Commission avant d'entamer la discussion des articles. Mes chers collègues, je vous informe. Que nous suspendrons la séance à 17h 25 afin, afin que chacun puisse prendre place pour la déclaration du gouvernement relative à la politique de l'immigration et le débat qui, qui, en ce qui suivra. Et donc si nous n'avons pas terminé à 17h 25. Nous reprendrons la suite de l'examen du texte ce soir.-- Nous commençons donc par les articles qui ont été appelés en priorité 20 23 et 24.-- Sur l'article un premier amendement le 16 rectifié monsieur Oui monsieur le le président. La Commission de l'alimentation et 42 référencement et de la gestion des ruptures d'offres de de soins et elle pourrait être remplacée par une commission plus large dans les problématiques des maladies rares. Actuellement la mise sur le marché des denrées alimentaires destinés à des fins médicales spécial fait l'objet d'une modification d'une notification pardon, près de la DGCCRF, puis d'une évaluation nutritionnelle par là Ils sont ensuite présentés à la commission nationale d'experts de l'Agence générale des équipements et des produits de santé qui évalue l'intérêt médical de ces produits. Le présent amendement vise à ce que ce soit l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et la commission d'alimentation des maladies héréditaires du métabolisme qui arrête conjointement les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spécial du règlement de l'Union européenne. Je vous remercie.--

de la commission d'alimentation cependant sur la forme. Cet amendement ne satisfait pas l'objectif que vous voulez donner à cet amendement parce qu'il vise en réalité les denrées destinées aux nourrissons. Alors sur le fond. Oui, le passage à une distribution finale va nécessiter de nouvelles inscriptions sur la liste des produits et prestations. C'est pour cela qu'une transition est aménagée à la fin de l'article 20 qu'un maintien transitoire de possibilités étendues distribution en pharmacies à usage intérieur. les mêmes arguments vont servir aussi aux amendements qui qui suivent. Donc pour ces raisons en fait, il me paraît pas opportun de revenir sur la règle d'action qui a été retenu en commission et donc j'émets un avis défavorable.-- Merci. Madame Darrieussecq qui sera. Qui donne l'avis du gouvernement qui sera avec nous pour les articles appeler en priorité.-- Merci beaucoup monsieur le le président. Monsieur le sénateur. Bah j'ai un avis identique à celui de Madame la rapporteure donc je je ne détaillerai pas davantage. Merci madame le rapporteur d'avoir été exhaustif dans cet avis donc avis défavorable.-- Oui merci Madame la Ministre Madame la rapporteure, moi ma préoccupation concerne, vous l'avez compris, les maladies du métabolisme héréditaire et et de manière à ne pas remettre en cause en fait la prise. des malades qui qui qui sont victimes de de de ces maladies et j'entends les arguments qui ont été présentées par Madame la rapporteure et je remercie de cet éclairage. Et en conséquence je retire mon amendement, je vous remercie.-- merci Monsieur Sautarel, vous pouvez rester au micro parce que le suivant et présenté par vous. C'est le 19.-- En fait cet, cet amendement va dans le même sens. Il vise à supprimer l'alinéa 22 de cet article. en fait à supprimer les périodes de transition afin de ne pas perturber le circuit de distribution des denrées alimentaires destinés à des fins médicales spécial suivant le même argumentaire que j'ai développé. En faveur des malades du métabolisme héréditaire, merci.-- Madame la rapporteure.-- Merci monsieur le monsieur le président. Moi je vais mettre un avis défavorable, mon cher collègue. Cet amendement tend à exclure les pharmacies d'officine du Champ des distributeurs autorisés des denrées alimentaires destinés à des fins médicales et réservé ainsi leur délivrance aux pharmacies à usage intérieur cela interdirait la distribution de certaines denrées aujourd'hui déjà délivrés par les pharmacies et comme certains les spécialisé pour nourrissons dont on a besoin de de trouver ça en en proximité cela laisserait seulement les pharmacies à usage intérieur comme seul acteur et dans les faits, la seule AGEPP. Or la JEP appelle elle aussi à la bascule vers le réseau officinale pour les denrées sans risque majeur. Donc c'est un avis défavorable ou un retrait. Merci monsieur le président. Oui. Madame la rapporteure là dit. Ces, ces produits ne se limite pas aux acides aminés aux produits il faut prothétiques. Que vous citez le Champ couvert par cette notion est bien plus larges puisqu'elle couvre aussi bien des compléments nutritionnels oraux les les spéciaux hypoallergénique pour les nourrissons ou encore les produits destinés à la nutrition Terral. À l'aide de pompes donc. L'adoption de votre amendement conduirait à ce que ces produits aujourd'hui délivrés en pharmacie d'officine ne puisse plus l'être demain et ce serait un vrai problème pour les. ayant ayant besoin de ses ses produits. Exclusivement disponible en pharmacie d'officine ou encore. Des produits hyper protides que pour les patients dénutris D A D F Ms destiné aux patients avaient maladies héréditaires du métabolisme. Il est prévu de consulter la filière maladies rares héréditaire du métabolisme et les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé pour définir les modalités de délivrance, les plus adaptées pour ses patients et si à la suite de ces consultations la délivrance par la APEI lui semble la plus adaptée. Alors, nous mettrons en oeuvre cette faculté ouverte par l'avant-dernier alinéa du nouvel article L 51 37 tiré 3 du code de la santé publique. C'est pour ça que je suis défavorable à votre amendement. Monsieur le sénateur.--

vous l'avez bien compris à ce que j'j'ai bien conscience que mon amendement était d'une portée trop large ou plus large que que que la finalité que je défendais par rapport aux maladies du métabolisme héréditaire, mais je pense que c'est un amendement d'appel pour entendre en fait. Les perturbations dans la distribution qui pourrait dégénérer pour les ces malades et sur lesquels effectivement une vigilance particulière devrait être mise en oeuvre et, et j'entends les éclairages. Madame la ministre, et je vous en remercie. En conséquence je retire mon amendement.--

Un alinéa 2 de cet article de façon à à à éviter là aussi une période de de transition mais au regard des des arguments qui ont été développés et compte tenu que les avis j'imagine sont les mêmes que sur l'amendement précédent. Je vais faire gagner du temps à nos débats en retirant cet amendement après avoir entendu les arguments qui ont été développés. Bien merci Monsieur ce est le suivant, qui est le l'amendement 18. Également Même position merci.-- moi je voudrais dire à mon collègue Stéphane Sautarel que c'était aussi important quand même de de défendre et de pouvoir exprimer ici les inquiétudes qui sont sur le terrain, notamment chez chez les patients hé bien entendu aussi les entreprises

Bien merci je vais soumettre aux voix l'article 20. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. Nous passons l'article 23 amendements 44 Madame Imbert.-- Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à préciser les dispositions introduites par la Commission relatives à l'approvisionnement en dispositifs médicaux en prévoyant que lorsque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qualifient elles-mêmes un dispositif d'indispensable ou prend des mesures visant à prévenir une rupture. Elle doit au préalable entendre les opérateurs concernés. La consultation des opérateurs est en effet indispensable pour permettre à l'ANSM d'apprécier le risque de rupture comme ses conséquences sur l'accès aux soins des patients.-- ce sera un avis favorable parce que c'est important effectivement de bien d'inscrire. Cette consultation préalable des opérateurs concernés par la fabrication ou la distribution du dispositif. À l'ANSM qui permet de mieux évaluer le risque de rupture qui est quand même aujourd'hui une une inquiétude sur sur le terrain, donc avis favorable. La. Merci à vie du gouvernement. Madame la ministre.--

Qui est contre. Il s'abstient. Il est adopté. Je suis moins on voit l'article 23, ainsi amendé qui est pour.-- Qui est contre. Qui s'abstient il est adopté, je mets aux voix l'article 24. Qui est pour. Qui est contre. Il s'abstient il était adopté. Nous revenons donc au cours normal de la discussion des articles puisque les 3 articles ont. Appelé en priorité ont été adoptés. Donc je mets aux voix l'article 1er.-- Qui est pour.-- Qui est contre. Qui s'abstient il est adopté. Nous passons à l'article 2 amendements. 68.-- Madame ah pour. Merci Merci monsieur le président, s'est engagé à réformer le système de retraite et à réduire les droits de l'assurance chômage. Le président de la République a annoncé que la réforme des retraites serait présenté le 10 janvier prochain. Mais sans attendre cette date ce projet de loi prévoit à son article de de développer l'épargne retraite complémentaire. Ainsi, selon l'exposé des motifs. Cet article 2 prévoit d'améliorer l'attractivité du produit. Paneuropéen d'épargne-retraite individuel. Le gouvernement souhaite donc développer la retraite par capitalisation au détriment de notre système par répartition. Ce nouveau contrat d'épargne par capitalisation et complémentaire des régimes de retraites publiques et complémentaires. Il est intéressant d'observer qu'actuellement, aucune compagnie d'assurance française ne propose 2 Pepp. Les seuls contrats existants sont commercialisés en Irlande, au Portugal et à Chypre car il est prévu que le régime fiscal du pays d'origine du contrat sera applicable en cas de transfert dans un autre État. Il s'agit donc d'une retraite complémentaire financée par des paradis fiscaux, les PEP cassent notre système. Hé ben oui. Seul, je sais bien que ça vous fait pas plaisir. Cassent notre système solidaire de retraite au profit de fonds d'investissements comme BlackRock installées dans des paradis fiscaux. Pour notre part nous refusons l'expansion des retraites individuelle complémentaire financée par l'évasion fiscale au détriment des finances publiques des États souverains pour ces 2 raisons nous demandons la suppression de cet article, je vous remercie.--

à ce qui nous a été indiqué parce que on ne voit pas bien le lien qui existe entre. Le, le produit d'épargne retraite individuelle et la retraite la le le la réforme des retraites envisagée par par le gouvernement. Peut-être que le ministre nous éclairera. On ne voit pas bien le la la relation, on ne voit pas bien non plus toutes les références sur été faite au paradis fiscaux parce que. Aujourd'hui, en fait ce produit d'épargne retraite individuelle. c'est surtout un un échec retentissant parce que il y a un seul produit qui existe dans toute l'Europe, c'est en Slovaquie. Donc vous voyez qu'on est très loin d'un diktat de Bruxelles. On est très loin de de risques qui serait avéré et si on abroger cet article on on supprimerait en même temps la désignation des autorités compétentes en matière de supervision, ce qui veut dire qu'on arrivera à une dérégulation totale qui à mon avis n'est pas ce que souhaitent les auteurs des amendements donc pour cette raison, c'est une demande de retrait. Monsieur le ministre.-- Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs. Madame la la sénatrice. Oui le le rapporteur a a raison il y a une forme de confusion, puisque dans notre système de retraite, nous avons la retraite socle par répartition, la retraite complémentaire et nous avons un étage supplémentaire qui la retraite supplémentaire lorsque nous avons débattu de la loi pacte. Nous avons rénové cette épargne supplémentaire qui bénéficie d'ailleurs à un grand nombre de de nos concitoyens soit à titre individuel et c'est notamment le cas de nos concitoyens qui, qui sont des travailleurs indépendants, soit Tite collectif dans des produits qu'on appelle le perco par exemple c'est-à-dire sous la forme d'abondement de leur employeur, la constitution d'un supplément de retraite. Ce que vient faire. Cet article. que le le le le le le la version française de du produit d'épargne retraite européens puisqu'il y a une vue il y a une vocation européenne à ces produits d'épargne qui doivent pouvoir suivre les citoyens européens tout au long de leur carrière, même quand ils vont travailler dans un autre État-membre hé bien De manière conforme aux caractéristiques qu'on lui a donné, quand on a débattu de la loi pacte et de nous assurer que lorsque. Tout au long de sa carrière. Un de nos concitoyens va aller travailler dans un autre pays de de l'Union européenne. Que ce ce supplément de retraite qu'il est en train de constituer soit bien préservé, c'est cela que que que l'article 2 accompli. Donc demande de retrait ou avis défavorable.-- Bien un double avis défavorable, donc je suis saisi. D'une demande de scrutin public par le groupe CRCE sur l'amendement numéro 68 avec un double avis défavorable. Il va donc être procéder au scrutin public dans les conditions fixées par la dans l'article 56 de règlement. Le scrutin est ouvert.

Bien plus personne ne demande à voter

Bien plus personne ne demande à voter le scrutin est clos.

qui est pour.-- Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. Un amendement après l'article de le. 40 présenté par le gouvernement Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs effectivement un amendement. Du du gouvernement qui vient fixer les règles de fonctionnement et la fiscalité du sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne retraite individuelle à nouveau le, le plan d'épargne retraite individuelle au niveau européen, a vocation à harmoniser ce ce produit d'épargne supplémentaire qu'on retrouve dans l'ensemble des États en laissant la flexibilité à chaque État membre de fixer les conditions. De son propre produit d'épargne les. L'idée étant que il peut y avoir des différences entre les produits d'épargne ou le le le je dirais les les caractéristiques des produits d'épargne de chaque État membre. Mais, mais qu'il est nécessaire qu'ils puissent converger au sein d'un produit unique pour la protection des des concitoyens européens lorsqu'ils sont amenés à travailler dans un autre État membre de l'Union européenne et c'est ce que cet amendement vous propose.-- Merci à vie de la commission.-- Oui c'est un avis favorable. Il nous paraît pertinent d'aligner le fonctionnement et le et le régime fiscal des 2 dispositifs.-- Il y a un amendement du gouvernement un avis favorable de la commission il y a pas d'explication de vote, je le soumets aux voix qui est pour.-- Qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté. Je soumets aux voix l'article 3. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. Nous passons. Pardon, excusez-moi je soumets aux voix l'article IV. Qui est pour.

sous-Madame Cohen le présente 70 l'amendement 60. Nous souhaitons supprimer cet article qui porte sur le développement de la technologie dite de. Distribué ce sont des plateformes d'un nouveau genre par lesquels les transactions entre participants s'effectue sans intermédiaire d'une entité centrale et sont automatiquement enregistrées sur des serveurs commun. Il s'agit tout simplement d'un moyen de contourner le dépositaire central institution essentielle au bon fonctionnement des marchés financiers qui garantit que les transactions sont exécutés correctement et en temps voulu. il faudrait consacrer l'innovation financière pour permettre des gains d'efficience aux acteurs des marchés. Nous ne partageons pas cette position qui fait porter une menace pas seulement réglementaire comme il est indiqué dans l'étude d'impact, mais qui porte sur la nature même des transactions ce régime pilote sorte d'expérimentation vise à introduire la bloque I'm'sur des transactions côté opération permise que sur du non coté jusqu'alors les principaux risques que nous identifions sont de nature différente. Derrière le souci de démocratisation qui serait accru grâce à ces technologies se cache en réalité une capacité de fractionner à l'envi les titres détenus rendant la détention infinie et sectionne able également diluant le capital et les responsabilités en générant de la confusion pour les entreprises qui s'y adonneraient le mythe de la finance pour tous est une récit elle implique de disposer de capital dont les ménages sont privés, vous en conviendrez cette fausse démocratisation se fera on y assistera sur le temps long, au détriment des autres investissements et également au détriment des produits d'épargne réglementés. C'est ce que nous pensons au niveau de notre groupe derrière cette expérimentation l'objectif inavoué est de créer la connexion entre le mode de la finance traditionnelle et celui des cryptoactifs ce rapprochement à bas bruit avait été tenté en avril 2021 par la plateforme d'échanges de cryptomonnaies Binance les utilisateurs avaient la possibilité d'acheter via des crypto-monnaies pardon dossier à des monnaies réelle une fraction ou l'entièreté d'une action de l'entreprise Tesla ou Apple, par exemple comme le temps mais compter, je vais m'arrêter là mais vous aurez compris que c'est le sens de notre amendement. Merci. Avis du rapporteur.-- du dispositif telle qui était proposé par le gouvernement sans sans aucune modification pour tenter de rassurer, Madame Cohen. Je, je dirais que le régime pilote qui est proposé demeure très encadrée il ne pourra pas être utilisé par les plus gros acteurs. Qui sont exclus de ce régime pilote et qu'en plus, tout ça se s'effectuera sous. L'autorité des supervision nationale et et européennes donc avis défavorable. Avis du gouvernement. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs. Madame la la sénatrice. Oui je suis d'accord avec le le rapporteur et est l'avis du Gouvernement sera défavorable, pourquoi face à des innovations comme celles des des registres distribués, c'est-à-dire de la blockchain. Je crois qu'il faut essayer de se se retenir de de réflexe, le premier serait. De se détourner complètement de toute tentative de de régulation en laissant les choses se faire jusqu'à ce qu'un accident ne survienne. Et l'autre serait immédiatement de sur-régulé quitte à inhiber complètement l'innovation en matière financière, il faut évidemment avoir la main tremblante puisque la place de Paris traditionnellement est une place puissante en Europe et depuis le Brexit s'est considérablement renforcé venant d'ailleurs en terme de capitalisation boursière. La première place financière en Europe.

Et donc, s'agissant de l'application des des registres distribués donc de la blockchain. Aux opérations financières. Le choix qui a été retenu au niveau européen c'est c'est celui d'un régime expérimental d'un régime pilote qui va durer pendant 3 ans renouvelable une fois et qui va permettre de manière encadrée de laisser émerger sous le regard attentif du régulateur, un certain nombre de solutions. Dont nous pourrons juger dans 3 ans si oui ou non elles sont pertinentes et si oui ou non elles serve l'intérêt des Européens des entreprises européennes et des citoyens. Et donc pour cela, il nous paraît très précieux que cet article 5 puissent être conservé en l'état donc avis défavorable.-- Il y a un double avis défavorable je vais soumettre cet amendement voit qui est pour.-- Qui est contre.-- Qui s'abstient.-- Il n'est pas adopté un amendement suivant présenté par le gouvernement le 48. Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les les sénateurs. Par cet amendement. Le le gouvernement vous vous propose. D'amender la rédaction précédente de l'article 5 en étendant ce ce les les possibilités ouvertes pour le par le régime pilote ce régime expérimental. Que j'évoquais à l'instant au titre nominatif. Dans la rédaction précédente de l'article 5. Ça n'était ouvert que pour les titres au porteur.-- Monsieur le rapporteur.-- Oui, monsieur le Président c'est un avis favorable effectivement tout à fait logique et cohérent que ça puisse s'appliquer à la fois aux titres au porteur et aux titres au nominatif.-- Il y a un avis favorable de la commission sur cet amendement du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Il s'abstient. Il est adopté l'amendement suivant le 47 présenté par le gouvernement.-- Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs dans dans ce 2ème amendement du que le gouvernement. Vous propose un article 5 il s'agit de répartir les responsabilités entre les 2 régulateurs que sont l'ACPR d'un côté. Et l'AMF. De l'autre.-- Avis du rapporteur enfin avis de la commission. Oui c'est un avis également favorable. Il nous paraît opportun de prévoir un dispositif d'agrément spécifique pour les infrastructures de marché un recours à la technologie des registres attribué en répartissant cette responsabilité entre l'AMF et l'ACPR donc avis favorable.-- Bien, donc avis favorable de la commission sur cet amendement du gouvernement je le mets aux voix qui est pour.-- Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 5. Qui est pour.

Oui, merci beaucoup monsieur le président. Alors cet amendement. Sur lequel il y aura peut-être un petit peu moins de d'unanimité entre la Commission et et le gouvernement vise à imposer aux acteurs qui exerce la Poste la profession de prestataires de services sur actifs sur actifs numériques PSN d'être agréé au préalable par l'Autorité des marchés financiers à compter du premier octobre 2023. Pourquoi parce que. La faillite récente de la société FTX a mis en lumière les risques inhérents à toute investissements dans les cryptoactifs, la commission européenne ce s'est préoccupé de de cette situation et s'est mise d'accord sur la mise en oeuvre d'un règlement Mica relatif au marché des crypto-actifs mais celui-ci qui prévoira donc un agrément obligatoire comme le propose cet, cet amendement n'entrera en vigueur qu'au mois d'octobre 2024, avec une période transitoire. Qui de 18 mois pour les les entreprises qui auront déjà été enregistrés et qui donc, conduira à ce que cet enregistrement obligatoire finalement il ne soit une entrent dans les faits qu'en mars 2026

des marchés financiers. Nous proposons d'anticiper la mise en place de ce dispositif d'agrément et de le mettre en place à partir du, du premier octobre 2023, j'indique qu'aujourd'hui en France aucun. PSA and a demandé son agrément et il n'y a qu'une, une soixantaine d'entreprises qui en revanche sont enregistrées. Voilà donc c'est pour sécuriser, j'allais dire ce ce secteur assez. pour pas dire avec, en mettant des guillemets assez dangereux qu'on propose aux cet. Cet enregistrement à partir du 1er octobre 2023.-- Merci à du gouvernement. Le gouvernement entend évidemment les les préoccupations qui sont celles du rapporteur et en réalité les les les partage et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Néanmoins le Gouvernement est défavorable. À cet amendement pour des raisons.-- Un peu philosophique mais aussi pour des raisons techniques. Ceci étant dit cet, cet amendement est une piqûre de rappel bienvenu sur le fait que. Des des des des travaux doivent être poursuivis peut être accélérée. Étant donné l'actualité qui a été celle du marché des crypto-actifs. Je reviens quelques années en arrière, quand en 2018 on s'est posé la question de la manière dont on allait aborder la régulation de ces objets étranges qui étaient les cryptoactifs. La France a fait le choix d'une régulation flexible. Qui consistait à créer un enregistrement facultatif. Qui amène le prestataire en. Service de cryptoactifs à a donné un certain nombre d'informations sur ses clients sur sur son identité et cetera donc ça c'est l'enregistrement. Qui est facultatif, mais qui permet quand on est régi d'avoir pignon sur rue et puis un agrément qui qui qui est, qui est le niveau supplémentaire de régulation. Qui permet de garantir aux clients que là il y a notamment tout un tas de mesures de protection. Des comptes des clients qui aurait peut être évité le le l'épisode qu'on a vu se produire aux États-Unis avec FTX. C'est de. Ces 2 modes. D'enregistrement et d'agrément était facultatif et avait vocation à rendre la France attractive pour ces nouveaux acteurs. Pour 2 raisons. C'est un grand succès français. La première des raisons, c'est que le cadre européen qui a été créée depuis.-- C'est largement inspiré de l'initiative de la France, si bien que le rapporteur la rappeler le règlement Mica qui va entrer en vigueur à l'horizon. 2024 reprend essentiellement les conditions de l'agrément français si bien que les les les entreprises qui commencent à solliciter des enregistrements ou désagréments en France vont pouvoir ainsi facilement accéder. Au niveau. De d'agrément européen, ce qui rend la France extrêmement attractif et c'est le 2ème. Indicateur de succès de cette réforme qu'on avait engagé dans la loi pacte 60 entreprises ont sollicité l'enregistrement et il y a au moins une entreprise qui est en cours d'agrément, même si effectivement l'agrément n'a pas encore été extrêmement largement sollicitée.-- Et donc la raison philosophique pour laquelle. Cet amendement et peut être. Excessivement je dirais. Restrictive, c'est que nous avons un écosystème qui se développe dans notre pays, la France est identifiée en Europe comme le lieu où celles et ceux qui souhaitent avoir pignon sur rue ont tendance à à vouloir s'installer. Et que dans la transition vers Mika peut-être faudra-t-il à un moment donné. Inciter très fortement les entreprises à les solliciter la l'agrément peut être si elle ne s'y mettent pas suffisamment tôt éventuellement les y contraindre. Mais les y contraindre dès le premier octobre 2023 comme vous le proposez. C'est risquer. D'inverser la la perspective qu'ont les investisseurs en France ou à l'étranger et les entrepreneurs en France et à l'étranger de la place de Paris pour le développement des cryptoactifs et de mettre un coup d'arrêt à ce développement. De la finance crypto dans notre pays. l'argument technique c'est que pour avoir un agrément à l'horizon du premier octobre 2023. Il faudrait par exemple que les 60 acteurs qui ont d'ores et déjà obtenu l'enregistrement puissent l'obtenir dans des temps qui nous paraissent peut être intenable.

De la position de la France vis-à-vis de ce marché-là, alors même que et je crois que vous le soulignez un peu dans votre propos. Monsieur le rapporteur. Il y a une forme de continuité entre les choix qui ont été faits par la France en 2018 2019. Les choix européens. qui ont présidé à la rédaction du règlement Mica et que nous avons tout intérêt à nous inscrire dans cette continuité. Autrement dit, peut-être faudra-t-il prendre des mesures d'incitation forte toute coercition mais les prendre dès le premier octobre 2023 nous paraît très excessif.-- Il y a un avis défavorable. Monsieur le rapporteur. Après, c'est donc une demande de retrait. Avec un engagement de pouvoir poursuivre ces échanges sur le le fondement de des réserves exprimées par le rapporteur.-- Merci. Monsieur le rapporteur.

aujourd'hui le, le système d'enregistrement. Il n'est pas facultatif hein c'est uniquement le système d'agrément qui est facultatif. Le système d'enregistrement telle qu'il a été posé par la loi pacte est est obligatoire sur le fond on a déposé cet amendement que bien sûr nous maintenons dont de la commission des finances. Parce que le le superviseur lui-même c'est-à-dire l'AMF s'inquiètent de ce délai extrêmement long de cette période transitoire qui risque de provoquer un appel d'air, c'est-à-dire d'inciter les entreprises à à s'enregistrer au lieu de demander un agrément pour avoir un délai supplémentaire de 18 mois, d'où cet amendement. évidemment on peut dire que le premier octobre. C'est moins bien que le 15 bon la navette éventuellement on pourra se, s'atteler à ce à ce sujet épineux de savoir s'il vaut mieux être le premier octobre ou le 15 octobre ou le 15 novembre, mais nous maintenons cet amendement.-- Bien donc l'amendement est maintenu avec Monsieur le Ministre. L'enregistrement est obligatoire si l'on veut s'enregistrer en France mais nul n'est contraint de s'enregistrer en France pour offrir des services numériques. C'était bien ça. La subtilité de ces régulations dans un espace numérique qui ne connaît pas les frontières terrestres. C'est que si vous réguler de manière trop drastiques. Alors évidemment. Les les sociétés, les entreprises vont s'installer très vite à l'extérieur des frontières nationales, et donc le choix qui avait été retenue c'était venez vous enregistrer en France vous savez un 1er niveau de régulation qui est relativement souple. Vous pouvez de manière facultative solliciter un agrément qui cette fois-ci établira de manière. Certaine que vous avez pignon sur rue et que vous apporter toutes les garanties nécessaires à vos investisseurs. en l'entrée en vigueur de de Mika. Tous les opérateurs voulant opérer en Europe vont devoir passer par un agrément obligatoire. Je dis juste qu'il faut mettre dans la balance la protection des épargnants, comme toujours, mais aussi l'attractivité de la place de Paris.--

Qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté. Je mets aux voix l'article 6 qui est pour.-- Qui est contre.

Oui, merci Monsieur le Président cet. Cet amendement vise à tout simplement supprimer l'article 7. Alors déjà je je je l'ai dit dans mon intervention en discussion générale c'est vraiment j'allais dire une De légiférer par ordonnance dont on aurait pu se passer puisque le gouvernement a disposé. D'un an qui aurait pu être mise à profit pour que ce soit. Transposé dans le dur mais aussi et peut-être surtout, nous avons posé un certain nombre de questions au gouvernement pour avoir des des éclairages sur l'étendue de l'habilitation notamment pour savoir ce qu'il. Entendait mettre dans le Champ de la clause de sauvegarde. Pas de réponse et nous avons également posé la question au gouvernement pour nous assurer que ce ce nouveau dispositif ne créerait pas des contraintes supplémentaires pour les entreprises qui doivent déjà fournir un certain nombre d'informations aux administrations notamment aux administrations fiscales et qui là vont devoir. Les les ce double souci de connaître la clause de sauvegarde et de veiller à ce que ce Champ de de de la directive ne soit pas trop contraignant de son application ne soit pas trop contraignant pour les pour les entreprises et donc comme nous n'avons pas pu obtenir de réponse de la part du gouvernement, je suis contraint de demander la suppression de l'article.--

Fiscal des grandes entreprises pour reprendre les termes de notre rapporteur pour avis Hervé Maurey soit décidé en catimini et ceci par ordonnance. Le sujet est lourd obliger les multinationales dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros de rendre publique une déclaration d'un d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés, pays par pays. La liste d'information et d'une importance cruciale pour les citoyennes et les citoyens, la société civile et les parlementaires que nous sommes le nom de l'entreprise mère et de toutes les filiales, notamment lorsqu'elles sont dans des territoires fiscalement non coopératifs, autrement dit des paradis fiscaux. Une description de leur activité, le nombre de salariés employés. Le chiffre d'affaires. Le montant des bénéfices. Le montant de l'impôt sur les revenus des sociétés du. Le montant de l'impôt acquitté réellement. Quitter et enfin le montant des bénéfices non distribués donnant une idée de l'ampleur des versements de dividendes et des rachats d'actions, tout en permettant de concevoir ce qu'il restera pour chaque exercice financier pour l'investissement, ces informations nous les voulons nous les réclamons depuis des années, sauf que Monsieur le Ministre, nous n'avons pas confiance, nous jugeons indispensable que vous reveniez devant le Parlement pour présenter la transposition finalement nous demandons une transparence complète. Nous ne voulons aucune opacité qui entretient des comportements de contournement de l'impôt en Europe et ailleurs et mine des finances publiques et le consentement à l'impôt. Je vous remercie. S'agissant dans un 1er temps, de la question de la clause de sauvegarde qui effectivement est un élément très important puisque. Le ce ses BCR public comme l'on dit va conduire les exportateurs notamment à publier des informations qui lorsque notamment, ils nous ont que peu de client à l'export pourrait révéler un certain nombre d'éléments. Du relevant presque du secret des affaires, alors concurrent. Ce que je puis vous dire c'est qu'effectivement la directive prévoit une exception permettant de reporter d'au plus 5 ans. La publication de certaines de ces informations lorsque leur divulgation immédiate porterait gravement préjudice à la position commerciale d'une entreprise, c'est le cas dans l'exemple que je venais citer puisque le le CBC. Dans ce cas, s'il était appliqué de manière de manière rigoureuse permettrait de reconstituer les coûts et les marges d'une entreprise et livrerait donc des informations très précieuses et concurrence étrangère. Le gouvernement compte utiliser ce dispositif qui permet de préserver l'exigence de transparence vis-à-vis du public sans fragiliser certaines de nos entreprises stratégiques. sur le 2ème point. C'est-à-dire les les critères les informations qui seront rendues publiques la directive prévoit peu de marge de transposition dans la mesure où les informations qui devront être divulguées par les entreprises ils sont décrites et je les listes. Le nombre d'employés. Le chiffre d'affaires. Le résultat avant impôt, l'impôt sur les sociétés du et acquitté et la part des bénéfices non distribués. Et je me permets d'ajouter à la corbeille. Si vous me permettez. Trois autres arguments le 1er c'est que le seuil d'assujettissement comme vous le connaît comme vous le savez. Est de 750 millions d'euros pour 2 années consécutives. En terme de chiffre d'affaire, sinon vous n'êtes pas assujetti à ces publications. Nous ne ferons pas de ce, de surtransposition, c'est l'engagement que je. Que je prends devant vous et le 3ème élément c'est que nous aligneront autant que possible le texte avec celui transposant le CBC fiscal, c'est-à-dire le le transfert, non pas au public ou la publication à destination du public mais à destination des autorités fiscales pour assurer l'intelligibilité du droit et puis éviter évidemment que les entreprises soient soumises à plusieurs reporting en même temps j'espère avec ces compléments d'information vous a redonné suffisamment de motifs pour retirer les amendements et évidemment cette invitation s'adresse également à Madame la sénatrice.-- Monsieur le ministre a de la chance, je suis bien luné aujourd'hui donc je vais retirer mais franchement monsieur le Ministre, c'est pas des méthodes de travail. Franchement. Quand on interroge des services quand on interroge le cabinet quoi. Alors c'est vrai qu'on a eu des délais très courts, ça je ne vais pas vous dire le contraire mais c'est plus la responsabilité du gouvernement que celle du Sénat qu'on n'a pas de réponse et qu'on est obligé de déposer un amendement pour séance vous nous donniez des informations. Voilà je vais pas jouer le moralisateur. Mais c'est pas c'est pas satisfaisant. Donc vous avez de la chance, je suis de bonne humeur aujourd'hui ça étonne monsieur Marchant mais ça m'arrive parfois. Donc j'ai retiré cet amendement.

Nous on est en train de se questionner pour savoir si on est de bonne ou de mauvaise humeur. Vous voyez, vous, vous êtes de bonne humeur. Moi je le suis un peu moins parce que je trouve quand même qu'avec ce texte on n'a pas eu le temps de discuter. est obligé d'attendre. Cette séance pour pouvoir avoir des informations et on trouve ça quand même dommageable, on pense qu'on aurait pu avoir un peu plus de temps pour discuter en commission et notamment au Sénat de tous ces articles qui sont quand même qui qui ne sont quand même pas rien donc. Je pense que nous allons maintenir l'amendement.-- Donc il y a un amendement qui est maintenu. L'amendement du groupe communiste, je le soumets aux voix qui est pour.-- Qui est contre.-- Qui s'abstient. Qui n'est pas adopté. Et je vais donc soumettre aux voix l'article 7. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. L'article 7 est adopté. Nous passons à l'article 8 avec 4 amendements en discussion commune. Monsieur Didier Marie le premier. Merci monsieur le président. L'article 8 vise à transposer la directive c'est SRD qui renforce significativement les exigences de publication d'informations en matière de durabilité des entreprises. Il convient de faire 2 remarques importantes sur cet article. Cette transposition tout d'abord, c'est quand même particulièrement difficile de travailler sur une directive dont le texte n'a été finalisé par le Conseil européen qu'à la fin du mois de novembre et qui n'est pas encore publié au Journal officiel de l'Union européenne et donc. Difficile pour les parlementaires. De travailler sans ces informations ensuite le recours à une habilitation pour une opération qui va bien au-delà de la simple transposition en droit interne est également particulièrement étonnant. Nous considérons que cette directive et cet enjeu particulier de la transparence des entreprises nécessite un travail approfondi ainsi un texte à part entière. D'autant plus que de nombreuses questions restent en suspens sur cette petite directive sur le contenu des obligations d'information sur le périmètre des entreprises concernées concernées sur l'assurance des informations en matière de durabilité sur le contrôle de l'équivalence des normes non- européenne ou encore en matière de publicité des rapports de gestion, les délais d'entrée en vigueur par ailleurs avec une première strate strate d'entreprises concernées à partir seulement du 1er janvier 2024 nous laisse le temps de retravailler sur ce texte. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement de suppression de cet article et nous demandons au gouvernement de bien vouloir nous déposer un texte en dur pour pouvoir discuter, merci. Merci donc autre amendement de suppression le 28 monsieur. Allez-y-y là.-- Monsieur le président, Monsieur le Ministre, je vais défendre cet amendement de notre collègue Martine Berthet, qui demande la suppression de l'article 8, la transposition de cette directive c'est SRD doit être effectuée par le Parlement et non par voie d'ordonnance car il n'existe aucune raison objective de soustraire la transposition d'une telle directive à la procédure législative ordinaire. La directive c'est cerner multiplie par 5 le nombre des grandes entreprises concernées en Europe mais impactera également dit indirectement ETI et PME située dans leur chaîne de valeur. Elle accroît la quantité d'informations a publié qui devront être certifiés par un tiers indépendant donc coûteux autour du concept de doubles matérialité que l'Union européenne, défend lors de négociations internationales pour définir un standard commun. Il manque une évaluation du coût financier et organisationnel précis par catégorie d'entreprises des informations extra-financière qui seront demandés. Ces éléments auraient pu être obtenues dans le cadre de la procédure législative ordinaire. Ils ne seront pas connus avec une transposition de la directive par ordonnance pour ces raisons on demande la suppression de l'article 8. Merci monsieur Ferrand également à mon de suppression. Oui tout à fait donc mes collègues l'ont déjà bien défendu, je l'avais évoqué dans ma déclaration générale. Cette directive représente une étape importante dans la dans la mise en oeuvre du Pacte Vert européen il y a des questions essentielles sur le périmètre notamment qui demeure. Il y a des choix déterminants qui sont à faire et il y a le temps de les faire, voilà pourquoi nous demandons la suppression.-- Merci. Également un moment de suppression madame pour.-- Oui, s'est défendu Monsieur le Président, nous demandons et. La suppression de l'article aussi merci.-- Il y a un avis de la commission.

Je ferais une demande de retrait pour plusieurs raisons, la, la première c'est que c'est une. Une directive qui offre un peu de marge de manoeuvre en terme de transposition. Et ensuite. Il y a des délais contraints une fois de plus, vous me direz, et qu'il n'y a pas il n'y aurait pas aujourd'hui de véhicule législatif qui se prêteraient réellement à ce que l'on puisse. Faire cette cette transposition J'ajoute que que la version de de l'article 8 telle qu'il a été modifié par la commission. Peut déjà vous donner en partie satisfaction puisqu'on a réduit le le Champ d'habilitation qui était, qui était très large et donc de ce point de vue là au moins il y a, j'allais dire quelque chose qui doit aller dans le, dans le sens des auteurs des différents amendements auxquels je donc je demande donc le retrait.-- Première éléments c'est que c'est évidemment un sujet très important puisqu'on parle de la responsabilité des entreprises et de leur engagement dans la transition écologique est un sujet. Qui est prioritaire pour le gouvernement et pour Bruno Lemaire évidemment au 1er chef. Le 2ème point, c'est que s'agissant de cet article 8, ça a été très bien dit par le rapporteur tous les choix politiques ont déjà été faits, soit par le législateur national soit par le législateur européen est ce qu'il s'agit de faire. C'est tout simplement de mettre les décisions du législateur français et du législateur européen en cohérence pour que nos entreprises puissent à disposer d'un cadre clair et pas trop compliqué et pas trop multi-factorielles pour ce reporting extra-financier qui est qui. Une qui est une vraie révolution en matière de de de comptabilité.-- Alors est-ce qu'on aurait préféré un texte en dur.-- Peut être mais il se trouve que les délais. Que nous avons devant nous. Pour que ces textes entre en vigueur sont très serrés et c'est la raison pour laquelle il vous est plutôt proposé je crois que ce sont des amendements qui arrive juste ensuite. De d'affiner la rédaction des habilitations pour faire en sorte que notamment les craintes. qui ont pu être exprimée en commission sur les seuils sur le type d'entreprise qui pourraient être concernées soient bien indiquées dans les habitations. Mais qu'on puisse aboutir dans les délais à à la publication de ces textes.-- Merci monsieur Marie. Oui. Explications de vote. Merci monsieur le président. Nous allons maintenir bien évidemment. Cet amendement de suppression. Car si c'est un choix essentiel pour le ministre-Lemaire. Ce n'est un aussi pour nous. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Et et nous souhaitons que la représentation nationale puisse avoir. La possibilité de s'exprimer sur le sujet. D'autant que la transposition de cette directive. Viendra en parallèle de la transposition future d'une autre directive qui est en cours de discussion actuellement dans les instances européennes qui est celle sur le devoir de vigilance des entreprises et nous pensons qu'il faut regarder tout cela globalement. Et veillait effectivement à la cohérence des textes mais veiller aussi à ce qu'ils soient efficients, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons pouvoir en discuter ici au Sénat.-- Bien, donc avec un double avis défavorable je vais maintenir enfin les les, on va voter sur les. Amendements maintenu monsieur Babary, celui de Madame Bertrand est maintenu.-- donc les quatre amendements de suppression sont maintenus. Donc je vais les soumettre aux voix qui est pour.-- Qui est contre.

Ensuite. Donc du coup les amendements suivants tombe évidemment puisque l'article a été supprimé. Je mets aux voix l'article 9. Qui est pour l'article 9.--

Passons. L'article 11 avec un amendement de Madame ah pour Olivier le 73 amendements de suppression. Voilà. Peut-on contourner lorsque l'on est une entreprise des décisions prononcées par le juge judiciaire. C'est à cet article le permettra en autorisant les entreprises condamnées pour des infractions pénales gravissime de prouver leur bonne foi et de bénéficier ainsi de l'argent public. Le droit aujourd'hui, prévoit que les, les opérateurs privés peuvent être empêchés de candidater à des passations de marchés publics ou des contrats de concession pendant une durée de 5 ans à compter de la date du jugement définitif, cette exclusion est dite de plein droit. Notons et il faudra modifier la loi en ce sens il est absolument scandaleux que cette condamnation et aucune implication sur les contrats en cours. Je referme la parenthèse pour vous dire que la France faisait figure d'exemple en ayant refusé transposer le mécanisme d'auto-apurement pour pour toutes les infractions prévues à l'article 38. De la directive de 2014 sur les marchés publics. Ce mécanisme est indigne de nos institutions, tant il permet à une entreprise condamnée de pouvoir prouver sa bonne foi. Concrètement, l'opérateur exclus à cause d'une infraction pénale peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent et que ces preuves sont jugées suffisantes. La France au moment de la transposition avait estimé que certaines condamnations mérité de ce droit de repentance des entreprises y compris des multinationales méconnaissance du code du travail non acquittement des impôts taxes contribution aux cotisations sociales ou encore du travail illégal. Voyez déjà les largesses du dispositif pour les entreprises qui fraudent. Et là, il conviendrait de permettre à une entreprise de bénéficier de l'argent des contribuables sans attendre le délai de 5 années lorsque l'entité a été condamné définitivement pour traite d'être humain, je vous remercie.-- Merci. Je comprends parfaitement l'inquiétude de nos collègues du groupe CRCE quant à l'insertion dans le code de la commande publique d'un mécanisme de régularisation pour les opérateurs économiques qui ont été sanctionnés. À des peines entraînant l'exclusion des des procédures de passation de marchés. Je tiens cependant à les rassurer. Car conformément aux de directive européenne de 2014 régissant les marchés publics et les contrats de concession. Nous avons complété en commission le dispositif prévu par le gouvernement, en précisant que les mesures concrètes. Prises par les opérateurs. Pour démontrer leur fiabilité, comme c'est indiqué dans le texte font l'objet d'une évaluation tenant compte de la gravité de l'infraction commise par conséquent le caractère dissuasif des peines d'exclusions. Sont préservés. J'ajoute en outre que sauf à prendre le risque que la France fasse l'objet de recours en manquement les directives européennes, ainsi qu'une récente décision du Conseil d'État ne nous impose ce mécanisme de régularisation et donc je demanderai le retrait de votre amendement, faute de quoi, ce serait un avis défavorable.-- Monsieur le ministre. Cette nouvelle. Même avis. Donc un double avis défavorable. L'amendement est maintenu. Et je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE sur cet amendement numéro 73 avec 2 avis défavorables, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos.-- 26 contre 317, il n'est pas adopté. Je passe à l'amendement 59 présenté par le gouvernement.-- Merci monsieur le président, il s'agit de rétablir la rédaction initiale du projet. Présenté par le gouvernement au Sénat mettant en conformité le code de la commande publique avec les directives européennes de 2014. Et notamment en supprimant un un alinéa. Qui ne précisé que que de manière imparfaite les cas dans lesquels le taux a purement et prescrit.-- Avis défavorable pour les raisons que je viens notamment d'évoquer, il nous paraît effectivement très important que la gravité de l'infraction commise ne soit pas masqué par la mise en place de mesures correctives d'un opérateur économique après sa condamnation et une évaluation prenant en compte ce critère doit donc être prévues par notre droit de façon claire et précise, notamment pour s'assurer que ce mécanisme de régularisation soit équilibré. Donc, avis défavorable.-- Donc, un amendement du gouverneur.-- Monsieur le Ministre, vous voulez ajouter quelque chose.-- Oui simplement pour peut-être préciser mes mes propos. Ce qui compte c'est à la fois le critère de gravité de l'infraction. C'est ça qui a été ajouté par. Par la commission mais la directive européenne prévoit que doivent aussi être prises en compte les circonstances particulières de l'infraction ou de la photo que. Pour si si vous avez si vous étiez amené à à sous-amender votre. Ou je sais pas s'il est encore temps de d'amender le. La, la rédaction de de la commission là ça pourrait satisfaire le gouvernement il s'agit vraiment d'englober les les 2 dimensions que la directive prévoit.-- Monsieur le rapporteur.-- Merci. Désolé monsieur le Ministre mais. La notion de circonstances particulières, est un concept quand même qui est assez peu développé dans le code de la commande publique et cet égard, on ne peut pas le retenir.-- Donc l'amendement. Du gouvernement va être soumis aux voix avec un avis défavorable de la commission. Qui défend le maintien du texte qui l'a adopté en commission qui est pour l'amendement du gouvernement.--

Qui s'abstient. Il est adopté ou passons à l'article 12 avec un amendement présenté par Madame puis ça. Oui, merci Monsieur le Président c'est un amendement que j'ai corédigé avec mon collègue Philippe mouiller, qui a été signé par bon nombre de sénateurs, donc sans vouloir vous forcer la main. Monsieur le Ministre c'est ce sont déjà 2 arguments de poids pour donner un avis favorable à cet à cet amendement. Au-delà de ça. Nous sommes tous conscients que l'adaptabilité des produits et services pour les personnes atteintes de handicap est fondamental. Nous sommes néanmoins conscient qu'elle a un coût et notamment mais pas que pour les terminaux en libre-service notamment pour les distributeurs de billets. Nous sommes aussi conscients parce que nous le vivons au quotidien qu'il y a derrière ces terminaux de paiement et notamment ses distributeurs de billets des enjeux de rentabilité et que jusqu'à preuve du contraire, ni les banques ni les services, quel qu'il soit ne sont des philanthropes. Or nous sommes aussi conscients que la notion de rentabilité ne répond pas toujours à celle de l'aménagement du territoire. De la même façon. Monsieur le Ministre Mesdames et messieurs, chers collègues, nous savons que les personnes qui sont atteintes de handicap sont présentes partout sur notre territoire partout, que ce soit dans les endroits dense que ça soit dans les endroits qui sont les plus reculées, les milieux ruraux en particulier. Et nous savons qu'il n'est pas question, au travers ce type de directives davantage du privilégié des gens qui seraient en secteur. Dans ce type au centre de Paris, au Centre de Grenoble et que du coup des personnes qui seraient sur des milieux où les distributeurs seraient en l'occurrence. Des lieux qui ne serait pas rentable. De ne pas effectivement répondre à leur attente. En l'occurrence de quoi nous souhaitons à travers cet amendement. Monsieur le Ministre de rajouter à cette notion d'adaptabilité une notion de répartition territoriale de sorte que nous soyons pas dans des logiques. Où nous ayons des personnes qui puisse avoir un certain nombre de services qui soit adapté et des personnes là où les services ne sont pas rentables ou les services ne serait pas adaptée.-- Merci cher collègue. Madame.--

Comprend aussi une dimension physique et territoriale et le meilleur exemple, ce sont les distributeurs automatiques de billets. Or, on en a déjà pas tous en milieu rural. De façon générale donc nous constatons en matière de handicap des difficultés territoriales d'accès aux services qui vont au-delà de ceux qui sont évoqués dans la directive. Cette situation est source d'inégalités. Nous devons donc être attentif à réduire ces inégalités d'accès et à ne pas en créer de nouvelles et surtout dans ce texte, hein je pense que l'objectif n'est pas de créer de justement de nouvelle rupture d'égalité surtout pour quand on parle de handicap. Alors l'amendement de nos collègues vient rappeler que la politique d'accessibilité numérique ne sera réelle que si les produits visés sont physiquement accessible sur l'ensemble du territoire. Les obligations prévues par la directive doit se traduire par une mise à niveau des équipements et pas par leur arrêt sur des parties entières du territoire. Surtout quand on parle de, de coups et donc la commission des affaires sociales a émis un avis favorable.-- Monsieur le Ministre.-- Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, sénatrice partage évidemment a l'intention de de l'amendement. Je crois cependant qu'il, il ne faut pas enfin il faut il faut savoir distinguer les les objets de politique publique. Il y a la question de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Et il y a la question de l'accessibilité sur l'ensemble du territoire national en Hexagone et dans l'Outre-mer de l'ensemble des services publics et de certains services privés qui sont visés. Par cette. Direct directive que nous transposons. S'agissant par exemple des bornes de billets de transports, ils sont évidemment attachés au maillage des des gares s'agissant des distributeurs de de billets. Nous avons, ça a été dit par Madame la la rapporteure. L'un des réseaux les plus denses d'Europe avec 74.000 distributeurs de billets sur l'ensemble du, du territoire et évidemment un acteur qui a, qui garantit la la la la la proximité des distributeurs de billets qui est la Poste. J'ajoute à cela que toujours dans cet esprit de vouloir en le plus accessible possible. Les services publics, voire même certains services privés à nos concitoyens dans l'ensemble du territoire. Nous avons déployé des milliers de maisons France service pour que dans chaque canton, on puisse avoir accès. À certains des services. Les les les plus essentielles et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous inviter à à retirer votre amendement pour ne pas que nous nous nous nous mélangeons si l'on peut dire 2 objectifs de politique publique. Ils sont. Et évidemment tous de très important, celui de l'accessibilité pour les personnes en situation d'handicap, celui de l'accessibilité pour l'ensemble de nos concitoyens, quelle que soit leur lieu d'habitation sur le territoire national. Merci Monsieur le Ministre donc. Juste. Allez-y, allez-y pour la commission.-- Ce ministre quelques mots, pour vous dire que je suis extrêmement choqué par vos propos. Je vous invite à relire les conclusions du CNCPH. Je vous invite à relire les conclusions du comité national du handicap, je vous ai dire lire les conclusions des annonces faites pas prendre la République et par la Première ministre

Donc je pense vraiment que c'est un point essentiel et que, au regard de la proposition faite par le, par notre collègue sénatrice il est il faut voter cet amendement parce que nous avons besoin de vérifier que l'accessibilité ne soit pas la contrepartie de la rareté et donc c'est vrai en matière de de distributeurs bancaires ses valeurs en matière de transport. Si on écoute votre argument. Ça veut dire que le risque est extrêmement fort d'opposer l'accessibilité pour les personnes handicapées à l'accessibilité territoriale. Donc voilà donc je voulais simplement vous dire que voilà je suis extrêmement choqué de ces propos-là et au regard de de cet élément, je vous rappelle que c'est une habilitation. Vous avez la main. Vous avez le crayon et donc vous êtes capable amender de définir cette équité territoriale. Voilà donc le maître dans le texte à l'Avantage de clarifier les choses vis-à-vis du monde du handicap qui sud au débat. Par contre vous avez toute la liberté de faire en sorte d'avoir une politique équilibrée sur le territoire donc de cesse regarder alors votre argumentaire parce que je trouve qu'il est extrêmement choquant.-- Monsieur le ministre.-- l'ensemble des services qu'ils soient privés et publics, et par ailleurs, j'invite toutes celles et ceux qui se réjouissent avec nous de la transposition de cette directive à réfléchir aux raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas fait lorsqu'ils étaient en responsabilité. bon. Simplement l'accessibilité territoriale. C'est un principe de fait et c'est un principe pour nos concitoyens qui sont en situation de handicap et pour nos concitoyens qui ne le sont pas, il ne faut pas mélanger les dessus.-- allons nous allons procéder oui madame puis ça. Non mais simplement, Monsieur le Président pour dire que je je maintiens mon amendement bien entendu. Parce que, très honnêtement je je pense que notre réalité alors je je ne pouvais pas de je vous fais pas de de de de de reproche. Monsieur le Ministre mais mais par contre on on est vraiment à se battre en milieu rural pour défendre nos nos distributeurs de billets si on prends que cet exemple là et on le sait très bien, on a beaucoup de personnes âgées, beaucoup de personnes qui sont en fauteuils beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap qui ne peuvent plus retirer de l'argent dans nos campagnes, donc à un moment donné et c'est de notre responsabilité de notre responsabilité en tant que parlementaire, de dire que la notion d'aide ménagement du territoire, elle doit être inhérente à cette directive et je crois qu'il faut maintenir Bien donc je soumets je suis mal amendement voit avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Il est adopté. Je soumets aux voix l'article 12. Ainsi amendée qui est pour. Qui est contre.-- Qui s'abstient il est adopté. Je suis je mets aux voix l'article 13 qui est pour.-- Qui est contre.-- Qui s'abstient. Est adopté après l'article 13, un amendement 78 défendue par Monsieur Marchand. Merci Monsieur le Président, effectivement je défends cet amendement. On Madame avait l'article 48 de la loi Dadu de 2021 entendait soutenir le développement du financement participatif obligataire des collectivités territoriales et de leurs établissements à compter de 2022 sous forme expérimentale l'obligataire en financement participatif se présente comme un instrument simple et sécurisée et peut permettre aux collectivités de diversifier leurs sources de financement. En outre, lorsqu'il s'inscrit dans une démarche participative. Le financement est employé par les collectivités pour fédérer engagé les citoyens entreprises autour d'enjeux du territoire ou de transition. Cependant l'expérimentation n'a pas pu débuter faute de publication de l'arrêté qui avait été prévu le présent amendement propose de rétablir le dispositif qui avait été adoptée par le Sénat l'année dernière afin de le rendre applicable le 2ème entend permettre aux opérateurs de financement participatif de financer les investissements des collectivités donc compris dans le Champ du règlement européen sur les prestataires européens de services de financement participatif, à savoir les activités non commerciales, cette mesure a été défendue sur plusieurs de nos bancs. Je vous remercie.-- Merci, monsieur le Président, je connais bien le dispositif, évoqué par Monsieur Marchand puisque c'est nous qui sommes à l'origine de ce dispositif dans le cadre du précédent Dadu. je ne sais pas s'il faut revenir à la version que nous avions voté ici sachant qu'il y a eu une version de consensus qui a été adoptée à l'issue d'une CMP positive avec avec l'Assemblée nationale, en revanche ce qui est certain, je suis très heureux que ce soit rappelé depuis ces bancs. L'arrêter que devait prendre le ministre des finances monsieur Bruno Lemaire n'a jamais été pris et ça n'est pas faute de lui avoir adressé plusieurs courriers restés sans réponse. Donc sur ce sur ce sujet également sur le statut des prestataires de services de financement Il y a un sujet parce que ce statut ne relèverait pas du règlement européen. Donc sur ces 2 points. La publication de de l'arrêter et sur le statut des prestataires de financement participatif. Hé bien je me tourne vers le gouvernement pour savoir où en est l'arrêter et et où en est la question que j'ai posée sur le statut des finances des. Prestataires de services de financement participatif. Pas car comme les auteurs de l'amendement. Je souhaiterais évidemment que le dispositif voté par le Parlement entre enfin en application.-- Monsieur le ministre.-- et ce qui nous permettra d'évaluer l'efficacité de ce dispositif de la finesse si besoin et c'est la raison pour laquelle je vous propose de retirer votre amendement monsieur c'est. Monsieur Marchand étant moi aussi victime du syndrome Moret donc je retire cet amendement.-- Bien. L'amendement est retiré donc je mets aux voix maintenant. L'article 14 qui est pour.-- Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté un amendement dans l'article 15, le 67, madame pour.-- Merci monsieur le président. L'article 15 du projet de loi transpose la directive du 20 juin 2019 relatives aux conditions de travail transparentes et prévisibles. La durée maximale de la période d'essai est fixé actuellement selon la catégorie professionnelle du salarié de mois pour les ouvriers, employés, 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise et 4 mois pour les cadres. Cette période peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit l'article 8 de la directive européenne fixe une durée maximale de six mois, le gouvernement prévoit donc de supprimer la possibilité qu'un accord de branche étant de la période des CO2 la de six mois. Mais alors que le texte prévoit explicitement une dérogation pour l'exercice d'une fonction managériale de direction d'un poste dans le service public, le gouvernement sous transpose la directive en maintenant une dérogation pour les cadres, avec une période d'essai maintenu à huit mois, cette sous-transposition n'est pas sans conséquences pour les quatre et demi million de cadres du secteur privé qui devront se soumettre à une période d'essai d'huit mois alors même que la majorité d'entre eux n'occupe ni une fonction managériale ni un poste de direction. Le gouvernement a clairement adopté une définition des exceptions qui dépasse le cadre fixé par la directive lorsqu'il s'agit de mettre en place des protections collectives. Le gouvernement n'hésite pas sous transposer les directives et lorsqu'il s'agit de favoriser les entreprises où le marché le même n'hésite pas sur transposer les directives bref 2 poids 2 mesures, comme toujours. Comme souvent avec vous. Ce monsieur le Ministre, pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article, je vous remercie.-- Oui, merci Monsieur le le président. Alors la commission et approuvé la l'article 15. Qui assure la mise en conformité nécessaire et suffisante du droit du travail au droit européen. le maintien dans le droit du travail de durée périodes d'essayer de 8 mois pour les cadres et permis par le droit de l'Union européenne. Je rappelle que le droit du travail l'autorise à condition qu'un accord de branche étendu le prévoie il nous a semblé utile de laisser aux partenaires sociaux le soin de fixer ses durer selon les secteurs d'activité sans dépassé le délai de de huit mois renouvellement compris. Et d'autre part, si on supprime cette Sertic hein ça empêchera d'assurer la conformité du droit du travail au droit européen notamment pour l'information du salarié sur les éléments relatifs à la relation de de travail ou encore et ça c'est assez important pour l'information des salariés en CDD ou en contrat d'être d'intérim sur les postes qui sont ouverts en CDI, dans l'entreprise dans laquelle il travaille. Alors pour toutes ces raisons, nous avons émis un avis défavorable.-- Merci madame la ministre. Même avis que la commission. Même avis que la commission et un peu surprise de la suppression de cet article présenté par ce groupe, qui défend les les les cadres peut-être. Pas de second que je n'aurais imaginé qu'un qu'un qu'un amendement puisse de suppression Bien donc je soumets aux voix l'amendement de suppression de Madame pour polique avec d'où un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté, je mets aux voix l'article 15 qui est pour.-- Qui est contre qui s'abstient-il être adopté article 16 même votre. Article 17 même vote. Sur l'article 18, un amendement rédactionnel monsieur Marie.-- Oui c'est un amendement logistique rédactionnelle. Pas de souci.-- Avis de la commission sur cet amendement.

L'article 20 a été précédemment examiner. Je mets aux voix l'article 21 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. L'article 22 même votre. votre. Vote. Les articles 23 et 24 ont été précédemment examiner je mets aux voix l'article 25 qui est pour. Qui est contre. Il s'abstient il est adopté. Je vais suspendre la séance elle sera reprise. À 17h 30 dans, dans quelques minutes pour la déclaration du gouvernement en application de l'article 50 tirer 1 de la Constitution relatives à la politique de l'immigration. La séance est suspendue.--

L'ordre du jour appelle une déclaration du gouvernement suivie d'un débat. En application de l'article 50 tirer 1 de notre Constitution. Relatives à la politique de l'immigration.-- Je vais immédiatement donner la parole à Madame. Élisabeth Borne Première ministre.-- Et messieurs les sénateurs. L'immigration est un sujet complexe. Il nous conduit à parler de politique publique. Mais aussi de notre histoire et de notre conception de la nation. Il est parfois l'objet de passion, de tension, voire de fractures.-- Et pourtant, il est essentiel de pouvoir en débattre sereinement.-- Je sais en introduisant ce débat au Sénat que nous partons sur des fondements solides.-- La haute assemblée a toujours eu à coeur de porter des débats d'idées et de chercher des solutions communes.-- Vous avez aussi je le sais et j'y reviendrai travailler sur la question migratoire sur ses implications et sur les grands chantiers à mener.-- Parler d'immigration c'est aborder bon nombre de sujets. C'est évoquer les causes profondes des migrations. La pauvreté, le dérèglement climatique et notre indispensable coopération avec les pays d'origine et de transit.-- C'est parler de nos frontières hein de nos procédures et de notre droit.-- C'est relever le défi de l'intégration.-- Dans quelques semaines, le gouvernement présentera un texte sur notre politique migratoire. Les ministres reviendrons dans un instant sur ses principes directeurs.-- Comme je l'avais annoncé ce projet de loi fait l'objet d'une vaste concertation. Le ministre de l'Intérieur a conduit avec l'appui de la secrétaire d'État à la citoyenneté. Le ministre du Travail. S'il est également pleinement engagée.-- Le texte doit consolider les avancées de la loi asile immigration et adapter notre droit aux défis actuels de la question migratoire.-- Je l'ai dit à l'Assemblée nationale et je le répète devant vous. Nous n'avons qu'une boussole, l'efficacité nous porterons un texte équilibré aux effets utiles et concrets.-- Il me semblait donc important essentiel même avant la finalisation du projet de loi et comme je m'y étais engagé de venir devant vous pour vous présenter des faits des orientations et pour en débattre.-- Alors Mesdames et messieurs les sénateurs. Commençons par les faits.-- D'abord oui il existe une immigration légale. Je le dis car à entendre certains, on l'oublierait.-- Cette immigration légale, ce sont des salariés qualifiés ou encore les personnes que les Françaises et les Français ont choisi d'épouser.-- J'entends souvent dire que le nombre de titres délivrés a progressé. C'est juste la tendance ne date pas d'hier et elle s'est vérifiée sous des majorités de gauche comme de droite.-- Ainsi en 15 ans le nombre de titres de séjour délivrés est passé de façon progressive, de 172.000 en 2007 à 271.000 en 2021.-- Mais ne nous trompons pas sur les causes de cette augmentation.-- Contrairement aux caricatures, l'immigration familiale a baissé sur cette période. S'il y a eu une augmentation, c'est pour 3 raisons.-- D'abord parce que notre enseignement supérieur est attractif et que depuis 2017 le nombre d'étudiants que nous accueillons a doublé. C'est une bonne nouvelle. Ces étudiants apprennent à parler français à connaître notre pays et le font rayonner dans le monde. 2ème raison de Sète hausse le nombre de salariés qualifiés et de chercheurs que nous à qui que nous accueillons a augmenté en 15 ans. Et cela a bénéficié à notre économie, à nos entreprises à notre innovation. Enfin, dernière raison de la hausse l'augmentation modérée du nombre de bénéficiaires de l'asile. Ce sont 30.000 personnes menacées dans leur pays que nous accueillons chaque année.-- C'est le nord de la France, de leur donner leur place c'est l'honneur de notre pays d'avoir accueilli 3000 ressortissants afghans juste après la chute de Kaboul l'an dernier, c'est le nord de la France d'avoir accueilli 108.000 Ukrainiens depuis le 24 février dernier sous le statut de la protection temporaire. Au nom du gouvernement, je tiens à remercier l'Ofpra. Les élus locaux, les associations et les uns et les employeurs qui les accompagnent au quotidien.-- Bien sûr nous devons donner à toutes les personnes arrivées légalement les moyens d'une intégration dignes et complète.-- Certaines difficultés existent encore, notamment en terme d'insertion professionnelle. J'y reviendrai. Voilà, Mesdames, et messieurs les sénateurs. Quels sont les faits concernant l'immigration légale. Mais le principal enjeu, ça n'est pas tant la situation de ceux à qui nous avons délivré un titre que celles des personnes qui se maintiennent sur notre territoire sans y avoir droit. Ces personnes ne sont pas éligibles à l'asile. Il aura souvent été explicitement refusé.-- Pourtant le flux de demandes augmentent nettement ces dernières années et celles et ceux à qui nous n'accordons pas la protection reste encore trop fréquemment sur notre territoire. Souvent victimes de passeurs qui leur promettent l'eldorado et mettent en danger leur vie. La plupart d'entre eux vivent dans la grande précarité sans disposer du droit à travailler et parfois sombrent dans la délinquance.-- Face à ce défi, les amateurs de solutions toutes faites sont nombreux, on trouve les partisans du yakafokon qui voudraient renvoyer d'un coup d'un seul l'intégralité d'entre eux. Alors oui, je souhaite que le droit et nos frontières soient respectés. Oui, je souhaite des éloignements rapide et efficace des personnes en situation irrégulière. Mais non, on ne peut pas prétendre que les choses soient si simples comme si nous pouvions nous affranchir de l'indispensable coopération des pays d'origine et des règles de l'état de droit. De l'autre côté. Certains appellent à des opérations de régularisation massive, je le dis aussi clairement, il n'en est pas question. Nous ne créerons pas de tels précédents qui ne réglerait pas les difficultés des personnes concernées qui donnerait des arguments aux passeurs et qui ne serait ni accepté ni acceptable par les Français. Pour notre part, nous voulons prendre le sujet à bras le corps et proposer des solutions, utile et efficace. Je crois que nous pouvons nous retrouver sur une préoccupation commune. Éviter que des étrangers restent durablement dans une situation indéterminée qui ne serait ni le droit au séjour ni l'éloignement aussi nous voulons clarifier beaucoup plus vite la situation des étrangers arrivés sur notre sol. D'une part nous voulons accélérer les procédures d'examen des demandes d'asile et du droit au séjour pour lutter contre les pratiques dilatoires et d'autre part une fois la situation clarifiée. Nous souhaitons éloignée plus rapidement ceux qui doivent l'être. Quant aux personnes qui ont vocation à rester. Nous voulons engager plutôt les actions pour réussir leur intégration, d'abord par la langue et l'emploi. Ces principes sont les grands axes de travail du gouvernement. Ce sont des objectifs qui, je le crois peuvent rassembler largement en particulier au sénat.-- Car je sais pouvoir trouver sur ces bancs des partenaires pour pour pour construire ce texte ensemble. Les constats que vous avez formulées dans votre rapport d'information et qui faisait l'objet d'un large consensus parmi les groupes au Sénat. Monsieur le Président buffet, nous les partageons.-- Le projet de loi que présentera le gouvernement reprendra ou s'inspirera de bon nombre de vos propositions pour celles qui relèvent du domaine législatif. Nous en mettrons d'autres en oeuvre je pense à celles qui concernent l'indispensable amélioration de l'accueil en préfecture et les modalités de recueil et de traitement des demandes de titre de séjour. J'y reviendrai et le ministre de l'Intérieur également.-- Je retiens cette volonté de travail commun, cette volonté de bâtir des solutions au delà des clivages et des postures et c'est pourquoi, comme pour la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Je vous confirme que nous examinerons le futur projet de loi d'abord au Sénat. Je souhaite ainsi que nous puissions bâtir une majorité solide sur ce texte. En nous appuyant notamment sur l'important travail déjà réalisé par les sénateurs sur ces sujets migratoires. Mesdames, et messieurs les sénateurs, comme l'a dit le président de la République. Nous devons déployer une action complète cohérente et efficace en amont des flux migratoires et après l'arrivée sur notre territoire. Nous voulons d'abord prévenir les départs irréguliers en contribuant grâce à notre aide publique au développement, à traiter les causes profondes des migrations que sont la pauvreté et de plus en plus les effets du dérèglement climatique. Ensuite, nous devons mieux protéger nos frontières pour y parvenir notre 1er levier d'action est européen. Pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne, nous sommes parvenus à plusieurs avancées autour du pacte sur la migration et l'asile en particulier pour rendre plus efficaces les contrôles à l'arrivée en Europe et pour renforcer le mécanisme de solidarité pour les états de première entrée dans le respect du droit maritime. Nous devons maintenant continuer nous poussons pour un renforcement des moyens de Frontex et pour une réforme de l'espace Schengen. Nous voulons également consolider le système d'asile européen et c'est aussi à l'échelle européenne que nous lutterons plus efficacement contre les réseaux de passeurs. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna et la secrétaire d'État en charge de l'Europe. Laurence Boone sont pleinement mobilisés en ce sens.-- Le 2ème moyen d'action, c'est au niveau national en renforçant le contrôle à nos frontières et en accélérant les procédures en novembre 2020, le président de la République a annoncé le doublement des effectifs à nos frontières. Les résultats sont là, 10.000 refus par mois ont été prononcées en 2021 contre 3000 début 2020 avant le Covid.-- Ensuite nous devons accélérer les procédures d'examen des demandes d'asile dans ce domaine, des progrès ont été réalisés dans le précédent quinquennat, les délais de l'Ofpra ont considérablement diminué mais ceux des procédures contentieux sont encore trop long. Au total, le délai moyen de traitement d'une demande d'asile est encore de l'ordre d'un an. Nous devons donc accélérer et visé un Dédé global de 6 mois pour l'ensemble de la procédure. Nous voulons notamment réformer le contentieux des étrangers. Pour le réduire et le simplifier. Nous voulons passer de 12 procédures contentieuses A4 suivant en cela les recommandations du Conseil d'État et du rapport d'information du président buffet. Le ministre de l'Intérieur. Il reviendra et travaille également avec le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti à une réforme de la Cour nationale du droit d'asile. Enfin, nous voulons éloigner plus systématiquement et plus efficacement les personnes déboutées du droit d'asile. Nous devons augmenter nos capacités en centre de rétention administrative et nous continuerons à agir dans nos relations bilatérales avec les pays qui refuse de réadmettre leurs propres ressortissants.-- Par ailleurs, nous devons être intraitable avec les étrangers délinquants, même en situation régulière. S'engager dans la délinquance c'est se placer en dehors de notre communauté nationale c'est porter une atteinte grave à notre pacte social et à nos compatriotes c'est également nuire à tous les étrangers qui vivent en France et qui construisent paisiblement des parcours d'intégration réussi dont on ne parle pas. Grâce à l'action déterminée du ministre de l'Intérieur et des préfets. Plus de 3000 lettres étranger, auteur de troubles à l'ordre public ont été éloignés en 2021 et 2022. Enfin, sous le contrôle du juge et dans le respect de nos engagements conventionnels. Des mesures d'expulsion doivent désormais pouvoir être prises contre les étrangers, quelle que soit leur situation qui commettent des infractions graves. Mesdames, et messieurs les sénateurs, je le disais, nous portons une vision équilibrée. Si nous voulons que ceux qui ne doivent pas rester partent hein c'est aussi pour pouvoir mieux intégrer ce que nous accueillons. Cela passe d'abord par une refonte en profondeur de l'accueil en préfecture pour les les démarches de renouvellement des titres des étrangers en situation régulière. Nous devons éviter les pertes de droits notamment d'emplois que peuvent connaître certaines personnes faute d'accès au guichet pour les demandeurs d'asile. Nous devons aussi continuer à renforcer nos capacités d'hébergement en 5 ans, nous les avons déjà augmenté de plus de de 36.000 places. Enfin le pivot de notre politique d'intégration. C'est le travail. Dans un pays dont le taux de chômage est de 7,3%. Nous devons d'abord cherché à pourvoir les postes à pourvoir les postes vacants en proposant ses employes à nos ressortissants et en aux personnes en situation régulière. Le taux d'emploi des immigrés en France et 9 plus faible que celui de l'ensemble de la population, nous devons travailler à réduire cet écart. Ensuite, si les employeurs ne sont pas parvenus à trouver la main-d'oeuvre dont ils ont besoin, ils peuvent la faire venir de manière légale. Un employeur peut toujours solliciter une autorisation de travail s'il démontre qu'il n'a pas pu pourvoir le poste en déposant une offre auprès de Pôle Emploi pour certains métiers, particulièrement en tension l'employeur et même dispensés de cette justification. Nous avons simplifié ces dispositifs en 2019 pour mieux répondre aux besoins. Enfin, la question de la régularisation peut se poser pour des personnes en situation irrégulière présentes sur notre sol depuis des années et qui travaille depuis longtemps.-- Ce sujet mérite mieux que des caricatures. Il ne s'agit en aucun cas d'une régularisation massive, ni des ni de laisser penser que la régularisation serait la réponse aux tensions sur le marché du travail. Il s'agit de régulariser certaines personnes qui contribuent depuis longtemps à la richesse nationale n'qu'ils subissent parfois des conditions de travail indignes et reste enfermé dans un statut précaire. Le ministre du Travail Olivier Dussopt. Il reviendra plus en détail. Enfin, mesdames et messieurs les sénateurs s'intégrer c'est parler la langue de la République alors que nous proposons des cours de langues dès l'arrivée sur le territoire. Nous souhaitons qu'un niveau minimal de français soient désormais. Pour obtenir des prix des titres de séjour de plus d'un an.-- Mesdames, et messieurs les sénateurs. J'ai tracé devant vous les grands principes de notre action, une action fondée sur la volonté d'équilibre et la recherche d'efficacité d'abord agir sur les causes profondes de l'immigration en lien avec les pays d'origine et de transit. Assurer ensuite le respect de nos frontières et de notre droit par des procédures plus rapides et des mesures d'éloignement mieux appliquer et donner enfin à celles et ceux que nous accueillons les moyens d'intégration pleine entière et réussie car l'intégration c'est bien la finalité de toute politique migratoire autour de ces principes, je suis et je reste convaincu que nous pouvons construire des réponses ensemble. Je sais que le Sénat fidèle à sa volonté de dialogue et d'action. Il prendra avec nous toute sa part. Je vois bien.-- Je vais donner la parole.-- Gérald Darmanin, ministre de l'intérieur des Outre-mer. Monsieur le ministre.---- Madame, la Première ministre. Messieurs les Ministres mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président. C'est un honneur après madame, la Première ministre de pouvoir. Dire quelques mots sur ce débat qui porte sur la politique migratoire de notre pays au moment où comme l'a annoncé madame, la Première ministre un texte sera déposé en premier devant la Haute Assemblée, un texte que je porterai avec. Le ministre du Travail en lien parfait avec Monsieur le le garde des Sceaux et qui prévoit finalement 4 sujets ou 4 thèmes que je voudrais détaillé après la Première ministre de premier, celui de la fermeté le deuxième celui de la simplification. Le 3ème, celui de l'intégration et le quatrième celui du travail je laisserai évidemment ce 4ème thème. Évoqués par le ministre du Travail lui-même. Celui de la fermeté parce que comme l'a dit le président de la République dans sa campagne électorale comme. La haute assemblée là déjà réclamé comme la Premier ministre vient de le signifier, nous avons aujourd'hui, trop de difficultés à expulser des personnes qui sont sur notre sol que nous ne voulons plus et qui commettent des actes délictuels graves ou des actes criminels ou des personnes qui sont fichées par nos services de renseignement, non pas par la jurisprudence des tribunaux. Non pas par les engagements constitutionnels ou conventionnels, autres pays mais par les propres règles que nous nous sommes mis nous-mêmes dans les années 2000 à l'occasion sans doute d'un temps qui n'était plus tout à fait celui que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit de mettre dans le texte de la République la fin. Des réserves d'ordre public, c'est-à-dire la fin de la fin de la double peine qui empêche le ministre de l'Intérieur et les préfets d'expulser du territoire national. Toute personne qui a commis des actes graves condamné ça sont définitives. Pas les tribunaux à plus de 5 ans de prison et qui relève souvent des crimes des personnes qui s'en prennent. Aux femmes, aux enfants, les personnes dépositaires de l'autorité publique ou par exemple les trafics de stupéfiants. Aujourd'hui il y a cette réserve d'ordre public, nous proposons de regarder qu'une qui essaie de l'engagement international que nous avons porté notamment vis-à-vis des mineurs, il s'agit en effet des mineurs qui commettent des actes délictuels ou criminels lorsqu'ils sont mineurs, parce que là, il appartient évidemment à l'autorité judiciaire de suivre directement ces personnes mais nous proposons de lever les autres restrictions à l'expulsion de nos concitoyens étrangers qui commettent ces actes délictuels ou criminels graves et de pouvoir mettre ainsi dans la Loire, l'impossibilité qu'préfet de présenter à l'expulsion ces personnes en respectant l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme qui prévoit. Une sorte d'équilibre entre la vie privée et familiale et le droit au séjour entre la Sûreté nationale, la sécurité publique et la vie privée et familiale. Mais ce que nous disons nous, c'est que ce n'est pas à la loi de s'autocensurer pour empêcher ces discussions, 4000 par an, pourraient être prononcées exécutées et comme l'a rappelé madame, la Première ministre nous en sont à 3100 depuis 2 ans. Mais c'est bien au juge de confirmer ou non. Cet équilibre entre la vie privée et familiale et les impératifs de la sécurité nationale. Ce que nous proposerons au Parlement, c'est de supprimer, donc, ces réserves d'ordre public et de copier/coller. L'article 8 de la Convention européenne. De sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Le 2ème, sujet sur lequel je voudrais ici évoquer c'est celui de l'augmentation des places de rétention administrative dans le cas de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, le gouvernement a accepté un amendement du député Éric Ciotti d'augmentation jusqu'à 3000 places de centre de rétention administratif ce centre de rétention ministre sont nécessaires pour pouvoir mieux expulser un certain nombre de nos. Concitoyens étrangers qui commettent des actes de délinquance ou qui sont fichés pour des services de radicalisation. Nous connaissons aujourd'hui une spécificité désormais dans les Centres de rétention illustratif puisque nous y mettons désormais à 92% c'est le chiffre de ce matin, des personnes qui ont un casier judiciaire ou qui sont suivis par les. Services de renseignement. Nous n'y mettons plus les étrangers en situation irrégulière qui sont sous le coup certes d'une OQTF mais qui ne présentent pas de danger pour nos concitoyens. D'autres formules sont apprends c'est-à-dire l'assignation à résidence par exemple depuis que je suis ministre de l'Intérieur. J'ai aussi demandé que progressivement et c'est désormais plus le cas aujourd'hui, à l'exception du territoire de Mayotte, territoire bien spécifiques s'il en est, nous pourrons reparler dans le débat bien évidemment d'enfants dans ce centre de rétention administratif. Et à la demande de madame, la Première ministre et du président de la République, nous mettrons dans le texte que nous vous présenterons l'interdiction de mettre des mineurs dans des centres de rétention administratif. Dans les prochaines années, une fois que ce texte sera voté l'assignation à résidence. Sera évidemment la règle la spécificité du centre de rétention administratif et notamment son aspect carcéral mais aussi les publics que nous y mettons désormais c'est-à-dire des publics qui sont dangereux pour nos concitoyens méritent. Évidemment que nous puissions aller vers ce genre de propositions à la fois d'une augmentation considérable de place de gras, nous en avons ne serait-ce que l'année 2022, augmenté de 450 le nombre de places de crèches éligible et malgré les contraintes du Covid mais évidemment correspondre à l'augmentation voulue par le Parlement et peut-être dans quelques jours, promulguée par le président de la République dans la Lopmi tout en y mettant pas des mineurs qui n'ont pas à connaître ce type. De rétention. Le 2ème sujet après la fermeté et je passerais évidemment sur d'autres dispositifs qui seront contenues dans la loi, il s'agit des un grand acte de simplification nos aspirants comme l'a dit mais un Premier ministre directement du rapport du sénateur buffet qui prévoit en effet de simplifier, de 12, A4, le nombre de procédures possibles pour nos. Concitoyens qui viendraient contester. Évidemment des actes administratifs pris par les préfets de la République. La longueur. De l'attente et des recours suspensif empêche d'avoir une politique d'immigration digne de ce nom, digne de ce nom pour notre pays qui n'arrive pas à faire exécuter correctement les lois de la République et lorsque les tribunaux au bout d'un an d'un an et demi deux ans lui donne raison. Les personnes sont souvent plus expulsables parce que notamment, ils ont fait leur vie privée et familiale. Ce sont deux République et notamment eu par exemple des enfants et qui rendent inexpulsable. De notre sol et en même temps à ce que nous disons oui, notamment dans le cadre de la demande d'asile. Un an et demi, deux ans c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long pour pouvoir s'intégrer et pour pouvoir travailler pour pouvoir vivre dans le pays qui les accueillent. Parmi les simplifications. Il y a une simplification effectivement de la CNDA le garde des Sceaux, sans doute reviendra en partie sur cette question il. S'agit pour nous de la territorialisée pas garder une seule CNDA mais de faire des CNDA, il s'agit pour nous de permettre le juge unique. Alors, nous entendons la demande du Conseil d'État et de la CNDA de garder une instance collégiale pour des arrêts de principe. Je crois que le texte de présenteront correspondra à la demande du Conseil d'État, mais que l'immense majorité des décisions puissent se prendre en juge unique afin de pouvoir être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide, il s'agit de mettre en place. Visio-conférence par exemple et il s'agit évidemment de pouvoir simplifier le lien entre le refus, ce qui est le cas à 70% de la demande d'asile et l'OQTF puisque les dispositions que nous vous présenterons. Il s'agira de correspondent à la à la au souhait de la campagne du président de la République, le refus d'asile à l'Ofpra ou à la CNDA en cas d'appel vaudra OQTF et le tribunal administratif aura 15 jours pour pouvoir juger. L'acte ainsi contesté aujourd'hui une demande d'asile, c'est entre un an et un an et demi, voire 2 ans pour avoir une réponse. La loi que l'on a permis de passer le travail de l'Ofpra de 9 mois 5 mois mais la CNDA malheureusement pour les raisons que nous avons évoqués prend. Un peu trop de temps, en tout cas par manque de moyens et par manque de simplification. L'idée c'est qu'au mois de 9 mois. La demande d'asile complète de n'importe quel demandeur d'asile puissent être jugés. D'autres accès de simplification évidemment lieu je ne vais pas détailler ici ils reprennent largement le le rapport. Du président du c'est fait je crois à l'unanimité de votre assemblée, le 3ème. Sujet, ce qu'elle, je voudrais m'appesantir encore les pour les deux minutes qui me restent, c'est celui de l'intégration. Vous avez voté dans la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, une augmentation de 25% du budget intégration plus de 100 millions d'euros et notamment de l'apprentissage du français comme l'a dit madame, la Première ministre, 25 pour des étrangers réguliers sur notre sol parle très mal le français, donc, ont beaucoup de mal à s'intégrer. Certes il y a des cours de français obligatoires mais ils ne sont pas sanctionnés par un examen qui conditionnerait le titre de séjour et ce que nous proposons c'est que les titres de séjour soit conditionnée à la réussite et non pas simplement au passage de l'examen de français et ah. Conformément à ce que nous avons évoqués dans la loi dit des principes de la République. À l'adhésion des valeurs de la République et s'il n'y a pas la réussite de cet examen de français c'est quand même pour 270.000 personnes par an que cela serait organisée. Et s'il n'y a pas de réussite à l'examen sur les valeurs de la République, il ne peut pas y avoir 2 types de séjours comme les mêmes, l'immigration serait une immigration familiale. C'est évidemment très important. Le ministre du Travail reviendra également sur l'apprentissage du français dans le cadre du travail et des obligations que nous pourrons imposer sa demande ce quelque chose qui n'est pas législatif mais ça demande quelque chose qui relève évidemment du travail réglementaire du travail d'organisation de ministère de l'Intérieur, une révolution dans l'organisation des préfectures qui doivent arrêter de demander la vérification de titre de séjour, de gens qui sont depuis de nombreuses années sur le sol national qui travaillent et qui n'ont au 15 du casier judiciaire. Il faut que ces titres-là soit automatique avec un devoir de rappel de la part des fonctionnaires en cas difficultés ou en cas de casier judiciaire, évidemment de ces personnes. Mais sa demande de concentrer l'intégralité des agents de préfecture du travail des préfectures. D'une part sur les primo-arrivants. vérifié que ces personnes. Parlent bien le français veulent s'intégrer au accès un métier puisse faire vivre leurs familles dans des conditions acceptables, d'intégration et également d'expulsion puisque évidemment il faut améliorer très largement. Les exécutions de quitter le territoire national et comme je l'ai dit, le retrait de titre de séjour aussi de toute personne qui a un casier judiciaire j'en terminerai par là, mesdames et messieurs les sénateurs. Depuis 2001 et depuis la circulaire que j'ai pris à la demande du président de la République, 92.000 titres de séjour ont été refusés ou retirés pour des étrangers qui avait une difficulté avec les règles de la République, on va dire ça comme ça évidemment désormais l'étape supplémentaire, c'est de pouvoir s'assurer qu'ils aient quitté le territoire national. Pour cela il faut que les moyens de la préfecture. Arrête d'embêter. Administrativement, ce qui ne pose aucun problème à la République et se concentre plus largement sur ce qui pose des près de la République. Je crois que c'est ce que demandent les Français. Merci monsieur le ministre de l'Intérieur. La parole. Monsieur Éric Dupond-Moretti Garde des Sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président. Madame, la Première ministre, messieurs les ministres, Monsieur le président de la commission des lois, mesdames et messieurs les sénateurs. Comme l'a souhaité madame la Première ministre. Le Sénat est aujourd'hui.-- Réunis pour débattre d'un sujet important. Un sujet extrêmement complexe. Qui peut se résumer au fond d'une question simple, comment et sous quelles conditions accueillir sur notre sol. Des femmes et des hommes de nationalité étrangère. L'immigration à, à l'évidence est un phénomène qu'il faut voir de façon globale.-- Et pragmatique. Global et la question de l'immigration, implique, vous le savez de nombreux périmètre ministériel.-- Comme en témoigne d'ailleurs la présence de plusieurs de mes collègues. Pragmatique car pour trouver des solutions, il faut se départir de tout dogmatisme de toute démagogie et bien sûr de tout angélisme. Ont depuis longtemps. Le ministère de la justice travaille et tous les autres ministères impliqués sur la question de l'immigration et plus particulièrement sur les procédures administratives et pénales applicables aux étrangers de quoi parlons-nous exactement. Il faut tout d'abord réfléchir à la simplification. Du traitement du contentieux des étrangers.-- Ce contentieux constitue l'activité principale des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Comme le souligne avec acuité le rapport Stahl publié en 2020. Sous l'égide du Conseil d'État, il faut avant tout rechercher. Une plus grande efficacité des mesures juridictionnel. Cette réflexion rejoint celle de l'excellent rapport. Du président François Noël Buffet. Qui draine les champs. Droits des étrangers devenue illisible. Des procédures inefficace et un manque de moyens des services de l'État pour les mettre en oeuvre. Fort de ce diagnostic partagé par toutes les juridictions administratives. Parlementaire. Par nous. Le gouvernement va comme l'a indiqué, mon collègue Gérald Darmanin ouvrir prochainement le chantier de la réforme du contentieux des étrangers. Il n'y aura évidemment aucune question taboue. Ainsi, la réforme du contentieux de l'asile devra également être mis à l'ordre du jour.-- Toutes ces questions sont en débat aujourd'hui et le seront lors de l'examen du projet de loi et je sais bien sûr que vous aurez à coeur de bâtir une procédure à la fois efficace respectueuse de nos principes. Si je devais en une phrase résumé le propos. La protection des droits et la protection qu'offrent le droit oui bien sûr.-- L'instrumentalisation du droit et le dilatoire non.-- Le second axe de travail que je. Vous propose concerne bien sûr la sphère pénale. Mais c'est moi tout d'abord insisté sur un constat.-- Il faut le faire lucidement. Oui bien sûr il y a des étrangers délinquants. Oui il y a des étrangers dans nos prisons, de ce point de vue d'ailleurs. La moyenne. Qui est la nôtre est une moyenne européenne. Mais disons-le l'écrasante. L'écrasante majorité.-- Des personnes que nous accueillons sur notre sol M. notre pays. Et. On respecte les lois. Au revoir. Et je dis ça avec force parce qu'il ne faut pas accepter, me semble-t-il des amalgames parfois facile. Ou des généralisations entre immigration et délinquance Pour autant, messieurs les sénateurs, Mesdames les sénatrices je me garde de tout angélisme et je souhaite que nous puissions dans le cadre du projet de loi. Permettre un autre droit pénal d'être plus efficient à l'égard des étrangers qui ne respectent ni nos lois ni de notre pacte républicain. Pour y parvenir, il nous faut réfléchir à un élargissement de la peine d'interdiction du territoire français. Il s'agit aujourd'hui vous le savez, d'une peine complémentaire. Prévue dans de nombreuses infractions qui constituent les infractions les plus graves. Crimes contre l'humanité infractions terroristes atteinte volontaire à la vie par exemple. Pourquoi. Ne pas harmoniser les conditions d'interdiction judiciaire du territoire français avec celle des mesures d'expulsion. N'est-il pas légitime. Qu'un juge correctionnel puisse protéger notre territoire et nos concitoyens aussi bien qu'un préfet qui décide d'une expulsion pour un étranger délinquant. Pourquoi également ne pas explorer l'élargissement du Champ infractionnelle de cette peine complémentaire avec bien sûr toutes les précautions qui s'imposent. Car cet élargissement ne pourra avoir lieu sans que soit garantie les grands principes de l'État de droit auquel nous sommes tous particulièrement attaché. Voilà ces pistes sont sérieusement à l'étude. C'est tout l'enjeu des débats qui vous attendent, être ferme à l'égard des étrangers qui s'affranchissent de nos règles tout en garantissant à chaque femme. À chaque homme qui souhaitent s'installer régulièrement sur notre territoire un examen individualisé de sa situation personnelle et familiale mesdames et messieurs les sénateurs. Les Français nous attendent. Ils nous regardent, ils les donnent de notre responsabilité collective de nous montrer à la hauteur de leurs attentes bien légitime. Monsieur le président, madame, la Première ministre, messieurs les Ministres mesdames et messieurs les sénateurs. Une politique d'intégration doit naturellement envisager le travail comme un outil essentiel pour cette intégration car c'est à nos yeux le seul moyen durable pour un étranger arrivant sur notre territoire d'assurer sa subsistance. Il faut aussi souligner et rappeler que le contexte professionnel facilite grandement l'apprentissage de la langue et l'apprentissage de la culture d'un peuple. Par ailleurs, la France comme de nombreux autres pays a besoin de talents étrangers. Cela ne signifie aucunement que nous sommes de notre obligation de former et d'accompagner nos compatriotes les résidences notre territoire, c'est notre priorité dans notre marche vers le plein emploi, mais cela signifie aussi que nous devons accompagner cette politique d'un recours subsidiaire recrutement d'étrangers non communautaires pour faire face à nos besoins de compétences. En réalité, nous le savons, nous avons déjà des procédures pour permettre l'introduction de main d'oeuvre étrangère et de talons venus de l'étranger. Nous savons aussi délivrer des titres de séjour à des personnes présentes depuis plusieurs années sur le territoire. Mais nous ne pouvons pas nous soustraire plus longtemps à une analyse lucide de notre système et constaté qu'il était inefficace par plusieurs aspects et injuste par d'autres. Il n'est d'abord pas efficace car il ne mais à de nombreuses étrangères il est régulièrement sur notre territoire de former, d'être accompagné pour exercer un emploi. Cela se voit dans les chiffres dans les résultats de la politique de l'emploi aux premiers trimestres 2022. Le taux de chômage des personnes étrangères était de 13% contre 7 et demi pour l'ensemble de la population et ce rapport ne varie pas, ni en fonction des crises ni en fonction des périodes de croissance. Dans le même temps nous enfermons aussi dans l'illégalité des étrangers présents depuis longtemps sur notre territoire et travaillant notamment dans des secteurs en tension. Ils sont pourtant essentiels à la prospérité au développement de notre pays. Ils sont le plus souvent déclarés. Ils payent des impôts, des cotisations mais leur situation relève parfois aussi d'une grande difficulté d'une précarité et de la traite des être s'humains. La absence de droit au séjour, les rend vulnérables et précaires. Il arrive aussi que les employeurs peu scrupuleux les oblige à travailler parfois plusieurs semaines sans repos ou encore être hébergés dans des conditions indignes. Cela ne vaut évidemment pas généralisation mais nous savons que cela existe et que ces situations peuvent se présenter. Aussi progresser sur ce sujet, c'est progresser sur l'ensemble des conditions de travail en supprimant ces situations du pire et en revenant un socle commun pour l'ensemble des salariés. Ce constat si il est partagé nous oblige et nous devons sortir d'un système perdant-perdant tout en même temps, il nous incombe aussi de faire davantage pour lutter contre le travail illégal et qu'le travail dissimulé. Ainsi des étrangers présents depuis plusieurs années sur le territoire travaillant depuis plusieurs mois en France dans un métier en tension sont en situation régulière et irrégulière et sans porte de sortie. Il travaille il s'intègre veulent s'intégrer sont intégrés et il demeure pourtant, sans droit au séjour ni au travail. Nous souhaitons que ces étrangers puissent obtenir un petit temporaire pour une année renouvelable pour leur permet de travailler légalement dans les secteurs de en dans les secteurs rencontrant les plus grandes tensions de main-d'oeuvre. Ils pourront ensuite s'insérer dans un parcours plus classique, toujours par le travail par la longue, ça s'appelle tout simplement l'intégration et c'est ce que nous voulons promouvoir, comme nous l'avons indiqué avec le ministre de l'Intérieur. Je le dis au passage certains feignent de penser que nous allons ainsi favoriser le travail des étrangers au détriment du travail des Français. C'est faux, par construction les secteurs en question ont besoin de main d'oeuvre, ils en ont déjà besoin les étrangers dont nous parlons ne prennent le travail de personnes ils occupent un emploi. Pour lequel il est bien difficile de recruter. Et par ailleurs ne nous n'avons donc évidemment pas l'important effort de formation de l'ensemble des actifs et c'était objectif de plein emploi pour tous. De plus, l'introduction de ce type de séjour est aussi une demande forte de nombreuses entreprises qui souhaitent ainsi pouvoir régulariser accompagné la régularisation de celles et ceux qui travaillent pourraient. Dans ce même état d'esprit nous avons d'ores et déjà initié la révision de la liste existante des métiers en pension. Elle comporte quelques incongruités quelques manques. Les métiers de la restauration. Ils sont par exemple aujourd'hui peu présents, tout comme ceux de la près de propreté. Alors cette liste doit être plus en phase avec la réalité des tensions de recrutement. Ensuite, si nous devons regarder la réalité en face. Pour ce qui concerne la part des employes tension occupée aujourd'hui par des étrangers en situation régulière ou irrégulière. Nous devons aussi constaté la faiblesse ou plutôt la lenteur des sanctions infligées le ce que le travail illégal et constater. C'est une certitude, la lutte conte le travail illégal passera par des sanctions plus facilement et plus rapidement applicables. Il existe aujourd'hui des sanctions pénales que nous ne prévoyons que nous ne prévoyons pas de modifier, elles sont nécessaires au traitement des situations les plus graves. Dès lors que l'intentionnalité la dégradation des conditions de travail sont manifestes. Il existe aussi des fonctions administratives, par exemple la possibilité pour les préfets de fermer l'établissement pour une durée maximale de trois mois. C'est une sanction lourde que nous devons faciliter. Il nous faut aussi une sanction administrative mais calibrés pour être plus systématique comme une amende de plusieurs milliers d'euros pour un emploi illégal. Elle n'aurait pas un caractère automatique mais seraient déployés en fonction de l'appréciation d'un certain nombre de critères tels que les ressources, les charges mais aussi et peut-être surtout l'intentionnalité le contexte et la gravité. Enfin, je termine par là, l'intégration et c'est une évidence. Le ministre de l'Intérieur a dit se fait aussi par la langue en cohérence avec cette exigence de maîtrise de la langue. Nous considérons que les employeurs doivent aussi faciliter l'intégration leurs salariés étrangers par la langue. Bien des employeurs comptent sur la main d'oeuvre étrangère pour faire tourner leur entreprise. Il n'est donc pas normal que les employeurs puissent contribuer à la réussite de l'intégration de leurs salariés par la langue. Nous avons ouvert un dialogue avec les partenaires sociaux pour voir comment par les opérateurs de formation par le financement de la formation continue à la possibilité de libérer des heures sur le temps de travail pour participer aux formations, nous pouvons mettre à contribution les employeurs pour la formation en français. De leurs salariés étrangers. Nous abordons ce débat sans naïveté en voulant ne plus être les complices passifs d'injustices existantes. Quant au travail des étrangers sans naïveté ni Diane idéalisme mais avec du réalisme et la volonté de protéger les travailleurs comme les chefs d'entreprises qui n'ont pas d'autre alternative. Nous allons aborder maintenant la suite de nos débats. Et je vais donner la parole aux orateurs des groupes. Tout d'abord le président François. Le buffet. Pour les républicains. Monsieur

Monsieur le président, madame, la Première ministre, mesdames et messieurs les Ministres, chers collègues. Il n'existe pas le pays qui peut accueillir l'ensemble des migrants économiques. Il n'existe pas. Nous n'avons, nous avons besoin d'améliorer l'intégration dans la République plus vite et mieux. Je ne veux plus de femmes et d'hommes dans les rues. Mais partout dès la première minute un traitement administratif qui permet de déterminer si on peut aller vers une demande d'asile ou non et derrière une vraie politique de reconduite aux frontières.-- Ces 3 phrases ne sont pas les miennes. Certains peut être s'en souviendront, elles ont été prononcées, il y a déjà 5 ans par le président de la République lui-même à Orléans.-- On aurait pu être séduit. Il y a 5 ans par ses propos qui semblaient annoncer une grande ambition de moderniser et, dirais-je, de penser enfin. Dans sa globalité. Notre politique migratoire. Mais regardons les choses en face, la triste réalité, c'est que notre politique d'immigration, d'asile et d'intégration est aujourd'hui dans l'impasse. Je vous concède madame, la Première ministre que cette faillite trouve ses racines dans les errements d'un quinquennat de monsieur le président Hollande dont vous avez en partie hérité mais force est de constater que 5 ans après le discours à Orléans. Le gouvernement n'a pas pu se donner les moyens de redresser totalement la barre. Nous avons d'abord renoncer à la maîtrise de l'immigration légale dont chacun sait qu'elle nourrit pour partie l'immigration irrégulière. Pour la seule année 2021 et je reprends les chiffres publiés en juin 2022 par le ministère de l'Intérieur, 270.000 premiers titres de séjour ont été délivrés en France métropolitaine, 100.000 de plus qu'en 2011, le stock de titres valide a lui grimpé de 1 million pour atteindre aujourd'hui 3.400.000. L'ampleur de ces chiffres et de la évolution parlent d'elles-mêmes certains sur ces bancs soutiendront que l'immigration est une chance pour les pays européens sans doute. Mais à condition que cette immigration soit un apport pour ce pays et non une charge. Or, comme le souligne l'OCDE. La contribution de l'immigration à la société et l'économie d'un pays quel qu'il soit est étroitement liée à son niveau de qualification et le niveau de qualification constaté en France. Hé bien moindre que chez nos voisins européens. Quant à l'intégration, elle ne peut véritablement à devenir qu'avec la maîtrise de notre langue et le respect des principes et des valeurs qui font notre nation. Alors vous l'avez dit vous-même la semaine dernière, monsieur le ministre de l'Intérieur. Un quart des étrangers en situation irrégulière parlent ou écrivent très mal le français.-- Côté immigration irrégulière. Nous allons d'échec en échec avec d'abord une maîtrise insuffisante de nos frontières. Je veux dire presque aujourd'hui presque nos frontières européennes, c'est un euphémisme en 2006 sur ces mêmes bancs. Le gouvernement de l'époque, estimait le nombre de clandestins présents sur le territoire national, entre 200 et 400.000 devant la commission des lois, le 2 novembre dernier, vous avez Monsieur le Ministre évaluer ce chiffre entre 600.000 et 900.000. Il a donc multiplié par au moins 2 ans 15 ans et la poche est encore plus amer, s'agissant de l'éloignement. Le taux d'exécution des OQTF se situe, selon les chiffres transmis par le ministère un niveau famélique de 6,9% au 1er semestre 2022. On peut toujours discuter la pertinence de ce taux. Mais nous ne pouvons pas ne pouvant que constater à indicateurs constants nous exécutions encore 22% de nos OQTF. En 2012,

C'est d'autant plus regrettable que nous renouant avec les niveaux exceptionnels des demandes connus avant la pandémie. Nous devrions même dépassé l'année prochaine. Le record de 2019 avec 135.000 demandes attendues. Je ne dresse pas madame, la Première ministre ce tableau ni par malice ni par fatalisme car se laisser aller à l'une ou à l'autre ce serait renoncer à chercher des solutions pour se réfugier derrière des postures stériles ce ce serait alimente ce serait des peurs qui n'ont pas lieu d'être et ce serait surtout ouvrir la porte en grand aux extrêmes. Vous l'avez dit à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Madame, la Première ministre. Si nous voulons débattre sérieusement de la politique migratoire. Nous devons nous astreindre à un langage de vérité un langage de vérité, appuyé sur des données partagées et indiscutable qui affirme le constat lucide d'une immigration qui n'est pas maîtrisé et d'une politique publique qui a perdu tout son sens. Un langage de vérité qui énonce clairement les objectifs à atteindre et dénonce les postures l'immigration zéro est une chimère. L'accueil au fil de l'eau est une folie. Dans ce contexte, ce qui nous fait aujourd'hui cruellement défaut c'est en réalité une réelle stratégie migratoire car faute d'anticipation et faute de volonté clairement exprimée. Nous ne faisons que subir les soubresauts des flux migratoires. Nous avons été dépassés par l'intensité des flux en 2015. Nous ne sommes encore aujourd'hui avec la reprise post-Covid. Nous venons de vivre encore un événement très particulier avec l'Océan Viking notamment dans les conditions. Dans lesquelles les procédures ont été suivies tellement complexe. Ce n'est pourtant pas un gros mot que de dire que comme tout État souverain, c'est à nous qu'il revient de dire qui nous accueillons sur notre territoire et qu'il n'y a pas sa place. Pour nous, il y a 3 principes. Le premier une immigration régulière choisis prioritairement économique et qui trouvera d'autant plus sa place dans notre société qui elle y contribuera pleinement. La 2ème de l'intransigeance dans la lutte contre l'immigration irrégulière et le 3ème de l'efficacité dans l'application de la procédure d'asile. Voilà les trois piliers sur lesquels doit reposer ne semble-t-il notre stratégie migratoire. Ces stratégies, c'est celle que défend le Sénat en tous les cas sa majorité depuis de nombreuses années. C'était le sens des propositions que nous avions portée de l'examen de la loi Collomb en 2018 et qui ont été pour partie balayé d'un revers de main par l'exécutif, à l'époque je constate néanmoins avec satisfaction plus qu'une infection de la part du gouvernement qui envisage désormais de reprendre plusieurs de nos propositions dans le texte, qui devrait venir devant le Sénat en première lecture, nous vous en remercions. Au mois de mars prochain. Certaines pistes du gouvernement peuvent être intéressantes, d'autres sont moins acceptable mais j'y reviendrai. Monsieur ministre de l'Intérieur vous rappeler régulièrement. Vous êtes inspiré pour la rédaction de votre texte du rapport, services de l'État émigration retrouver sens et efficacité que votre serviteur a rédigé au mois de mai dernier. C'est, je dois le dire bien un bon début, mais pour éviter tout malentendu. Et comme l'on est jamais mieux servi que par soi-même. Je vais vous faire des propositions assez concrètes ancré dans les positions constamment soutenu par le Sénat depuis plus de 10 ans et qui vise à doter la France d'une stratégie migratoire réellement ambitieuse et efficace. Madame, la Première ministre, vous avez déploré la semaine dernière devant l'Assemblée nationale, le manque de propositions, les notes vont être sur la table. Permettez-moi de vous en présenter quelques grandes lignes. La première priorité est de retrouver notre souveraineté en matière d'immigration régulière décidé il l'on accueille sur le territoire en assumant de prioriser l'immigration économique. Pour mémoire, celle-ci représentaient à peine 13% des premiers titres le séjour délivrés en 2021. C'est au Parlement qu'il revient de fixer ses orientations annuelles avec disons-le franchement. Le débat sur des quotas ou en tous les cas de grandes orientations.-- Recouvrer notre souveraineté c'est aussi assumer de restreindre les voies d'accès au séjour je pense à la procédure étrangers malades pour laquelle il est urgent de revenir aux critères de l'absence de soins dans le pays d'origine. Rien que pour 2021, nous avons reçu 5000 demandes émanant des pays du G20, qui dispose pourtant de système de soins, développer. Je pense aussi au regroupement familial pour lesquelles nous proposons de resserrer les critères naturellement dans le respect du droit européen. Mais avoir une politique d'immigration régulière cohérente. C'est aussi mieux traités. Ce que nous acceptons sur notre territoire. Je ne reviens pas sur les situations ubuesques générées par les difficultés aux guichets des préfectures pour obtenir ou renouveler un titre de séjour. La solution est pourtant là avec une refonte des pratiques d'instruction autour d'une logique dite 360 degrés que votre gouvernement a expertisée ou. Auprès de la préfecture danger pardon où l'on examinerait dès la première demande et une fois pour toutes l'ensemble des motifs qui pourrait fonder la délivrance d'un titre de séjour est une très bonne démarche. Mieux traiter les étrangers en situation régulière demande également de muscler notre dispositif d'intégration. Ou proposer. Monsieur le Ministre, d'augmenter le volume d'heures de français et c'est une bonne chose. La contrepartie c'est le renforcement des devoirs de l'étranger. Vous avez repris la proposition du Sénat de conditionner la délivrance des titres de séjours de longue durée à la réussite à un examen de langue fort bien nous estimons nécessaire d'aller encore plus loin et de la. Également à la réussite d'un examen civique pour lequel l'étranger démontrerait sa bonne appréciation des valeurs de notre histoire et de la culture de la réplique de la France. Passez une logique de moyen à une logique de résultat c'est, je ne crois. La vraie révolution pour le contrat d'intégration républicaine. Cette expropriation des valeurs républicaines n'est pas négociable et l'obtention d'un titre de séjour n'est pas un blanc-seing. Elle vient avec des responsabilités à cet égard, nous aurons quelques difficultés à vous suivre dans votre idée d'automaticité de renouvellement de titres plus annuel en tous les cas à ce stade. Attendons de voir le texte lui-même la 2ème priorité c'est fluidifier le traitement des demandes d'asile et de lutter plus efficacement contre le détournement de notre politique d'accueil. Il est crucial de faciliter l'instruction des demandes de protection internationale en permettant notamment à l'Ofpra de statuer plus rapidement sur les dossiers les moins problématique par exemple en cas de retrait de la demande ou d'abandon du lieu d'hébergement, mais aussi en lui imposant de refuser l'asile en cas de menace pour l'ordre public. Ce faisant, l'Office pourra concentrer son expertise sur les dossiers les plus complexes. Je tiens à cet instant à cette tribune, a salué le travail qui est fait par l'Ofpra. La qualité des agents qui travaillent au sein de cette de cette Nous devons de faire de la lutte contre l'immigration irrégulière une priorité nationale et d'agir enfin pour la mise en oeuvre et des décisions d'éloignement. Prévenir l'immigration irrégulière. C'est d'abord assumer d'établir un rapport de force avec les états d'origine. Le Sénat avait voté en 2018 une disposition autorisant les restrictions de visas à l'égard des pays délivrant peu de laissez-passer consulaires le gouvernement à l'époque ne l'avait pas retenu. Il s'y est finalement résolu. Et là encore cela a produit quelques résultats puisque le nombre de retours forcés vers l'Algérie certes modeste en volume ont malgré tout été multiplié par 16 en moins d'un an. La montée en puissance de la lutte contre l'immigration clandestine ne se fera pas non plus sans réforme de l'aide médicale d'État avec 400.000 bénéficiaires et un coût supérieur à un milliard d'euros. Celle-ci atteint des sommets. Nous ne pouvons pas nous satisfaire des derniers ajustements paramétrique. C'est une des réformes structurelles dont nous avons besoin, là encore, le Sénat défend de longue date son remplacement par une aide médicale d'urgence, centré sur la prise en charge des pathologies les plus graves. L'AME. Madame la mais un Premier Ministre se justifie pour des raisons de santé publique mais on ne peut obérer le fait qu'elle constitue aussi parfois une incitation à l'immigration irrégulière. Il en va de même du projet de titre de séjour métiers en tension. Qui est une opération de régularisation finalement qui ne veut pas dire son nom. Soyons clairs, qu'est-ce que l'attribution d'un titre de séjour à une personne en situation irrégulière sinon une régularisation la problématique pourtant est réel, je veux le dire à cette tribune. La situation est bien réelle. Nous ne pouvons nier que nombres de métier parfois indispensable sont exercés en majorité par des étrangers et ne pouvons en débattre. La solution passe-t-elle pour autant par une régularisation massive sans aucun ciblage ou risque de créer un nouvel appel d'air. Je pense que non et nous savons tous que dans ces conditions là. Si cela devait être le cas. Les affaires des filières criminelles qui industrialise le passage des clandestins et jouent avec leur vie se formerait immédiatement mais il faudra, il faudra des critères. Il faudra des conditions il faudra préciser les choses dans la loi parce que la problématique est bien existante et depuis le début je dis qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont pas telles qu'on les aimerait que où les n'irait. C'est également le cas de la réforme du contentieux. Nous le savons tous le droit des étrangers, est d'une complexité qui frôle l'absurde. Il suffit de voir le le Cesid à la taille qu'il a pris. C'est une charge pour les magistrats chargés de l'appliquer une source d'insécurité juridique pour les justiciables et une aubaine pour les clandestins se cherchant à se soustraire à l'éloignement. Le gouvernement a souhaité réduire à 4 le nombre de procédures contentieuses. Nous vous proposons de descendre jusqu'à 3 mais la discussion se fera naturellement. Nous ne sommes pas là pour discuter. De ces points de détail, en tous les cas. Et madame, la Première ministre, avant de terminer mon propos. Je voudrais vous dire que je pense que ça n'est pas en masquant les problèmes que l'on va les oublier. Ce n'est pas en les nommant, que l'on va les aggraver. Mais c'est certainement avec des propositions concrètes qu'on arrivera à les résoudre. Cela tombe bien, nous en manquons pas celle que je vous ai exposées et bien d'autres feront part de nous serons dans nos propositions, il y a eu 20 une loi immigration en 30 ans, ce qui fait à peu près une tous les 16 mois. Je vous propose que nous prenons l'engagement de doter notre pays d'une vraie stratégie en tous les cas pour notre groupe, nous y sommes prêts. Merci.

Merci monsieur le président, madame. La Première ministre, messieurs les les ministres. L'asile est un droit. C'est un engagement conventionnel. Et c'est aussi une part de notre identité constitutionnelle. L'immigration c'est autre chose, c'est une politique qu'il convient de mener en respectant nos principes. Et. Et en respectant aussi au mieux les intérêts de notre pays. Avant 2018, jamais ces 2 sujets n'avait été abordée dans les mêmes lois.-- Parce que ce sont deux sujets distinctes. Malheureusement, maintenant, nous devons les aborder ensemble. Nous devons constater que la question de l'immigration est un sujet sur lequel les Français semblent relativement fermé entre guillemets lorsque la question leur est posée d'une manière globale, mais par contre ils sont fondamentalement ouvert et généreux, dès lors qu'ils font face à des situations concrètes et ils sont attachés à notre tradition d'accueil et d'asile. Rappelons quelques fait la France est restée relativement à l'écart des grands mouvements de demande de protection, que ce soit au moment de la crise syrienne ou au moment. De actuellement avec la crise ukrainienne. Nous ne sommes pas le pays qui avons accueilli le plus. D'Ukrainiens. Deuxièmement nous délivrons finalement relativement peu de 1er titre de séjour. Tous les ans par rapport à des pays de taille similaire avec une économie de telles de même nature. Enfin. Plutôt que de penser que. L'émigration croissent de manière exponentielle. Au début du XXe siècle.-- 5% de la population mondiale était migrantes aujourd'hui c'est moins de 3,5%. Enfin, l'immigration familiale en France. Elle n'est pas open bar, il faut plus de 18 mois de présence en France et des conditions précises de ressources et de logement. Madame, la Première ministre sur ce goût. Votre gouvernement.-- Sur ce sujet c'est le c'est la politique du désordre et de l'affichage désordre. Des préfectures dysfonctionnel où il est impossible de prendre rendez vous des personnes en situation irrégulière qui deviennent irrégulières parce qu'elles ne peuvent pas avoir de documents renouveler

désordres lorsque depuis vous êtes monsieur le ministre de l'Intérieur, ministre depuis 2 ans, rien n'est fait pour régler la question des personnes qui sont ni expulsables ni régularisables, il faut absolument faire un examen à 360 degrés de l'ensemble des situations et pour cela il faut du du personnel désordre lorsque, lors d'une préfecture à l'autre. Nous ne traitons pas de la même manière les demandes des les examens de demande d'admission exceptionnelle au séjour parfois même c'est impossible désordre lorsque pour le chiffre et l'affichage. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous exigez pour des préfets plus d'OQTF, contenter de se concentrer sur ce qui est faisable en 1er lieu sur les personnes. Qui représente réellement un risque pour l'ordre public et pas simplement lorsqu'elles sont inscrites otages. À vouloir faire du chiffre, on ne fait pas correctement l'essentiel vous instrumentaliser les instrumentaliser les dublinés pour faire du chiffre, ils reviennent une semaine après et les personnels de la PAF. Ils ont perdu. Absolument, le sens de leur action.

Désordre lorsque vous rappeler le rapport Stahl lorsque vous appelez à simplifier le droit des étrangers, et nous sommes d'accord avec cela. Mais alors pourquoi annoncer un acte administratif comme. Une OQTF dès lors que l'Ofpra refuserait une protection. Ce serait un acte administratif qui n'aurait de de que le nom si nous respectons la Convention de Genève désordre aussi lorsque ces défaillances de l'État pèsent sur l'intégration lorsqu'elles. Lorsqu'elles conduisent les personnes à s'appuyer sur leur communauté plutôt que sur les services publics et font peser le devoir d'humanité sur les collectivités locales et sur les associations. Monsieur le Ministre, j'arrête les les choses désagréables. Je constate une évolution entre l'Assemblée nationale et le Sénat, à l'Assemblée nationale vous aviez évoqué que vous ne mettrez plus ancrée à des personnes de moins de 16 ans vous avez précisé ici que ça ça adopterait à tous les mineurs. Je salue cette évolution en une semaine. Il faut aussi saluer que pour la première fois depuis longtemps. Ces questions ne pas ce ne sont pas exclusivement des questions du ministère de l'Intérieur, parce qu'une intégration réussie, elle passe monsieur et vous, ça a été rappelé, Monsieur le Ministre, messieurs, madame, la Première ministre par le travail. Elle passe par le travail. Elle passe par l'école. Historiquement, c'est ainsi que ça s'est passé en France. Et on doit constater que face aux deux plus grands mouvements actuels au Venezuela avec la Colombie et l'Ukraine avec l'Union européenne dans les 2 cas les accueille se font avec une reconnaissance du statut toute de suite et le droit au travail tout de suite, c'est la meilleure manière de faire et le droit au travail, c'est la meilleure manière d'éviter le dumping social. La meilleure le droit au travail, c'est la meilleure manière de liquider l'esclavage moderne dont nous sommes témoins chaque jour dans des actes essentiels de la vie. Et vous avez madame, la Première ministre énormément de marge de manoeuvre pour faire beaucoup plus que ce que vous avez fait au cours des dernières. Années sans changer la loi. D'abord, la liste des métiers. Attention, elle n'a bougé qu'une fois en 2021 depuis 2008. Deuxièmement les situations de des jeunes apprentis en situation irrégulière qui choque la population hé bien elles ne sont pas mieux aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années, enfin. les les par rapport à ces annonces qui sont faites. Quels moyens nouveaux seront données aux préfectures pour réellement changer la donne. Le titre. De séjour métiers en tension s'adressera-t-il d'abord à des nouveaux arrivants. A-t-il vocation à ouvrir un droit au séjour à des personnes déjà engagés dans ces activités, la personne la perquisition du gouvernement qui refuse la présomption de salariat pour des travailleurs des plateformes sera-t-elle maintenue rendant insolite de la situation de milliers de clandestins qui aujourd'hui participe à notre économie.-- Mes chers collègues, la France et dans l'espace Schengen. C'est un espace de libre-, circulation et une commission d'enquête du Sénat il y a quelques années, a rappelé l'intérêt et l'utilité de cet espace de libre-circulation dès lors qu'il y avait entre nos pays des échanges d'informations solides et la confiance et d'autre part une surveillance sérieuse des frontières extérieures et nous avons entre 2012 et 2017. Réformer l'interro bilatéral habilité des systèmes mis en place le PNR lancé le projet Ethias et renforcer le mandat de Frontex, l'Europe, sur ces questions n'est pas un problème. C'est une solution. État doit donc respecter le droit européen. Le pacte Asile migration avocat renforcer encore la cohérence de cette action et ce que nous avons constaté l'année dernière avec. Ce qui se passait à la frontière des pays baltes et de la Pologne avec la Biélorussie, souligne qu'il peut y avoir des nouvelles arrivées des nouvelles situations imprévues qui mérite d'être de manière construite solidaire entre les pays européens mais cela oblige chaque pays européen à respecter le droit européen. Le droit européen, l'Italie, elle doit respecter le droit de la mer, mais la France elle doit le respecter aussi le droit européen lorsqu'il s'agit de respecter le fait que, en Europe il y a la libre-, circulation et on ne peut pas systématiquement on va mettre en place. Des contrôles aux frontières intérieures de l'Union. La Cour de justice de l'Union européenne la correctement rappelé et il est important de respecter le droit européen, si on veut. Elle a rappelé au Conseil d'État autrichien, Monsieur le Ministre, vous voulez pas l'entendre. Mais regardez ce qui se passe avec l'Autriche, la politique de visas, Monsieur le Ministre, ce que vous avez mis en place en partie depuis quelques mois, qu'est-ce que c'est des délais incroyable de refus arbitraires des projets de vie détruit voilà aujourd'hui une politique de visas qui détruit progressivement les Liens historiques que nous avons avec les pays du sud de la Méditerranée. Ce n'est plus Paris, mais Istanbul Dubaï même parfois Moscou qui font référence aux yeux de beaucoup et nous n'avons qu'un en prendre qu'à nous-mêmes et à votre politique dans de très nombreux pays les communautés d'affaires se plaignent de contrat qui ne peuvent plus être. De visites signe que peuvent plus être faites. Cela doit cesser. Plus de 17.000 morts en Méditerranée. Au cours des 6 dernières années, des milliers d'enfants disparus, sur la route des Balkans. Monsieur le Ministre, madame, la Première ministre. Cela doit cesser. La lutte contre les passeurs n'est pas compatible avec le financement de structures étrangères opaque au jeu trouble tels que les garde contre les les gardes frontière libyen obtenir des laissez-passer consulaires lorsque cela est nécessaire, ne peut pas se faire dans un d'une démarche. De coups de menton. Elle doit se paraissait dans une démarche bien compris avec les pays d'origine et de transit. Une démarche qui doit donner une place significative. À des politiques de mobilité légale.-- Enfin.-- La ville qui depuis notre révolution est au coeur de notre identité. Elle est essentielle. Cette politique. Les personnes qui méritent d'être protégés.-- Et elles viennent après avoir vécu des chocs terrible. Elles ne peuvent pas être en mesure en quelques jours de préparer leur récit correctement. Alors Monsieur le Ministre, que vous annoncez un guichet France asile très bien.-- Mais auront-elles le temps de se préparer. Deuxièmement vous nous annoncez une réforme de la CNDA. Nous refusons le juge unique systématique. Nous ne voulons pas que le HCR soit mis en dehors des CNDA et nous considérons aussi qu'il faut avancer sur une reconnaissance sur une reconnaissance européenne.-- Des instructions des demandes d'asile et cela doit passer par une cour européenne du droit d'asile. Enfin. En. Il était son fief. Qu'aucune minute ne soit perdue pour une personne qui entendent demande des îles pour lui reconnaître le droit au travail, le droit à la formation et le droit à l'apprentissage de la langue. Aucune minute de toi. Pour lui Pour lui donner la possibilité d'être autonome le plus vite possible. Enfin.-- Il y a encore beaucoup de choses à dire en particulier sur les questions liées à l'outre-mer.-- Mais si nous sommes une république. Il n'y a qu'un seul territoire sur lequel il n'y a qu'une seule loi.-- La situation à Mayotte et très compliqué mais il est Nisa acceptable qui à un titre de séjour à Mayotte ne donne pas le droit de voyager dans l'Hexagone. Toutes les larmes qui sont versés sur Mayotte ne sont qu'hypocrisie. Si les étrangers qui sont en situation régulière à Mayotte ne peuvent pas tous venir en France s'ils le souhaitent.-- Voilà. Une politique humaine, cohérente et résolue profondément européenne avec ce type de politique. Nous pouvons retrouver la voie de la confiance en nous-mêmes corriger nos erreurs afin de récupérer une capacité d'intégrer celles et ceux qui viennent se réfugier viennent travailler et étudier en France et contribue ensuite à l'édification de notre pays. C'est ainsi que notre pays s'est construit Gass à des apports à des diversités étrangère et c'est avec cette force et avec cette volonté que nous pouvons continuer si nous avons confiance en nous, si nous avons confiance dans notre histoire, si nous avons confiance dans nos principes et si nous avons confiance et nous donnons confiance à l'Europe. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Philippe Bonnecarrère pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le président, madame, la Première ministre, messieurs les Ministres. L'immigration mettent en tension. La souveraineté qui font de l'État et la citoyenneté qui font de la nation. Avec mes collègues centristes. Nous souhaitons présenter nos propositions. Dans le délai bref imparti. Elles seront cursive et je viens d'excuse par avance. Nous ne partageons pas l'idée suivant laquelle l'action de l'exécutif serait empêché ou interdites par l'état de droit. Les 2 sont compatibles. Aussi nous ne vous ferons aucune proposition de nature constitutionnelle. Le 1er niveau de solutions est européen. La révision du paquet asile est un échec probablement durable. Relevons quelques avancées avec la montée en puissance de Frontex. La création de l'Agence européenne pour les. Il avait l'objectif d'harmoniser les politiques en particulier la liste des pays dits sûrs. Nous proposons une reconnaissance mutuelle des décisions de rejet d'une demande d'asile afin d'éviter l'émigration dite de rebond. Si cet objectif n'est pas atteignable. À 27 il pourrait l'être par une coopération renforcée. Madame le 1er Ministre à partir de neuf États ou par des accords bilatéraux. Nous souhaitons aussi l'entrée en vigueur effective en 2023. Monsieur le ministre de l'intérieur du système entrée sortie système dit E S enfin robuste avec la précision qu'en cas de refus de se soumettre au relevé d'empreintes. L'intéressé se verraient refuser l'accès au territoire européen. Pour revenir en France la première voies d'immigration et familiale otite du droit à la vie privée. Nous faisons de propositions. Porté de 18 à 24 mois le délai de présence régulière sur le territoire à partir duquel pourrait être fait la demande de rapprochement c'est le délai plafond fixé par la directive de 2003. La 2ème proposition consiste à explorer les mesures conditionnelles visées par la directive de 2003, à savoir disposer de ressources suffisantes dans le logement, le respect de l'ordre public est fait pour la personne faisant l'objet de la demande de rapprochement de se conformer aux mesures dites d'intégration. Chaque mot a son importance. Nous pensons en particulier à la maîtrise préalable de la langue française otite du contrat d'intégration mais je reconnais bien volontiers que notre collègue François Noël Buffet a eu raison d'évoquer tout à l'heure, la connaissance de la culture française. Les visas étudiants qui ne semble pas faire de difficultés. La 2ème loi d'immigration et celle des permis de séjour. Votre proposition majeure madame, la Première ministre, messieurs les Ministres. Porte sur un permis de séjour pour les métiers en tension. Nous serions favorables à des permis de séjour pour des métiers en tension. Qualifié qualifié. Chacun est conscient de cette vieille pratique française. En as t'a confié les métiers que nos concitoyens ne souhaite pas assuré à bas prix à des étrangers. Avec ce système. Rien ne changera. C'est une trappe à bas salaire assuré ces métiers ne seront jamais attractif financièrement pour nos concitoyens ne monteront pas en qualifications en gamme ne feront l'objet d'aucun investissement d'automatisation. Les bas salaires entraînent des problèmes de logement, la nécessité de faire appel aux autres ressortissants du pays d'origine et nous sommes repartis vers du communautarisme. Mes chers collègues. L'idée d'une main-d'oeuvre immigrée.-- Bon marché sans cesse renouvelée.-- Est nuisible à notre pays. Bien rémunérés renouvelé lorsqu'elle est nécessaire, elle peut être positive. Notre proposition serait de vous suivre. Madame Première ministre, messieurs les ministres, à condition que le salaire versé soit égal ou supérieur à la moyenne des salaires payés dans notre pays, ou a minima dans la branche concernée. Ceci nous semblerait aussi le gage d'une bonne intégration. Notre groupe est aussi favorable à ce qui vous a été présenté tout à l'heure un débat annuel ou biennal sur les objectifs en matière de permis de séjour qui ne sortent notre sens à aucun obstacle constitutionnel. Les Français ont en effet leur mot à dire et c'est la responsabilité de la représentation nationale, c'est votre responsabilité chers collègues de l'exprimer. Nous vous suivons aussi sur la conditionnalité des visas, voire de l'aide au développement sur la demande d'asile. Nous serions ouverts à la possibilité pour le demandeur de travailler sans. Sans attendre un délai de 6 mois. Une manière, même si l'objet de la demande d'asile est différent de jauger si je puis me permettre sa capacité à s'intégrer. Nous ne vous suivrons pas du tout. Par contre sur une approche que je qualifierai de communicante le aller vers Monsieur le Ministre de l'Intérieur pour le fera et la CNDA. Le fera a fait de gros progrès dans ces délais de traitement et nous espérons que l'objectif de traitement à 60 jours pour être respectés. Nous doutons qu'il le serait si vous commencez à saupoudrer des agents de l'Ofpra dans les préfectures, les officiers dit de protection instructeurs sont des spécialistes. Cette expertise ne peut pas être fragmenté et le froid il perdrait en efficacité. De même l'idée d'éclater la CNDA je Module de la territorialisée pour reprendre vos mots. Monsieur le ministre de l'Intérieur tout à l'heure nous paraît tout aussi. Il est extrêmement difficile de faire coïncider dans la vraie vie, tel type de dossiers concernant des ressortissants de tels pays avec la présence de tels interprètes et de tels cabinets d'avocats spécialisé dans le traitement des ressortissants dudit pays la CNDA est effectivement le maillon faible de la chaîne et nous sommes de la chaîne de l'asile et nous sommes très loin de l'objectif de cinq mois prévus sur un procédure classique et de 5 semaines en procédure accélérée. Vous proposez des audiences à juge unique et de 6, Pete et de systématiser les visio-audience nous sommes réservés sur le 1er point mais très favorable au second qui est à notre sens la clé d'un traitement dans les délais raisonnables. Le Conseil constitutionnel n'a pas conditionné la tenue d'une visio-audience à l'accord du demandeur d'asile et c'est pourtant ce qui a été obtenue par les avocats dans un protocole dit d'expérimentation. Tout ceci passe à notre sens par une négociation monsieur le garde des Sceaux, avec la profession d'avocat. Nous sommes sceptiques à l'idée d'une OQTF dès le rejet par le froid. Nous envoyons mal qu'elle pourrait être l'efficacité pratique puisque de toute façon. Il y aurait une possibilité de recours et préférions qu'une décision de rejet par la CNDA soit. Assortie de plein droit de l'OQTF sans avoir besoin de saisir de saisir l'autorité préfectorale. Sur la dernière catégorie de l'immigration, les régularisations de la circulaire dite Valls. Nous rappelant ce qui a déjà été voté par le Sénat, à savoir que la seule condition d'une résidence de plus de 5 ans en France ne devrait pas être la seule condition de la régularisation sur la question de l'éloignement nous approuvons ce qui a été dit par tous, la simplification du contentieux dans la, dans la logique de accepter le. Le président François Noël Buffet de l'excellent rapport que vous avez rédigé, nous souhaiterions également une évaluation de la pratique des certificats d'hébergement fourni au soutien des visas de long séjour. Est-ce qu'il existe une harmonisation des pratiques dans notre pays. Quel est le niveau de contrôle. C'est un sujet pour lequel la participation des collectivités locales et nécessaire, nous pensons, madame, la Première ministre, mes chers collègues, quelle serait aussi utile. Cette participation des collectivités locales sur le contrat d'intégration républicain auquel il nous sommes justement manqué cette dimension locale pour s'assurer de la réalité et des résultats. Sur la question de l'aide médicale d'État, un classique du Sénat nous sommes peut être plus réservé que certains de nos collègues quant à l'idée de la modifier une nouvelle fois, nous pensons que sa limitation aux soins dits nécessaire est correct et il n'y a pas de grande différence entre nécessaire et urgent. Elle est aussi complété par un délai de carence par contre nous suggérons comme l'a formulé le président buffet et je voudrais insister là-dessus de regarder une procédure méconnue celle dite de l'étranger malade par lequel notre pays offre une faculté de permis de séjour avec des accompagnants quand la possibilité d'apporter des soins satisfaisants n'existe pas dans le pays d'origine, c'est une exception française, chers collègues. Aucun autre pays ne la pratique à travers le monde et elle était à guichet ouvert. C'est le terme même figurant dans le rapport de louche. Nous Sud-Gironde conditionner la procédure d'étranger malade à une convention préalable entre le système social français et le système social du pays d'origine. Nous sommes également ouvert à la proposition bien connu du président buffet d'une peine complémentaire qui l'a détaillé en d'autres temps et monsieur le garde des Sceaux a un a tracé aussi quelques. Éléments permettrai de. Conclure cette trop rapide près présentation mes chers collègues, vous l'avez compris. Pour les sénateurs centristes. L'immigration n'a pas vocation à être un fonds de commerce politique. Mais être régulée, pour que le contrat social qui structure la France reste solide. C'est le sens de notre proposition Madame le 1er Ministre messieurs les ministres, et le sera demain de nos votes. votes. Je vais donner la parole à notre collègue de précis. Jean François Patriat. Du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Vous avez la parole. Monsieur le prix. Bien. Monsieur le président, madame, la Première ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes soeurs collègues. Ce débat de bonne tenue auquel nous demande de participer, était nécessaire. Nous remercions le gouvernement de l'avoir inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée.-- Ce débat. Mes chers collègues. Il est l'occasion de regarder en face la question migratoire et cela en toute objectivité. Nous devons tenir un discours de vérité aux Français, un discours loin des caricatures et loin des procès d'intention.-- Dire la vérité, c'est d'abord admettent que oui l'immigration régulière et régulière est en progression mais non la France n'est pas confronté un tsunami migratoire se chauffe ce chiffon rouge est agité par l'extrême droite dans le seul but d'attiser les peurs et la colère et de diviser les Français. Le démographe. François Héran, décrit la situation de notre pays en disant. Un nombre d'immigrés en hausse. Mais pas en pointe une immigration familiale contenu un essor important des étudiants internationaux des régularisations en nombre limité. Et je voudrais à cette époque, dire à ceux qui alimente le fantasme du grand remplacement. Je voudrais leur rappeler que la proportion d'immigrés dans notre pays avoisinait 10% est nettement inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Loin du raz de marée décrit par les idéologues xénophobe. Dire la vérité. Mes chers collègues. C'est aussi reconnaître que plusieurs défis restent à relever que ce soit pour renforcer la maîtrise des flux migratoires ou pour améliorer l'accueil des réfugiés et la perception des Français sur l'immigration. Il y va. Du maintien de notre cohésion sociale et de la préservation de notre pacte républicain. 4 défis majeurs sont nouveau. D'abord préserver notre régime d'asile ensuite renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière en progression continue depuis 20 ans. En 3ème lieu, améliore les conditions d'accueil des primo-arrivants à commencer par les conditions d'accès au guichet des préfectures et enfin peut être et même surtout faciliter l'intégration des réfugiés et des étrangers en situation régulière. Contrairement à ce que certains affirment la politique du gouvernement et de sa majorité et lisible et cohérent depuis 2017 2 principes guident notre action à la fois l'humanité et la fermeté. Humanité avec les étrangers nécessitant une protection fermeté avec ceux qui n'ont pas vocation à demeurer sur notre territoire, c'est la cohérence qui amène le gouvernement à maintenir ce diptyque dans le texte que nous serons bientôt saisi, j'ai cru comprendre madame, la Première ministre et notre groupe le salut. Sans surprise, les premières propositions ont déjà été et ce qui s'est, nous n'non pas été aussitôt et ce qu'sait que les oppositions sont sont vite emparée pour les dénaturer les caricaturer ou les transformer en contre-vérité j'invite nos collègues. minorer leurs attaques sur les OQTF, chers collègues. Et il y a l'honnêteté de reconnaître que le taux d'exécution des OQTF n'a jamais dépassé 20% toutes périodes confondues, y compris lorsque chacun d'entre nous étaient au pouvoir aussi d'honnêteté de reconnaître que la faiblesse du taux d'exécution des OQTF est avant tout liée à la difficulté d'obtenir des laissez-passer consulaires. Elle est la la vérité d'ailleurs ce salut les les efforts déployés par la France pour convaincre les pays d'origine et de transit de délivrer ces précieux sésames. Ce travail de conviction commence à porter ses fruits. J'aurais préféré que nous nous faisons félicitons ensemble plutôt que d'entendre certains camper sur des positions partisanes. Je déplore d'autant plus que le gouvernement propose de s'inspirer du rapport du président buffet dont j'ai apprécié les propos tout à l'heure pour améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration clandestine. Je déplore aussi que certains de nos collègues de la majorité fassent preuve d'autant de dogmatisme sur le futur titre de séjour des métiers en tension. Notre groupe accueille très positivement à cette proposition qui relève du bon sens, Ce nouveau titre de séjour ne participe pas d'un soi-disant projet de résignation nationale et non il n'entraînera pas d'appel d'air. Nous en sommes convaincus, cette mesure est équilibré régulariser au cas par cas les travailleurs étrangers déjà présents sur notre territoire donc déjà intégré dans notre société et dans le même temps durcir les sanctions à l'encontre et les employeurs d'étrangers qu'on Stains. J'ai entendu dire ces propositions et le gouvernement. J'ai entendu les propositions qu'a fait. Tout à l'heure notre collègue et non. Mais par ailleurs je l'ai compris aussi dans les propos que la Première ministre, qu'il y avait déjà répondu positivement par avance plutôt que de lancer des procès d'intention contre CDD tâchons plutôt de réfléchir à la manière de les perfectionner. En tout cas c'est la direction qu'on pourrait être notre groupe, nous serons par exemple, attentif à ce que la perte d'un emploi n'entraîne pas automatiquement la perte de droit de séjour sur un autre plan. Nous veillerons à ce qu'une attention particulière soit portée aux aux territoires ultramarins concernés par les enjeux migratoires les fêtes par le d'de même ils nous ont ils n'ont que trop duré pour prendre l'exemple ce site par notre collègue à Mayotte. 50% de la population est immigrée mais 24.000 étrangers en situation irrégulière ont été reconduits à la frontière l'an passé, 78% de plus qu'en 2020 je ne vous parle pas ni de la Guyane ou de la Réunion ou mes collègues pourrait en parler bien pourrait compter sur les sénateurs ultramarins du groupe RDPI pour co- construire le projet de loi le futur projet de loi ensuite. Comment ne pas évoquer les causes profondes de la crise migratoire. Vous l'avez dit madame, la Première ministre, la maîtrise des flux migratoires passe par le développement des pays d'origine, ne cédons ni au simplisme, ni au populisme nous tendons souvent cette musique insidieuse sur laquelle il vaudrait mieux a loué l'argent du contribuable. Seule priorité nationale plutôt que de le gaspiller dans une aide inefficace à des payer à des pays noyautée par la corruption. Il n'y a rien de plus faux et de plus caricatural. Nous ne sommes pas dupes, les relations entre migration et développement sont complexes. C'est pourquoi l'aide publique au développement, n'a jamais été autant conçu pour être l'Alpha et l'oméga de notre politique migratoire. C'est aussi pourquoi ne traite doit impérativement s'accompagner d'une sécurisation des parcours migratoire à savoir permettre aux migrants d'effectuer des allers-retours entre la France et leur pays d'origine sans craindre de basculer dans la clandestinité. Une première étape a été franchie en 2016 avec la création du passeport talent et c'est un franc succès. C'est pour cela que nous soutenons l'idée du gouvernement de simplifier ce titre de séjour pluri-et de l'étendre aux professions médicales enfin et j'en terminerai par là. Nous avons assurément des visions très divergentes sur la politique migratoire, mes chers collègues cependant accordons-nous sur un point, la gestion des flux migratoires relève de la souveraineté nationale mais nécessite dans le même temps un minimum de coopération européenne la présidence française du Conseil de l'Union européenne a obtenu cette année ces avancées essentielles sur le pacte de l'asile de la migraine, l'immigration, des efforts restent à fournir pour boucler les dossiers majeurs, à commencer par la réforme du système de Dublin et la création d'un nouveau mécanisme de solidarité. La France elle est au rendez-vous de la solidarité. Quand elle se mobilisent aux côtés des afghans ont fuyant le régime des talibans. Des Ukrainiens fuyant la guerre ou des migrants secourus en mer. Il est urgent que les États surmontent leurs divergences ne pourront pas nous ne pouvons pas faire l'économie d'un cadre européen commun pour la gestion de la migration et de l'asile. Sans cela, l'Europe

remercie. Et maintenant au président Pierre Laurent.-- Pour le groupe communiste républicain citoyen. Et écologiste. La parole monsieur le président. Monsieur le président, madame, la Première ministre, messieurs les minis chers collègues. Le débat d'aujourd'hui est censé ouvrir celui que nous aurons début 2023 sur un nouveau texte de loi sur l'immigration. Ce sera le 29ème en 40 ans.-- En prélude à ce projet de loi. Vous avez publié le 17 novembre une circulaire mettant gravement en cause le droit inconditionnel à l'hébergement d'urgence pour les étrangers, les structures d'accueil et les associations sont vent debout contre cette circulaire. La discussion commence donc très mal. Si elle partait sur de telles bases. D'autres ex-votre texte de loi pourrait être un nouvel appel d'air à tous les débordements. Tous les fantasmes sur la subversion migratoire sur les assimilation immigration délinquance qui pourrissent le débat public depuis tant d'années l'hystérie soulevée par la l'arrivée de la. Viking. On est le dernier exemple. Pourrions-nous au contraire enfin débattre sérieusement et sereinement. Les migrations sont un enjeu essentiel du monde et de l'époque actuelle. Depuis toujours, la France comme d'autres grandes démocraties s'est construite en accueillant des migrants. Pendant longtemps, c'est cela aussi qui a contribué à faire de la France aux yeux des peuples du monde. La patrie des droits de l'homme mais rompant avec cette histoire au fil des lois régressives. Nous sommes devenus un des pays les plus restrictifs d'Europe car, loin des fantasmes, c'est cela la réalité des chiffres. Nous vivons une grave crise de l'accueil et un traitement de plus de plus en plus dégradant des migrants en France et en Europe. Un traitement indigne des droits humains. Oui il faut débattre car les causes des migrations sont multiples guerres pauvreté extrême violence faites aux femmes, répression des droits humains. Catastrophe climatique jette des millions de femmes, d'hommes et d'enfants sur les routes de l'exil. La mondialisation aussi a changé beaucoup de choses car les habitants de la planète où qu'il vive considèrent que les inégalités mondiales et le 2 poids 2 mesures dans le traitement de la vie humaine ne sont plus acceptables.-- Agissons-nous contre ces inégalités ses insécurité mondiale, bien au contraire. La politique des pays les plus riches comme le nôtre ne cesse de les renforcer. Citons quelques exemples les opérations militaires à répétition qui déstabilisent nombre d'États du sud et du Proche-Orient. Les ajustements structurels et les traités de libre-échange qui laisse exsangue, les services publics de ces pays et assigne leurs économies à l'extraversion contre besoins de développement interne le contrôle monétaire que nous continuons d'exercer sur les pays d'Afrique de l'Ouest, via l'ex-francs CFA qui les empêchent d'avoir les moyens d'un financement de leur développement les atermoiements face à la crise climatique dont témoigne l'échec de la COP27, c'est de tout cela dont nous devrions parler si nous voulons débattent sérieusement des migrations. Mais nous n'allons pas en parler. Et certains nous retirons avec des mots nouveaux, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais à chaque fois que des solutions concrètes sont mises sur la table pour traiter les causes réelles de désordres mondiaux. Et des conséquences qu'elles entraînent toutes ces idées sont balayées d'un revers de main l'arrivée des réfugiés fuyant la guerre en Syrie aurait pu signer une nouvelle prise de conscience en Europe. Angela Merkel avait déclaré courageusement en 2016, nous y arriverons. Ce fut l'échec et le retour des murs et des barbelés en 2021 après la prise de Kaboul par les talibans. Emmanuel Macron ne trouvait plus qu'à s'inquiéter face au risque des flux migratoires irréguliers. L'Europe a tourné le dos à ses devoirs d'accueil et de solidarité humaine. La présidence française de l'UE a passé son tour sur le pacte Asile et immigration. Aujourd'hui, le non respect des clés de répartition solidaire à l'échelle européenne, un temps évoquée, associé à l'absurde au règlement de Dublin génère souffrance et indignité sur le continent. Nous vivons avec la multiplication des camps d'exilés des violences condamnable aux frontières des dizaines de milliers de morts en Méditerranée. Dans la Manche ou sur la route des Balkans. L'Europe n'a plus qu'une obsession, externaliser le traitement des migrants et marchander avec les pays de départ les reconduites aux frontières. Plutôt que de considérer ces états comme des partenaires pour la coopération et le développement. Ces politiques qui n'arrêteront rien tant les causes des migrations sont profondes ne font au contraire que favoriser les compter. On a les contournements et les migrations irrégulières. Quand il faudrait au contraire travailler à des voies légales et sécurisée de migration. Et ces voies légales et sécuriser sont possible car sinon comment expliquer que l'Europe puisse accueillir à juste titre d'ailleurs. Plusieurs millions d'Ukrainiens. Un afghans fuyant les talibans une Nigériane fuyant un mariage forcé ou l'excision un Congolais fuyant les massacres. Une famille du Pakistan fuyant les inondations valent-t-il moins à nos yeux. Mais de toute de tout cela nous ne débattrons probablement pas. Votre projet pour ce que nous en savons puisque nous n'avons pas le texte sans vouloir se concentrer sur 2 sujets présentés comme les 2 faces d'une même pièce, la régularisation par le travail pour les uns l'accélération des expulsions pour les autres, vous nous demandez donc de nous concentrer sur la situation de ceux qui sont déjà entrés sur notre sol. Donc sur ces 2 sujets quelques remarques sur la question du travail. Vous connaissez notre position, elle est claire, nous sommes pour la régularisation de tous ceux qui travaillent. Les grèves de sans-papiers ont montré clairement que des filières entières emploient ces travailleurs sans les déclarer au vu et au su de tous, il n'usurpe le travail de personne car nous peinons aujourd'hui à recruter, il travaille pour notre pays et sont pourtant maintenus dans une situation de vulnérabilité vulnérabilité insupportable. Nous ne voulons pas de quotas et nous serons vigilants sur cette affaire de liste des métiers en tension. Le gouvernement serait prêt donc à accueillir des étrangers mais à une condition leur utilité. Pour nous, il ne doit pas s'agir de régulariser des pratiques d'exploitation patronale. Il doit s'agir de régulariser des femmes et des hommes qui par leur travail peuvent enrichir notre pays et sécuriser leur vie. Nous sommes favorables à la suppression du délai de carence afin de permettre aux demandeurs d'asile de travailler dès les 6 premiers mois en France. Nous plaidons pour les travailleurs pour une régularisation de plein droit non soumises à la durée précaires, des contrats avec un titre de séjour d'une durée minimale de 2 ans pour permettre à ces salariés de sécuriser leur vie et leur installation. Le ministre de l'Intérieur monsieur Évoque aussi ça été rappelé ce soir, l'exigence de réussir un test de français pour l'obtention d'un titre de séjour pluri-annuel évidemment personne ne peut être compte que les étrangers en France et qui viennent travailler chez nous apprennent le français mais nous serons attentifs là aussi pour que ce ne soit pas un sujet de discrimination et d'ailleurs, combien de français aux origines immigrées ont mis des années avant de maîtriser notre langue nationale leur langue d'adoption. Si au contraire le titre que vous envisagiez pour les travailleurs sans-papiers ne se ne courait que pour la stricte durée du contrat de travail ça enfin vaudrait alors OQTF et expulsions. Le cycle infernal seraient perpétrées. Nous nous inquiétons donc de l'abus de vulnérabilité découlant de la dépendance économique et administrateur du travailleur à l'égard de son employeur. Quant au second volet, le renforcement des OQTF que vous présentez faussement comme une contrepartie à l'autre à l'autre. Sujet, le risque est grand. De prendre de plus en plus de largesses avec le respect du droit. Vous voulez qu'une OQTF Val expulsion. On peut aisément supposer qu'une telle décision sera sévèrement réprouvé par la Cour européenne des droits de l'homme car portant atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Du point de vue procédural vous affirmer la volonté de généraliser le juge unique à la Cour nationale du droit d'asile. Vous risquez de déshumaniser les procédures administratives avec un risque de rejet systématique. Cette d'user des amis déshumanisation passera aussi par la généralisation des audiences en vidéo que vous envisagez cet éloignement à sa symbolique car la présence le corps et ses marques la souffrances endurées par les migrants n'est pas perceptible de la même façon dans une procédure menée en présentiel. Voilà en quelques mots, mesdames et messieurs les Ministres madame, la Première ministre dans quel état d'esprit et avec quels principes nous aborderons le débat à venir sur notre projet de loi. Je vous remercie.

Madame, la Première ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues. Faire une loi et ne pas la faire exécuter c'est autoriser la chose qu'on veut défendre. La phrase du cardinal de Richelieu trouve une résonance particulière dans l'actualité récente autour d'un sigle dont aucun Français n'avait entendu parler il y a quelques mois et que tous se connaissent aujourd'hui OQTF. Depuis des années, moins de 20% de ces décisions sont exécutés. Il y a dans d'autres pays, des lois qui déterminent qui peut ou ne peut pas rentrer vivres sur notre territoire. Elles ne sont pas respectées. La situation actuelle est incompréhensible pour les législateurs que nous sommes pour les Français que nous représentons et même pour les étrangers concernés. La France c'est l'une des premières puissances mondiales, elle doit être en mesure de contrôler ses frontières. Depuis longtemps, ce n'est pourtant pas vraiment le cas. Cet état de fait ne date pas d'hier. Les gouvernements se sont succédé et la politique migratoire n'a jamais été jugées satisfaisantes dans notre pays. Ce n'est pas seulement gênant pour notre administration, c'est dangereux pour nos institutions. En n'étant pas en mesure ou en ne souhaitant pas donner un cap clair à cette politique Grimm migratoire. Nous mettons en danger notre démocratie et la cohésion de la nation. De plus en plus de peuple européen, portent au pouvoir des populistes et des extrémistes. Même si ce n'est pas la seule raison. Les considérations migratoires ont joué un grand rôle dans le choix des Britanniques de sortir de l'Union européenne. Si l'Allemagne connaît une montée de l'extrême droite. La crise migratoire de 2015 n'y est pas étrangère, c'est un problème que rencontrent également l'Autriche, la Suède ou l'Italie. Notre pays ne fait pas exception. D'élection en élection progresse une extrême droite auparavant très minoritaires au Parlement. Aujourd'hui, elle représente le 2ème groupe de l'Assemblée nationale. Certains sont parfois tenté de copier ses réponses simplistes Anne espérant que les Français préféreront la copie à l'original. C'est un pari hasardeux au succès très peu probable.-- Entre la porte grand ouverte proposée par une extrême gauche qui refuse de voir que notre pays comme aucun pays d'ailleurs n'a pas les moyens ni économique ni politique d'accueillir le monde entier et la fermeture à double tour réclamé par l'autre côté de l'hémicycle devenu marchand d'angoisse. Nos concitoyens ont le droit de se voir proposer une alternative crédible. Pour cela il faut d'abord dire clairement. Que l'immigration ne doit à aucun prix se faire au détriment de la cohésion de notre nation. C'est à la France qu'il revient de décider d'accueillir ou non des migrants sur son territoire. C'est à nous de fixer les conditions de cet accueil et nous ne devons pas à accepter que l'immigration puisse remettre en cause la façon dont notre société a choisi de vivre. Dans des conditions qui doivent rester contrôler la France accorde à certains étrangers l'asile sur son territoire. Cette procédure. Par sa nature mais aussi pour demeurer soutenable ne peut être qu'exceptionnel, sans la maîtrise des frontières qui permet de choisir d'accueillir ou non des migrants. Notre société risquent de se déliter. Il nous faut, au contraire, trouver une formule qui nous permettent de tirer au mieux parti de l'immigration. Bon nombre de nos entreprises font face à une pénurie de main-d'oeuvre. pour poursuivre leur activité pour conserver leur compétitivité. Beaucoup de nos entrepreneurs recours à l'immigration. L'exemple britannique est édifiant, à cet égard. En choisissant son immigration. La France pourrait sélectionner les compétences dont elle a besoin. Cela permettra à notre économie de maintenir son dynamisme et de pourvoir aux emplois pour lesquels une pénurie de main-d'oeuvre est constatée dans l'ensemble de l'Europe. Par ailleurs le travail éloigne de nous 3 grands mots. L'ennui, le vice et le besoin disait Voltaire. Le travail constitue en effet l'un des meilleurs facteur d'intégration. Cependant les capacités professionnelles seule ne saurait suffire. Il faut établir clairement les termes du contrat. Pour entrer dans notre société les immigrants doivent en accepter les règles en partager les valeurs et un embrasser la culture ce sont eux qui souhaitent nous rejoindre et il demeure libre de choisir où ils veulent aller. Il ne s'agit pas là seulement de protéger notre mode de vie. Ces conditions sont également nécessaires à l'intégration des immigrés par notre société et leur permettront de devenir ainsi des citoyens à part entière pour que cela fonctionne. Nous devons veiller à ce que celles et ceux qui seront entrés en France en respectant ses engagements ne fasse l'objet d'aucune discrimination. Si tous ces prérequis ne sont pas satisfaits. Nos concitoyens continueront d'avoir le sentiment de subir l'immigration et les immigrés ne parviendront pas à se fondre au sein de notre société. Je l'ai déjà dit la problématique migratoire ne concerne pas seulement la France. L'Europe dans son entier par son respect des libertés, son dynamisme économique. Fait figure d'eldorado pour beaucoup de personnes dans le monde. Dans tous les pays de l'Union, la population vieillit, la main-d'Oeuvres se raréfie et dans le même temps la dépendance de nos aînés s'accroît. De nombreux États membres font face aux mêmes défis, il nous faut donc trouver ensemble des solutions qui protège notre mode de vie, à la fois contre ses propres limites, mais aussi contre les ingérences étrangères. À la suite des chantages turc, l'Union européenne a pris conscience de l'impossibilité de continuer à sous- traiter à un pays tiers la gestion de ses frontières extérieures. Les Européens doivent assumer leurs responsabilités. La montée en puissance des moyens de l'agence Frontex doit à cet égard être salué. Au début de l'année prochaine, le gouvernement présentera un nouveau texte sur l'immigration. Vous avez dit monsieur le Ministre, vouloir être méchants avec les méchants et gentils avec les gentils. En d'autres termes vous nous proposez de choisir un peu mieux qui doit venir ou rester dans notre pays et qu'il ne le doit pas nous y sommes favorables. Nous ne feignons pas d'ignorer comme tant d'autres que l'immigration peut constituer une menace pour notre société, si elle est incontrôlée. Cela ne nous empêche pas d'être pleinement conscient qu'elle est à bien des égards nécessaires. Regardant la réalité en face. Nous notons bien la nécessité de faire évoluer une législation qui, par manque d'application a perdu beaucoup de sens. Nous vous soutiendrons donc dans votre démarche, avec une extrême droite en progression croissante et une extrême gauche chaque jour plus irresponsable. Nous sommes tous ensembles contraint de réussir là où nos prédécesseurs échoue depuis 40 ans. Je vous remercie. Merci ma chère collègue. Je vais donner. Maintenant la parole à notre collègue. Maryse Carrère. Pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen.-- Monsieur le président, madame, la Première ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues. Il y a quelques semaines, nous avons pu amorcer cette discussion à l'occasion de l'examen des crédits de la mission asile et immigration. Et la position du groupe RDSE n'a pas changé depuis. La question de la politique d'immigration de notre pays compte parmi les plus difficiles. Elle est sujette aux fantasmes et aux peurs parfois irrationnelles. À la charge d'une. Modéré d'éviter les écueils populiste pour aboutir à une solution équilibrée. Seulement, il existe une autre dérive qui doit attirer la vigilance du législateur et donc aussi du gouvernement, celle de faire une loi juste pour dire qu'on a légiféré. Je sais, Monsieur le Ministre, que vous portez de vraies ambitions, je ne les partage pas toutes. C'est le jeu de la démocratie. Seulement, le Parlement a déjà adopté en septembre 2018, la loi portée par Gérard Collomb pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. C'était il y a 4 ans, autrement dit il n'y a pas si longtemps. Quel est le bilan des mesures de ce texte et qu'en est-il des garanties d'exercices et d'effectivité du droit d'asile qui devait mettre en place. Presque 10 articles étaient consacrés au renforcement de l'efficacité et de la crédibilité de la lutte contre l'immigration irrégulière, qu'en est-il. Ici aussi, qu'en est-il en particulier de la mise en oeuvre des mesures d'éloignement et de modifications qui avait été fait en matière de rétention administrative et je pense en particulier à l'allongement à 90 jours de la durée de la rétention administrative. Avant de légiférer à nouveau il serait légitime que nous puissions analyser la disposition réduisant de 120 à 90 jours le délai pour déposer une demande d'asile à l'échelle de nos départements. Le constat n'est pas ah d'amélioration de l'accueil, ni du traitement des dossiers. Cette mesure était pourtant destiné à réduire les délais de réponse aux situations difficiles. Puisque nous devrions bientôt légiférer cet état des lieux, nous permettrait de savoir où et comment agir efficacement. Alors 2 aspects principaux occupe la question de l'immigration, ces derniers mois l'effectivité des OQTF et la place des travailleurs irréguliers. J'espère néanmoins que d'autres sujets ne seront pas écartées par exemple l'amélioration de l'accompagnement des personnes étrangères les plus vulnérables celles victimes de violences ou bien les mineurs isolés, l'accompagnement des familles également question cher au groupe RDSE. Nous allons beaucoup parler des OQTF. C'est normal c'est normal car il y a manifestement un problème avec ce dispositif si je maintiens à certains chiffres. La France délivre en moyenne 120.000 OQTF par an mais moins de 10% sont exécutés. L'écart entre ces 2 chiffres montrent bien l'absurdité de ce rouage administratif particulièrement pesante timbre pour notre nation que pour ceux qui sont l'objet de ces décisions quasi aléatoire. Tout cela justifie qu'il faille repenser les différents mécanismes qui. Pour les OQTF afin d'en permettre une meilleure application c'est-à-dire plus efficace et plus humaine.-- Derrière cette idée nous défendrons l'idée d'une simplification du contentieux des étrangers. À condition qu'elle leur garantissent un droit effectif à contester les décisions de l'administration en plus d'assurer un meilleur traitement des recours et la bonne administration de la justice. Nous regarderons bien sûr avec vigilance. Ces mesures. Pourquoi pas généraliser les audiences à proximité des centres de rétention administrative ou par moyens audiovisuels pour éviter les déplacements des des retenues. Pourquoi pas aussi créer des pôles territoriaux labellisé pour la gestion du droit d'asile. Mais il ne faut pas que ces dispositifs soient des contraintes pour les personnes migrantes et viennent mettre un déçu en difficulté le respect de leurs droits. Ensuite, nous entendons qu'il faille trouver le moyen de désengorger les préfectures. En effet il est constaté que dans de très nombreux cas, les décisions préfectorales sont simples à annuler devant le juge à raison de mauvaises appréciations par l'administration conduisant à de mauvaises. Décision toutefois ce désengorgement ne pourra consister qu'a délivré moins d'OQTF pour que chaque chacune soit mieux instruite et ainsi juridiquement fondée. La politique du chiffre consistant à prononcer massivement des OQTF se révélant inefficace en pratique. D'une autre manière à la surpopulation des centres de rétention administrative. Montre également les filles l'inefficacité de notre politique de contrôle de limites. Puisqu'elle ne permet pas de répondre au flux qui est imposé. J'espère que nous serons en mesure d'y apporter des solutions concrètes et en ce sens dans les aspects utiles. Il a été annoncé la possibilité de mettre en place un titre de séjour métiers en tension. Notre groupe n'a pas d'a priori de principe sur nos telle mesure mesure bien au contraire. Chacun sait qu'actuellement une part importante de l'immigration irrégulière travaillent sans être déclarés. Ce travail illégal permet d'offrir de la main-d'oeuvre dans des secteurs de métiers en tension. Je pourrais citer de nombreux exemples. Certains ont la chance d'être mis en lumière. Un artisan boulanger pour lequel un village se mobilise ailleurs un apprenti boucher. Ceux-là ont de la chance mais il y en a des milliers d'autres qui travaillent par exemple sur les marchés dans la restauration ou les métiers du bâtiment tout travail pour notre pays, leur métier sont souvent essentiel au quotidien de nos concitoyens. Pour autant, ils sont dans une situation irrégulière cette configuration places ces travailleurs et les employeurs dans une précarité difficile à admettre un poids. Faible rémunération, absence de tout dispositif de sécurité sociale, alors pourquoi pas un titre de jets de séjour spécial comme vous pourriez le proposer Monsieur le Ministre. Mais à la seule condition qu'il puisse être effectif et dans le respect du droit du travail, sans aucune dérogation. Autrement dit d'une part nous n'admettront pas qu'il soit question d'offrir aux entreprises une main-d'oeuvre à bas coût pour certains métiers boudés par les résidents nationaux et d'autre part, il faudra impérativement accompagner le dispositif par des mécanismes de contrôle et des sanctions pour les entreprises qui continueraient de recourir au travail non déclaré. Bref, vous l'aurez compris, ce projet de loi annoncée suscite de la part des élus du groupe RDSE des attentes importantes et nous resterons pleinement mobilisés pour vous accompagner dans l'examen de ce texte. Je vous remercie. vous remercie. Donner la parole à notre collègue Guy Bénard Roche pour le groupe écologiste solidarité et territoires. Merci monsieur le président. Madame, la Première ministre. Mesdames, messieurs les Ministres. Chers collègues, le débat du jour n'est que le prémices de l'étude du 29ème texte depuis 1980 sur ce sujet. La France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien voilà ce que déclarait le président de Bill 19 pourtant rien dans les derniers Budgets présentés ou des les dernières politique annoncée n'est le reflet de cette doctrine. Si mieux accueillir ces procédés dans le budget 2023, une baisse des crédits octroyés pour la location des demandeurs d'asile de plus d'un tiers la discussion risque d'être compliqué, tant le décalage entre les actes et la parole est grand. Je crois ouvrez en même temps sur la politique migratoire aussi disait-il toujours dans ce même entretien. Ce que nous voyons ne me semble être que la jambe droite de cette politique migratoire peut-être parce que c'est celle qui porte réellement ses convictions comment sinon justifier le prisme ultra présent de l'aspect sécuritaire. Comment comprendre qu'un sujet de société important depuis 7 considérés comme réellement prise en charge qu'au travers d'une vision sécuritaire, peut-être aurions-nous aimé voir et nous pencher sur la création d'un véritable ministère dédié à la politique de l'immigration de l'accueil et de l'intégration. Pourquoi ne pas regarder ce débat sous l'aspect humanitaire de fraternité et de solidarité et même de réalisme ou de pragmatisme économique sociale et climatique. Non, je le redis, les questions d'immigration ne peuvent pas se limiter ni même sabordé prioritairement via leur aspect sécuritaire. Le débat d'aujourd'hui devrait, je l'espère permet de recentrer l'immigration phénomène normal historique récurrent qui a participé et participera à la construction de notre pays. Phénomène. Complexe tributaire des guerres des famines conséquence lors du changement climatique. Un phénomène qui conduira encore plus de mouvement dans les années à venir entre les continents et au sein même de l'Europe. En 2017. Le candidat promettait nous examinera les demandes d'asile en mois de 6 mois recours compris c'est nécessaire pour accueillir dignement des réfugiés qui ont droit à la protection de la France. Pourtant, pour les juridictions administratives et pour la CNDA les Costa sur les mêmes une embolisation totale d'Assystem mal calibrée de l'accès aux préfectures et à pour l'obtention de sa nouvelle bande à titre de séjour en passant par l'accès au travail jusqu'à une prise en charge médicale effective. Les parcours des migrants sont trop souvent semé d'embûches. Tout le contraire de profiteurs du système maintenant des milliers de personnes dans la précarité. Et que dire de l'ambition portée de supprimer les protections contre l'éloignement pour motif d'ordre public. Par exemple pour les étrangers résidant en France depuis plus de 10 ans groupe écologiste solidarité et territoires sort clairement en faveur d'une meilleure célérité des procédures mais jamais aux dépens des droits des personnes jamais au dépend des conditions de travail des agents dans le service public jugé plus vite certes mais surtout jugé mieux. Vous avanciez comme objectif l'application de 100% des OQTF.-- Quel est cet affichage politique, quel est le chemin pour y arriver. Quels sont les dispositifs concrets mise en place, le taux n'a été que de 20% de manière assez constante ces dernières décennies. Nous pensons en 30 que la multiplication des craint pour répondre aux difficultés diplomatiques des éloignements est un non-sens et que dire des possibles placement manquera pour des OQTF vieille de 3 ans sans réévaluation de leur situation personnelle ou professionnelle. Il est clair que cela s'accorde bien avec la volonté affichée du ministère de l'Intérieur envers ces étrangers de leur rendre la vie impossible. Je pense aujourd'hui à l'enterrement définitif de la province d'Orléans de 2017 qui avait vu le président déclaré qu'aucun demandeur d'asile de dormir et dehors. Rien de ce qui nous a été présenté ne s'attelle pourtant à ce sujet essentiel à Calais 97% des expulsions des lieux de vie de sort pas suivi de mise à l'abri. C'est d'autant plus inacceptable que les peines encourues pour avoir facilité l'entrée la circulation ou le séjour irrégulier d'étrangers sera augmenté nos inquiétudes sont grandes, à ce sujet pour les volontaires bénévoles des associations. En 2022, le président candidat voulait poursuivent la refonte de l'organisation de l'asile et du droit au séjour pour décider beaucoup plus rapidement. Qui est éligible. La crise ukrainienne a montré que l'Europe, que notre pays pouvait accueillir bien accueilli rapidement accueillir lorsque la volonté politique qui est le dérogatoire. Qui a fait ses preuves de devrait il faut attendre à devenir la règle.-- Aller plus vite si permettent un système de rendez-vous plus efficace en préfecture souvent début d'une succession d'obstacles tels un mur administrative. J'étais déjà eu l'occasion de le dire, les agents sur le terrain ou qu'il se trouve, se retrouvent à difficulté face à une perte de sens de leurs missions et des moyens qui leur sont accordés. Cela débouche aussi sur une insécurité des personnes sans droit sur notre territoire qui devient de la proie des réseaux. Privés de titre de séjour. Les étrangers sont maintenus dans la dépendance d'un accompagnement assuré par des associations, ils ne peuvent pas obtenir de travail déclarées de logement ou, ah bon. Accès aux soins. Nous accueillir plutôt favorablement les prémices de la régularisation à danser des travailleurs exerçant sur notre sol ou la volonté nouvelle de ne plus. Détourner le regard face aux employeurs peu scrupuleux. Rien n'est cependant évoqué pour le parcours vers la nationalité française. Certains de ces travailleurs. Souvent dans des métiers de Première Live pendant la crise du Covid ont bénéficié de ce parcours de reconnaissance vers la nationalité pourtant rien dans le débat actuel ne permet de refonder cet accès à la nationalité pour ces personnes intégrées qu'qui le soit. Pour le reste nous sommes pour le moins circonspect sur la notion de travailleurs des métiers en tension sur notre sol une sorte de version de la notion de travailleurs méritants que vous nous présentez. Derrière ces annonces, il y a un vrai sujet, l'utilité sociale de l'immigré est-elle une assignation à résidence. Comme le disait le président.-- Imaginons une personne accueillie sur notre territoire car travailleurs dans un secteur en tension. Ce secteur est en détention pour des raisons bien particulières. Difficulté de conditions de travail, précarité de l'emploi, salaires insuffisants, ces travailleurs sera-t-il condamné à rester dans ce secteur pour rester en France. Pire, en cas de perte d'emploi bénéficiera-t-il toujours d'à titre de séjour. Cette vision qui pourrait devenir utilitariste très rapidement du travailleur étranger interchangeables nous est particulièrement problématique. Le gouvernement aussi présenté un désir de renforcer les exigences sur la maîtrise du français. Certes c'est normal mais avec quelles modalités d'accompagnement qui seront les évaluateurs qui seront les formateurs. La lutte contre l'immigration irrégulière et la priorité du gouvernement l'axe presque ludique de réflexion de sa politique migratoire. Dont acte. La position de notre groupe est connu de tous. Nous pensons au contraire que la question migratoire ne doit pas ne peut pas se limiter aux prix se veut du travail ou de la sécurité. Les moyens de l'administration doivent d'abord être tourné vers la facilitation de l'accès au séjour et de l'intégration. La criminalisation outrancière de l'étranger contraire à nos valeurs. La modification des procédures judiciaires administratives sous couvert de simplification, quitte à s'éloigner du contradictoire ou de la collégialité et d'autres principes des droits de la défense n'est pas acceptable et, last but not least, comment ne pas aborder votre silence assourdissant sur la problématique des frontières, y compris au sein de l'Union européenne surveiller plus que secourir. Nous l'avons bien vu avec le président Gothard et d'autres de mes collègues, j'ai bien vu la situation à mon Genève par exemple au delà de ne pas secourir beaucoup d'associations, rapporte encore aujourd'hui, le manque d'enregistrement des demandes d'asile. Malgré les appels répétés du Conseil d'État sur la réalité de ce droit. Où est la réflexion à ce sujet et l'ambition du gouvernement sur ces refoulements sauvages illégaux aux frontières notre pays sonore et c'est d'orgueil et d'accueillir et de sauver. Nous devons veiller à une éco-dossier à une inconditionnalité de la dignité dans l'accueil à juste titre car c'est vraiment d'autres odeurs. Je regrette que cette odeur puissent être variable entre l'Aquarius les océans une King.-- L'acceptabilité des refus doit s'ancrer dans le respect des procédures et des personnes. Chers collègues, n'y voyez ni naïveté ni idéalisme utopique mais au contraire, entendez le besoin de bien accueillir, de mieux respecter les demandes des personnes arrivant sur sur notre sol et notre ambition de travail au niveau européen. Donner la parole à notre collègue Esther Benbassa pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun gros. Monsieur le Monsieur le président, madame, la Première ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues. Coincé entre une extrême droite obnubilé par le grand remplacement et une droite en crise. Monsieur le ministre de l'Intérieur et ses amis sont prêts à occulter les vrais problèmes du pays à flatter les bas instincts encourager le rejet et la suspicion. Notre mini-s'enorgueillit d'accorder deux fois moins la ville aux exilés que l'Allemagne et nous promet que tout rejet d'asile vaudra obligation de quitter le territoire donc encore plus d'OQTF et combien d'entre elles seront exécuté. Vous savez que vous n'aurez jamais les moyens de vos ambitions. Cette loi et la 30ème depuis 1980, les gouvernements se succèdent, la rengaine ne change pas l'immigration coûterait un pognon de dingue et les exilés traverserez les ému les maires au péril de leur vie que pour bénéficier de tous les avantages sociaux tels l'aide L'idée est d'ailleurs partagée par la droite sénatoriale, qui a déjà exprimé le souhait dans un bel esprit d'humanité, de réduire de 350 millions, le budget de l'AME dans le PLF 2023. L'étranger à la peau sombre, est un profiteur. Un futur délinquant responsable de tous les maux de la France. Même sous un pont sous une tente d'infortune même privée d'une couverture pour passer l'hiver. Face à lui le bon réfugiés l'Ukrainien par exemple et reçu dignement et tant mieux. Parce que à la peau claire et chrétien on aura désormais le migrant économiquement utile à qui on délivrera cyniquement untethered. Un titre de séjour temporaire métier de en tension pour le lui retirer une fois l'attention passez. Votre politique d'accueil n'est que sinistre replâtrage visant juste à rendre acceptable, ces milliers d'immigrés. Destinées à régler notre crise du recrutement. L'État abandonne à leur sort les étrangers sur son territoire. La situation d'écran est catastrophique. La situation des mineurs non accompagnés aussi la France terre d'accueil.-- Un mythe désormais. Messieurs les Ministres avec cette politique attends prévenir les esprits compte les étrangers et le danger qu'il représente dans 10 ans, y aurait-il encore une place dans ce pays pour des Dupond Moretti ou même pour des Darmanin.--

Va maintenant être trop ministre monsieur Olivier Becht, Ministre délégué en charge du commerce extérieur.-- De l'attractivité. Les Français de l'étranger.-- Monsieur le ministre de la parole.-- Merci beaucoup monsieur le président, madame, la Première ministre, mesdames et messieurs les Ministres mesdames et messieurs les sénateurs. À l'issue de ce débat, permettez-moi de vous donner quelques éléments concernant l'aspect lié à notre politique étrangère. Qui ont été abordés dans ce débat.-- La Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui m'a demandé de la représenter. Aujourd'hui, il a rappelé la semaine dernière devant l'Assemblée nationale. La question migratoire est aujourd'hui à l'élément central dans la conduite de notre politique étrangère à cet égard trois principe nous guide en matière migratoire. Attractivité et organisation des mobilités légal. Solidarité avec les plus vulnérables. Et fermeté face au flux irréguliers. La France souhaite porter une vision équilibrée dans le champ migratoire d'abord nous sommes attachés au développement d'une migration légale bénéfique à notre groupe et nous veillons tout particulièrement. Au renforcement de notre activité à l'égard des étudiants et des talents. Nous avons cette année atteint le chiffre record de 400.000 inscriptions d'étudiants étrangers en France et la délivrance de 12.000 visas dans le cadre des passeports talent. Permettez-moi de vous dire également que notre politique de visas n'est en rien n'arbitraires comme j'ai pu l'entendre. Elle poursuit en revanche un objectif d'attractivité au service de l'influence de notre pays.-- Nous portons également avec force et Constance la défense du droit international et nous nous honorons particulièrement d'être dans le monde. L'un des pays les plus engagés en matière d'asile. Nous sommes attachés à la protection des migrants au respect de leurs droits fondamentaux et comparer non l'année prochaine à la demande du commissariat aux réfugiés. Le Forum mondial des réfugiés. C'est le même souci de la protection des migrants qui nous a conduits à lutter avec force contre les trafics et la traite des être s'humains. En effet et c'est la contrepartie naturelle de l'ouverture et de la générosité de notre pays à nous sommes intransigeants sur le respect de nos lois et de nos valeurs et c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés à lutter avec la même force contre l'immigration irrégulière pour le retour la réadmission et la réintégration dans leur pays d'origine des migrants irréguliers. La France sur la question de grattoirs comme sur bien d'autres questions recherche donc l'équilibre. Nous poursuivons cet objectif avec nos partenaires africains. La stratégie Migration et développement de la France couvre plus de 55 pays majoritairement africains. En 2021, les projets engagés par la France se sont élevées à plus de 1,5 milliards d'euros sur la base de financement conjoint de la France avec d'autres partenaires principalement européens. Nous portons également cette vision équilibrée dans le cadre européen et multilatérale. C'est dans cet esprit que la Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a participé hier à Bruxelles au lancement de deux initiatives dites équipe Europe consacré à de route migratoire. Celle de la Méditerranée centrale est celle de la Méditerranée occidentale, initiée par la France, l'Espagne et l'Italie c'est initiative associe les moyens des institutions européennes et des États membres pour chacune de ces routes migratoires c'est environ un milliard d'euros qui a été investi, et que la mise en place d'instrument qui doivent permettre de resserrer une coopération euro-africaine global dans la lutte contre les filières d'immigration irrégulière dans l'organisation des retours mais aussi sur les causes profondes des migrations irrégulières. La protection des migrants ou encore la migration légale. La France a soutenu fortement l'objectif européen de consacrer 10% des moyens d'intervention extérieure de l'Union pour des projets liés aux migrations et cela représente en tout 10 milliards d'euros sur la période 2021 2027. Nous avons donc un intérêt à nous inscrire dans cette logique coopérative indispensable à une meilleure maîtrise des flux migratoires. Nous devons construire ensemble des partenariats mutuellement bénéfique. Pour nous même, comme pour les pays d'origine. C'est la raison pour laquelle la France a aussi pris la présidence du Forum mondial sur la migration et le développement dont le sommet se tiendra à Paris début 2024. Enfin nous réfléchirons ensemble là en particulier à l'impact du changement climatique sur la mobilité humaine dans une approche transversale et inclusive, à des fins de dialogue et d'anticipation dans un esprit à la fois de solidarité et de responsabilité. C'est bien cet équilibre dans la politique migratoire que nous recherchons également à travers notre politique étrangère je. La parole La parole est à monsieur le ministre du Travail, du plein emploi, de l'insertion. Monsieur Dussopt. Le projet de création d'un d'un type de séjour spécifique pour les métiers en tension puisque. Nous, Monsieur le Sénateur buffet elle a évoqué notamment l'objectif que nous avons avec la création d'un type de séjour par la loi et justement de pouvoir au parlement à avoir un débat sur les critères. D'accès à ce type de séjour. Lorsque l'on pense à une admission exceptionnelle au type de la procédure dite Valls la circulaire dite Valls pardonnez-moi il y a des conditions de présence minimale sur le territoire d'ancienneté sur le territoire régulière ou irrégulière des conditions aussi d'ancienneté dans l'emploi exercé mais il y a l'accompagnement obligatoire de l'entrée du chef d'entreprise qui s'expose au risque d'une du paiement du paiement d'une contribution et le film avec le site que nous proposons, le salarié pourra demander sa régularisation en pouvant. Prouver l'ancienneté. De son emploi, il nous reste à définir. Quel est le bon critère d'ancienneté, tout comme l'ancienneté de sa présence sur le territoire et les critères ainsi définis par la loi seront le principal outil de contrôle de 7 août de cette, de ce nouveau titre pour éviter ce que vous avez dit craindre, c'est-à-dire un outil de régularisation massive, ça ne fera pas la régularisation massive et les critères permettront. De de nous en prémunir ce titre sera un type d'un an renouvelable. Le type n'est pas attaché un emploi. Ça fait quoi un certain nombre de de d'interrogations mais bien l'exercice d'un emploi dans un secteur en tension. La liste des métiers en tension. Plusieurs dizaines de métiers ce qui permet à une personne qui aurait régularisé sa situation par un tel titre et qui perdraient éventuellement son emploi de retrouver un emploi dans un des secteurs en tension, ou de trouver un emploi dans un autre secteur et dans ce cas-là sollicité. La délivrance d'un type de séjour pour motifs économiques pour motif salariés en répondant aux règles fixées par la loi qui existe et et que nous connaissons je je ne partage pas totalement. Par contre, l'inquiétude ou l'objectif du sénateur Bonnecarrere concernant la rémunération. vous avez évoqué, monsieur le sénateur, l'idée de réserver ce titre à des salariés qui seraient re-recruter avec un niveau de rémunération au moins supérieur à la moyenne de la de la branche dans laquelle ils exercent. J'ai de difficultés la première c'est que nous parlons là de régularisation de salariés qui sont présents sur le territoire et salarié depuis plusieurs mois au moins et donc avec un niveau de salaire qui est d'ores et déjà arrêté et. Et par ailleurs, nous savons aussi l'extrême hétérogénéité des situations concernées. Je pense par ailleurs et et je crois que nous pouvons nous retrouver sur ce point qu'il faut veiller à ce que soit pas une trappe à bas salaires et que très très très certainement le maintien dans l'illégalité agit comme une trappe à bas salaires en en maintenant un une situation de dépendance du salarié vis à vis de l'employeur, qui plus est, quand celui-ci peut s'avérer un délicat, mais je pense que nous aurons l'occasion d'en d'en discuter et de débattre de tout cela en, en écho à à la. L'intervention de madame la sénatrice Carrère. Il n'y a pas de volonté là aussi. De, de favoriser les situations de précarité ou de moindre coût pour l'employeur, puisque dès lors qu'il y aurait régularisation dès lors qu'il y aurait volonté d'un d'inscrire la présence du salarié dans le temps, c'est-à-dire avec une carte de séjour fuir annuelle. Il y aurait cette obligation des pour les employeurs de participer à la formation, ce qui implique évidemment qu'ils puissent soit libéré du temps sans participer sur son plan de formation à cette formation et l'apprentissage du français et donc nous cherchons le le bon équilibre pour que ce soit un titre qui sécurisent la situation des employeurs. je n'oublie pas que bien souvent. La situation est est créée par le fait que le contrat a été signé avec un salarié en situation régulière qui n'a pas eu le renouvellement de son titre et l'employeur ne le sait pas nécessairement et sécuriser le travailleur avec cette volonté de sortir. Celles et ceux qui connaissent les situations d'exploitation les plus dramatiques de cette situation de dépendance.-- Merci, monsieur le Ministre. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Les autres Robert la parole. Merci monsieur le le président peut-être pour répondre. Aux différents orateurs. Sur la partie qui me concerne plus directement après les explications de Monsieur le Ministre. Du du travail peut être à Monsieur le Président buffet. Vous avez fait de nombreuses propositions Monsieur le Président. Certaines ne recoupe. Celle que nous proposerons dans le texte de loi que nous allons présenter après ces débats au conseiller. Ça j'ai dit oh oh c'est temps Laurent là a priori sera souhaité que nous attendons la fin des concertations politiques, je crois que nous nous voyons, nous sommes vus, pardon, et nous voyons très prochainement. Le groupe d'ailleurs communiste la semaine nationale mais également les débats sa. Alinéa avant de transmettre le texte au Conseil d'État puis enfin.-- De le présenter en conseil des ministres et donc au Parlement. Nous avons donc un certain nombre de, d'avis convergents. Des sujets aussi que nous n'avons pas repris dans le texte après l'arbitrage. Du président de la réplique et de la Premier Ministre je pense à la question autour de l'aide médicale d'état ou des étrangers malades parce que nous considérons qu'il s'agit là de dispositions que chaque année vous étudiez dans le cas du PLF et du PLFSS, vous le savez mieux personne juste dire peut-être que sur les titres étrangers malades. Si la question évidemment se pose et si je ne retire rien au fait que seule la France le porte-dans ces conditions. Des chiffres qui ont été évoqués la tribune non pas par vous mais par différents orateurs ne sont pas tout à fait juste, il me le permet puisque nous avons fait de réformes du titres étrangers malades notamment. Dans la loi que l'on puisse ensuite dans des dispositions porté par le PLFSS et le PLF et si il y avait bien effectivement 5000 titres. Qui était. Étrangers malades. En 2019 6850. D'ailleurs en 2016, il y en a plus que 3700, c'est-à-dire une baisse de 45% par rapport à l'arrivée du président de la République en 2017 et de 25% par rapport. Aux années pré-Covid. Donc il y a plus que 3700 d'étranger malade essentiellement des étrangers malades ailleurs au titre des personnes qui sont atteints du VIH dans des pays qui connaissent pas, notamment les thérapies sur ce sur ce sujet et je veux dire que de ce que nous avons mis en place et vous le savez, monsieur le président. C'est-à-dire que lorsque nous expulsions d'étrangers notamment un étranger délinquant qui est en en centre de rétention administrative et qui, au titre de sa maladie parce qu'il peut avoir une maladie souhaite faire un appel aux titres étrangers malades humanitaires, on va dire cela comme ça désormais un médecin parfaitement indépendant vient constater évidemment la véracité de la pathologie et constater si dans le pays d'origine. Il a bien. la thérapie pour le faire et nous le faisons. Il y a des pays pour lesquels il n'y a pas de thérapie, donc nous garderons ces personnes conformément à l'engagement de la France, mais dans de très nombreux cas, et de très nombreux cas notamment de pays d'Afrique, il y a c'est c'est ces thérapies nous expulsons quand même la personne donc même si le titre en soit peut être évidemment interrogé comme tous les titres de séjour dans le cas de ce projet de loi. je ne pense pas que ce soit effectivement le débat le même débat qui a qui a 50 ans, je ne reviens pas sur la question de de l'AME. Il y a eu un échange de différences de vues entre les des sénateurs et il ne sera pas dans le, dans le projet de loi comme je l'évoquais puisqu'il est dans les textes financiers peut-être également sur les exécutions des mesures de de d'éloignement alors. C'est sûr que le débat autour des OQTF devient un peu totémique je dirais même un peu un peu un peu slogans. Et ne correspond malheureusement pas tout à fait à la réalité des choses, ce que compte le ministère de l'Intérieur mesdames et messieurs les les sénateurs, et d'ailleurs ce que vous avez mis dans votre. Rapport, me semble-t-il en en 2019 et 2020 c'est le nombre. De. Mesure qui à la connaissance du ministère de l'Intérieur ont été exécutés.-- C'est pas la même chose comme de mesures qui ont été exécutés.-- Je m'explique, ce que nous connaissons, nous c'est les personnes qui ont quitté. Le territoire Schengen. Il est très important de considérer que ces territoires Schengen puisque quand quelqu'un va de France en Belgique alors qu'il a une OQTF, nous ne savons pas je croyais. Exemple de avis de Tourcoing, il y a 17 points de passage avec la Belgique, il y a pas de contre-frontière. À la en Belgique eau quand les gens qui doivent quitter le territoire national vont dans un d'États. Schengen, qui n'est pas. Contrôlée aux frontières. Nous ne savons pas lorsque ces personnes sont partis alors c'est vrai, on y reviendra. Que le, le système entrée sortie Schengen puis Ethias nous permettra de savoir demain, mais aujourd'hui nous ne savons pas. nous ne pouvons nous ne comptons que ce qu'il en soit à départ aider passer par le. Soit une exécution de l'OQTF passer par la police aux frontières du fait de son nez éloignement effectif parce qu'il y a eu un laissez-passer consulaires ou parce qu'il y a un passeport qui permet aux policiers, aux frontières de maître dans un avion et de raccompagner dans son pays, qui respectent les règles de la République et quand ils voient qu'ils ne sont pas bienvenus sur le sol de la République, alors qu'ils ont en OQTF. Moi départ aidés ou un départ. Sur lequel ils ont fait un certain nombre de recours sont parties du territoire national sans jamais passer par la préfecture et par la police aux frontières. Et c'est d'ailleurs non madame la soeur et c'est tout à fait vrai, c'est pour ça que la circulaire que j'ai prise à la lueur des divers faits divers sur lequel je reviendrai pas permet justement de rentrer le nombre de personnes dans les personnes recherchées pour justement que passer à la police aux frontières. Nous connaissons exactement de personnes qui sont partis. Deuxièmement, le nombre d'OQTF que vous citez que nous citons tous où que vous citez, plus particulièrement, je parle des 121.000 qui a été répété ici fin 2021. Ce ne sont pas le nombre de mesures individuelles qui sont prises.-- Ce sont mesures tout court, il y a des personnes qui ont plusieurs mesures individuelles sur elles peuvent déjà on peut avoir plusieurs OQTF voire des OQTF et une interdiction de retour sur le territoire national, tout ça ça engendre les 121 mesures mais quand on compare le nombre de personnes que nous avons. Envoyé dans les pays étrangers et le mot de mesures qu'on a prise évidemment qu'on ne peut pas tomber à 100% puisque, par nature, il y a des personnes qui ont plusieurs mesures et c'est parfois jusqu'à 20%. Des personnes. Ils sont dans les fichiers dite des mesures administratives et puis moi je voudrais vous citer les chiffres puisqu'on, on les cite tous effectivement ça a été rappelé que personne n'avait dépassé 20%. Je dirais même que l'année 2011 2012. Ce que j'ai pris. Monsieur le Président son n'étaient pas des mauvaises années à peu près 85.000 mesures prises à cette époque il y avait je compte en 2011 7970 reconduite et en 2020 12 6204 conduite si je prends l'exemple. De l'année 2021, il y a eu 124.000 mesures tout confondu, c'est-à-dire y compris des gens qui ont plusieurs mesures. Mais en imaginant que ce soit le chiffre sur lequel on on nous correspondons tous ces 16.984 reconduite, c'est-à-dire que nous faisons le plus que le double des reconduites alors qu'il a eu moins de doubler de mesures prises. Donc on a à peu près le même taux d'exécution. Monsieur le président vous et nous. C'est ce que vous avez dit monsieur le président Patriat. C'est vrai que sous le quinquennat du président Hollande ça s'est beaucoup détériorée. si je prends exemple madame de La Gontrie. Si vous me le permettez, ne vous inquiétez pas, je vous réponds monsieur le sénateur de presse c'est pas la réponse, je suis pas sûr qu'elle va vous plaire. 122.000. Je prends je prends l'exemple. Des mesures qui, qui ont été prises par le quinquennat Hollande. On était avec à peu près une 100.000 mesures prises pour 7000 reconduites aux frontières. Bien que là ça c'est effectivement beaucoup détériorée mais je voudrais dire que la meilleure année. Reconduite à la frontière. Malgré les difficultés que nous avons connues en Syrie parce que je ne ferai pas l'affront de dire que le quinquennat du président Sarkozy n'avait pas connu les difficultés que nous connaissons totalement en Libye, en Syrie, en Afghanistan, au Soudan qui a multiplié évidemment les fonds de difficulté diplomatique et c'est juste pour expliquer le le contexte malgré les difficultés. Diplomatiques et des pays en guerre que nous connaissons depuis le début du quinquennat du président. Macron. Je constate que ces 2019 quelle année donc prêts Covid de meilleure réalisation frontière, est-ce que c'est suffisant. La réponse est non, ce que quoiqu'il arrive même 20% ça reste un 5ème seulement des mesures prises et donc effectivement nous devons réinterroger profondément. C'est ce que nous avons dit le système. Des reconduites aux frontières et des OQTF et du placement. Monsieur Bonnecarrere, vous évoquez l'entrée sortie Schengen justement qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire, Monsieur le comte Ethias. La France est prête. La France est prête à faire l'entrée sortie Schengen au conseil des ministre de l'Intérieur je répète sans cesse que nous reposons. La question de pourquoi la commission reporte sans cesse la date d'entrée et cette. Cette entrée sortie Schengen extrêmement importante parce que pour comprendre. Dans quelques instants, de quoi il s'agit tout étranger et même tout citoyen d'ailleurs d'l'espace Schengen va avoir une fiche créer de sa présence sur le territoire européen et de pourront suivent les entrées et les sorties, éviter les doublons de demande. De titre de séjour ou voir. Comment on pourrait s'il se là et tiens c'est très important parce que c'est l'interopérabilité entre les fichiers notamment de toutes les polices européennes de voir d'où vient cet étranger par où il est rentré par où il est ressorti par où il est revenu et nous permettent de lutter contre. Notamment les risques terroristes puisque ça a été lancé, je le rappelle, sous le quinquennat. Précédent, le précédent simplement si la France est le seul à mettre le système en sorties Schengen ça a pas grand chose, ça va rallonger les délais à nos frontières et singulièrement dans les aéroports et dans les ports sans que aucun pays européen ne nous accompagne donc nous disons nous que nous on mettra en place l'entrée sortie Schengen lorsque tout le monde sera prêt le plus rapidement et le mieux, nous aurions déjà dû le mettre en place. Voilà et donc nous sommes tout à fait d'accord en tout cas je peux vous assurer pour suivre ce dossier depuis 2 ans Nissan intérieur que ce n'est pas la France qui a, soit un manque de développement informatique, soit une volonté de ne pas le mettre en place simplement nous n'avons pas le même en train de tous les pays de l'Union européenne et l'ouverture de l'espace Schengen récent. Qui sera confirmé j'imagine par les chefs d'État n'améliore pas les choses et la sortie de nos amis britanniques de l'espace Schengen alors qu'ils étaient. À des pays qui le souhaitaient quand ils étaient membres de espace. Chez. Elle ne va poser un certain nombre de difficultés fortes, notamment pour le port de Douvres et pour notamment. Non mais dans l'espace européen, pardon. En fait, des citoyens de pays tiers et donc créer sans doute un certain nombre de difficultés pour eux d'ailleurs ma main mon homologue britannique me demandant sans cesse qu'on puisse reporter. Évidemment ce. Cette entrée ce sont quoi. Nous ne sommes pas favorables dans un, dans un premier temps en tout cas au niveau du ministère de l'Intérieur. Sur l'examen des valeurs de la République. Nous sommes d'accord, je le dis aussi au président à buffet. Nous avons d'ailleurs des dispositions législatives sur ce point mais on est prêt évidemment améliorer au Maroc en en complément. De l'examen de langue sur le refus d'asile. OQTF. Il s'agit bien de 2 actes administratifs différents dans l'occasion d'en reparler. Avec le Conseil d'État. Mais je pense que c'est pas en allongeant les débats ici qu'on y arrivera, il y a bien sûr un recours

Une chronique ou peut-être même un peu doit. Contre votre propre bilan parce que vous dites il y y a pas assez d'agents dans les préfectures. Bah oui vous avez tout à fait raison, monsieur le comte, 11.000 agents de que vous avez supprimé en 5 ans c'est vous qui les avez supprimé 11.000 la Cour des comptes, tout le monde le dit, nous sommes le 1er, gouvernement.

et depuis que je suis mise intérieur depuis Jean Castex Élisabeth Borne on augmente. Vous n'avez pas suivi la programmation du ministère de l'Intérieur. En tout cas vous l'avez voté en première lecture donc j'en étais fort heureux on augmente le nombre d'agents dans les préfectures. Vous, vous avez supprimé 11 mise post-11.000 postes n'attendez monsieur le sénateur, je vous ai écouté. Voilà avec attention. 11.000 postes, vous avez supprimé après vous nous dites comme le coq de Chanteclerc en pensant. Vous faites lever le soleil dit ben alors c'est c'est terrible ça. Mais les gens sont mal reçus en préfecture. Bah oui parce qu'il y a moins de personnes et vous effectivement si vous n'avez pas supprimer tous ces postes.

vous n'aurez rencontrer plus souvent Bernard Cazeneuve parce que manifestement vous êtes bien éloigné de la politique qui défendait lorsqu'il était en responsabilité au ministère de l'Intérieur et je ne cite même pas Manuel Valls parce que pour vous, j'imagine que ça ça ça devient quelque chose de urticaire mais en tout cas les deux, ministre de l'Intérieur que vous avez eu défendent exactement ce que nous défendons et vous aurez plutôt vous en réjouir sur les contrôles aux frontières, il y a 8 pays. Je rappelle d'ailleurs que dans cinq sociaux-démocrates de vos camarades qui ont mis des contrôles aux frontières effectivement une européenne pourquoi non pas pour des questions migratoires pour des questions de lutte contre le terrorisme et si nous avons rétabli les contrôles aux frontières encore très récemment, c'est justement. Dans le cas de l'atteinte aux 3 chrétien de la basilique de Nice et c'est évidemment personne à ce moment-là et c'est pas en ce jour d'attentats que pour dire le contraire ne pourrait retrouver une autre chose

pensez monsieur le sénateur que désormais il faut pouvoir permettre à tous les étrangers qui sont sur l'île de Mayotte de venir sur le sol réunionnais sur le sol métropolitain, ça se voit que vous êtes pas être extrêmement vend à Mayotte et que vous et vous l'avez pas dit avant. À vos gains Ganbara deux élus ici mahorais. C'est une situation absolument incroyable incroyable qui se passe à Mayotte, chacun en est convaincu et les VISA Balladur portent de il date du 1er Ministre Balladur ça ne rajeunir à personne j'étais même pas en sixième. Monsieur le sénateur, vous faisiez je crois déjà en partie de la politique sur l'asile. Vous dites il y a 2 types d'asile différent a il y a 2 types de sujets la suite d'un côté et il y a l'immigration de l'autre mais quand 70% des demandes d'asile sont négatives. Après la CNDA 70% après la CNDA. C'est bien qu'il y a un petit problème d'orientation, quand même, monsieur le sénateur, chacun sait. Il faut vraiment avoir les yeux. Fermés ou extrêmement naïf pour pas voir qu'il y a d'une part des gens qui méritent absolument l'asile bien évidemment et d'autre part de personnes qui utilisent asile pour rester illégalement sur le territoire de la République, mais chacun le sait, rencontrer les agents de l'Ofpra, ils vous le diront tous les jours sans aucune idéologie et notre travail justement est embêté du fait que les personnes qui doivent avoir l'asile mettent beaucoup trop de temps à l'avoir et donc vivre dans une HLM de paupérisation extrêmement important parce que tout ce qui ne doivent pas avoir l'asile l'utilise comme une voie d'immigration illégale, c'est c'est la vérité première et et d'ailleurs beaucoup de gens l'ont dit et c'est tellement vrai que je vous renvoie au débat parlementaire que portait également Manuel Valls c'est Bernard Cazeneuve. D'ailleurs je veux dire à chacun, ici, quand vous citez qui a eu 30 textes depuis 1982. Je vous rappelle que vous faites tout ce procès de votre votre propre passé, nous avons présenté un seul texte en un quinquennat, donc quand il y a eu textes. En en 40 ans. Je comprends la difficulté ça s'explique d'ailleurs il fait dans la ville et de la jurisprudence qui est complexe des engagements internationaux de la France qu'il faut rétablir ou des phénomènes migratoires qui naissent du fait de la déstabilisation des pays mais ce n'est pas en soi un argument qui est 30 texte

ce que Monsieur Hollande est arrivé aux responsabilités, 208.000. Irrégulier sur le territoire national inscrit à l'AME. On pourrait tout à fait penser, on ne sait pas combien d'irréguliers en France par nature. On peut penser que la émeut c'est quand même la chose la moins contestable puisqu'il faut être irrégulier et on peut penser que quand même beaucoup d'irrégulier. S'inscrivent à l'ANPE puisque c'est effectivement nécessaire pour soigner. Ces étrangers qui peuvent être malade. 315.000 en 2017. Donc on a augmenté de plus de 100.000 irréguliers inscrits à l'AME soit responsabilité. C'est vrai qu'il a augmenté sous le quinquennat du président Macron de 315.000 à 350.000 c'est une augmentation malgré le fait qu'en 2020 et 2021. Nous ne pouvions pas reconduire des étrangers dans leur pays du fait du Covid il y a pas d'espace aérien. C'était plus compliqué de le faire, cette augmentation elle est certes importante et elle mérite d'être régulé Monsieur président de la commission des lois, mais enfin elle n'a rien à voir avec l'augmentation exponentielle que vous avez connu et vous n'avez pas à l'époque fait le courage. courage. Par la Premier ministre et par le ministre du Travail de proposer des régularisations dans une loi puisque vous avez mis en place la circulaire Valls dont je vous rappelle et ça a été dit par le ministre du Travail, c'est 30.000 régularisations 23.000 familial 7000 au nom du travail. Ne donnez pas des leçons de régularisation et d'humanité. Quand vous n'avez pas été capable de le faire lorsque vous étiez aux responsabilités. Je crois qu'il faut qu'on soit un peu plus constructif et un peu plus objectif lorsqu'on parlera de de ce sujet, monsieur le sénateur, si vous le permettez sur la question de madame. Laurent sur le juge unique. Il s'agit pas selon si je peux me permettre. De généraliser le juge unique à la CNDA. Il s'agit de permettre le juge unique à la CNDA. C'est très dur. Laurent et de laisser la CNDA. Le choix de sa formation, soit elle con. C'est-à-dire qu'il s'agit de requérants assez facile soit pour donner l'asile, soit pour le refuser. Je prends l'exemple de nationalité pour lequel on a très peu de toute protection les Ivoiriens par exemple. Il se peut que quelques ivoiriens et l'asile en France. Mais enfin, l'immense majorité de ces niveau rien ne l'est pas, ça pose pas de question de principe. Ça peut être un juge unique, s'il s'agit de questions complexes, l'orientation sexuelle des réfugiés. D'une manière d'un pays qui serait en partition. Je prends l'exemple du Soudan qui est une question extrêmement complexe ou des questions de jurisprudence avant que les talibans n'arrive type jurisprudence Kaboul qui avait pris la CNDA on laisse. Un bon le soin à la Cour de choisir sa formation et de de siéger, soit au collégial soit au juge unique. Il s'agit pas pour le gouvernement de proposer la généralisation Juni qui c'est de laisser le choix, c'est une demande qui est formulée en partie elle même par le Conseil d'État. Par rapport qu'a rendu le président la serre. Donc on peut avoir des différences, évidemment mais je crois que sur ce point et ça, je sais pas si vous me permettez de vous corriger, de la proposition du gouvernement même si j'ai bien compris que vous aviez pas eu n'est pas le texte, qui n'existe pas encore. La généralisation du

il est parti mais de là où il est, il nous entend sans doute. Monsieur Ménard que je veux dire représentant de son groupe politique. On ne peut pas dire que. Ah. Est. Il y a des milliers de places d'hébergement qui soient supprimés. Il y a au contraire des milliers de places d'hébergement libre à Calais et dans toute la Côte d'Opale jeudi devant les élus du secteur, j'en suis hein. Ce qui est vrai c'est que en laissant les migrants en marge dans des jungles ou auprès des passeurs ont fait le jeu quand on leur explique qu'il ne faut pas prendre les hébergements dans toutes les villes du Nord Pas de Calais. On fait le jeu des passeurs qui veulent avoir sous la main pour justement passer de l'autre côté. De la frontière, d'ailleurs je salue la proposition du Garde des Sceaux, parce que dans le texte dont nous n'avons pas dit. Il y a le passage de délit en crime pour les passeurs jusqu'à 20 ans de prison. Je pense que c'est une bonne manière aussi on sera unanime. Je l'espère pour voter ce texte. En tout cas on ne peut pas dire qu'à Calais. L'État ne fait pas son son travail d'hébergement et d'accompagnement, on aurait bien aimé d'ailleurs que beaucoup de personnes nous accompagne à aider les personnes à se faire.

pour les demandeurs d'asile. Ça va être un petit peu compliqué pour vous idéologiquement parce que justement créé on ne leur donne pas l'asile le principe que nous avons utilise. C'est qu'on fait très vite, on leur donne pas l'asile ces trois ans et ils repartent. Voilà donc si si votre proposition de dire on arrête au droit d'asile et on donne une protection temporaire pendant un 2 3 ans. Quelque part je pense que vous serez bien plus à droite que ce que vous dénoncez. Ça me paraît tout à fait, tout à fait contraire à ce que vous essayez de défendre madame madame la sénatrice. Si vous me le permettez et je vais pas répondre à, à vos provocations parce que elles sont elles sont elles sont difficiles et à entendre parce qu'elles étaient insultantes pour une partie d'entre elles. Permettez-moi juste de répondre à la dernière, je ne sais pas pour monsieur Dupond-Moretti. Vous parliez. En me nommant. De mes 2 grands-pères. Alors vous êtes marrant si parce que dit est-ce qu'avec vous, il resterait il serait français, est-ce que vous seriez là. Madame la sénatrice, je j'avais un grand-père puisque vous parlez de ma famille qui est né en Algérie du temps l'Algérie était française. Qui et s'engager dans l'armée coloniale à 14 ans et qui ne savait ni lire ni écrire la France lui a apporté énormément et en 1962, il a choisi la France, il était militaire de carrière et c'était un, un Français de volonté donc oui avec ce gouvernement, les Français de volonté évidemment, on est tout à fait prêt bien évidemment à construire ces belles histoires bon 2ème grand père était juif Maltais n'est né en Tunisie est devenu dans les années 30 pour travailler dans les mines et oui il a voulu travailler ensuite rencontré ma grand-mère et ainsi me voilà voilà pour votre plus grand plaisir. Manifestement il est venu travailler. Hé oui avec le texte que nous proposons ce grand-père qui viendraient travailler dans un métier difficile, hé bien il aurait été régularisés naturalisés et ses du grand-père il avait une grande qualité parce qu'ils aimaient la France était travailleur il n'avait pas de casier judiciaire, donc oui je serai toujours.-- Et donner la parole maintenant. Madame, la Première ministre de Madame, Élisabeth Borne. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, quelques mots en conclusion de ce débat. D'abord pour remercier les oratrices et les orateurs qui ont pris la parole ce soir. Je note que nous avons des différences bien sûr c'est le principe même de la démocratie. Nous avons aussi sans doute des malentendus qui restent à lever.-- Je l'ai dit et les ministres également. Il n'est pas question de régularisation massive. Il n'est pas non plus question de faire croire que c'est par l'immigration que nous allons régler les tensions sur le marché du travail. Mais je crois fermement que pour celles et ceux qui sont sur notre sol depuis longtemps. Participent à la vie économique et sociale de notre pays depuis longtemps et sont enfermés dans la précarité. Nous devons trouver un chemin vers des régularisations ciblé en étant naturellement vigilants à ne pas créer des appels d'air ou à tirer vers le bas les conditions d'emploi. Je suis convaincu que si nous travaillons ensemble de bonne foi nous pourrons trouver des solutions et répondre à des craintes légitimes. Mesdames, et messieurs les sénateurs. J'ai noté dans la plupart des interventions des points de convergence et une volonté de construire ensemble. Nous sommes d'accord, collectivement pour agir aux racines de l'immigration illégale en travaillant avec les pays d'origine et de transit. Et en mettant de très doux au développement, au service de la lutte contre la pauvreté et pour la transition écologique. J'ai noté aussi des convergences sur la question de de procédure et du respect de notre droit, ça n'est pas une surprise puisque nos orientations s'inspire. Reprennent. Pour beaucoup de points. Les conclusions du rapport du président Buffet. Enfin je note aussi un consensus sur la nécessité. D'intégrer mieux notamment par le travail. Ce que nous acceptons sur notre sol. C'est un enjeu essentiel, là encore, nous pourrons avancer ensemble.-- Mesdames, et messieurs les sénateurs. Beaucoup d'entre vous, je l'ai entendu partagent notre volonté d'efficacité et d'équilibre. Dans les mois qui viennent et d'abord au Sénat nous examinerons un projet de loi pour notre politique migratoire. Un projet de loi sur lequel nous pouvons travailler ensemble. J'ai confiance dans notre esprit de responsabilité collective. Je vous remercie. Je vais maintenant mes chers collègues suspende la séance. Elle sera reprise à 21h 35 pour la suite de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie de la santé, du travail des transports et de l'agriculture, la séance est suspendue.